Et vous faire part du décès de nos anciens collègues Claude Saunier, qui fut sénateur des Côtes du Nord puis des Côtes d'Armor, de 1989 à 2008 et Henri Le Breton, qui fut sénateur du Morbihan de 1981. à 2000. Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d'honneur d'une délégation du Sénat roumain. Monsieur Angel-t-il var, président de la commission des affaires européennes du Sénat roumain Monsieur Robert Marius caserne Chuck, vice-président du Sénat roumain Madame en Tchat ragoût, président de la commission des droits de l'homme, il y a été des chances des cultes et des minorités du Sénat Romain et ancienne présidente du Sénat et le monsieur Vlad à pouf ou secrétaire de la commission des affaires européennes du Sénat, la venue de la commission des affaires européennes du Sénat roumain s'inscrit dans un agenda danse entre nos deux chambres puisqu'il y a exactement une semaine, le président Larché recevait la présidente du Sénat, de Roumanie, madame Jean duo. Une brune réunion commune entre les 2 commissions est prévue tout à l'heure pour débattre d'enjeux majeurs : la guerre en Ukraine la crise énergétique, les progrès de la Roumanie vers son entrée dans Schengen, sans oublier, naturellement, la coopération bilatérale entre la Roumanie et la France qui s'inscrit dans le cadre de l'amitié ancienne qui lie nos 2 pays depuis l'émergence de la Roumanie comme État au 19ème siècle, je me félicite que les commissions des Affaires européennes de nos deux chambres entretiennent ainsi un dialogue régulier qui continuent à nourrir cet qui contribuent pardon à nourrir cette amitié presque je tiens donc à souhaiter en votre nom à nos collègues Roumains un séjour fructueux en France.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi. Adopté par l'Assemblée nationale portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi dans la discussion générale, la parole est à monsieur Olivier Dussopt Ministre du Travail du plein emploi et de l'insertion. président, madame la présidente de la commission mais madame et monsieur les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, chère Carole j'ai beaucoup de plaisir et devant vous pour présenter ce ce texte premiers textes relatifs au plein emploi et pourtant un certain nombre de mesures d'urgence pour atteindre cet objectif du plein emploi, il s'agit en effet du 1er, texte qui renvoie à ce bel objectif de plein emploi et ce n'est sans doute pas le dernier texte du quinquennat en la matière, en tout cas c'est le 1er qui nous permet, collectivement, d'examiner un certain nombre de mesures permettant de concourir à cet objectif, il faut le rappeler de depuis 45 ans, la France n'a plus connu le plein emploi et nous ne devons pas nous résigner à cette situation, nous avons même fait un un, une part importante du chemin pour résoudre cette situation est atteinte de cet objectif, nous avons en effet créé la France a en effet créé par son économie sur les 5 dernières années 1,7 millions d'emplois temps comme salarié que comme indépendant et les deux dernières années ont vu quasiment la moitié de ses créations nettes d'emplois, ce qui est à souligner, puisque il y a 2 ans et demi au début de la période du Covid, personne n'aurait imaginé que 830000 emplois soient créés entre mars 2020 et la période qui nous réunit aujourd'hui, c'est réussi : ses résultats et cette réussite en matière de création d'emplois, nous les avons aussi obtenu par de profondes réformes avec une plus grande décentralisation de la négociation collective, avec des moyens plus importants donnée à la formation, je pense notamment au compte personnel de formation au plan d'investissement dans les compétences, je pense aussi bien évidemment au développement de l'apprentissage au cours des dernières années, il faut aussi souligner que tout cela et ses créations d'emploi, cette diminution du taux de chômage ne s'est pas opérer au détriment, soit des salariés sur des entreprises et ainsi je crois que nous avons dépassé une forme de fausses oppositions et peut-être pouvons-nous espérer une nouvelle forme de compromis social qui est en train de se développer ou l'emploi et les compétences deviennent une compléteront une composante essentielle de la compétitivité des entreprises et ne sont plus aborder uniquement au regard de leur coup, ou de leur de l'incertitude qui leur est attaché dans ce contexte, vous est donc proposé aujourd'hui le 1er projet de loi du quinquennat visant atteint le plein emploi, un projet de loi volontairement resserré centré sur les mesures les plus urgentes, mais pas les moins importantes, pourquoi ce texte maintenant pourquoi, dans cette période et pourquoi ces mesures, il faut d'abord là aussi le rappeler, nous avons actuellement un taux de chômage qui est encore le double de celui de nos voisins européens et les tensions de recrutement sont malgré cela à leur comble ce qui est une situation évidemment satisfaisante 60 % des entreprises éprouvent des difficultés à recruter 30 % des entreprises industrielles nous disent être obligé de limiter leur activité, de fermer des lignes de production de renoncer à une partie de leurs carnets de commandes pour des raisons de pénurie de main-d'oeuvre, ces difficultés témoigne des efforts que nous devons encore accomplir pour finir de libérer le travail en France et sans revenir sur les 8 textes de la feuille de route du ministère du travail que j'ai eu l'occasion de présenter devant la commission des affaires sociales, je voudrais simplement développé 3 idées devant la la première et que le plein emploi, c'est d'abord continuer à valoriser le travail, ce qui est un axe central de notre mission, en particulier, il s'agit de donner l'envie, le goût aux jeunes du travail et pour cela, l'entreprise doit être ouverte à l'école, l'école doit continuer de s'ouvrir aux entreprises et avec mon collègue de l'Éducation nationale avec notre ministre déléguée Carole Grangeon, nous souhaitons donner aux jeunes, aux enfants, la connaissance et le goût pour les métiers de l'artisanat de l'industrie des bâtiments, autant de métiers fondamentaux sur lesquels repose une grande part de notre vie économique, ce sont des formidables gisements d'emplois qui progresse sans cesse, ce sont aussi des compétences pointues qui évoluent de manière permanente, très en prise avec les nouvelles technologies et bien souvent à rebours de de leur image qui s'est parfois dégradée avec le temps, à travers l'apprentissage et lycées professionnels ces secteurs connaissent un nouvel élan et nous le développerons encore ces prochaines années, la 2ème idée que je partage avec vous, c'est que le plein emploi, c'est aussi l'emploi pour tous dans la société du plein emploi que nous voulons construire, il faut que nous nous attaquions résolument à tout ce qui freine l'accès à l'emploi des plus fragiles d'entre nous, ce ne sont pas toujours des problèmes de qualification de compétences, ce sont aussi des freins périphériques à l'emploi susceptibles d'enfermer des personnes dans des situations Didine d'inactivité subie de précarité, la garde d'enfant, la mobilité font partie de ces sujets structurels qui reste encore insuffisamment traitées de façon systématique, je suis convaincu que c'est désormais le temps d'avancer sur ces sujets, et c'est d'ailleurs le chantier que nous avons engagé au Tour de France travaille, nous avons un certain nombre d'expériences à valoriser, notamment à travers le service public de l'insertion vers l'emploi à travers le plan d'investissement dans les compétences que nous devons capitaliser pour passer à une nouvelle échelle, je souhaite aussi que les nombreux outils numériques expérimenté ça et là, se déploient pour que les différents acteurs puisse travailler en réseau, d'une façon plus efficace qu'aujourd'hui dans France travail il y a aussi le projet d'accompagner de manière beaucoup plus intensive personnalisée et adaptée, l'ensemble des bénéficiaires du RSA et au-delà les bénéficiaires des minima sociaux, c'est un projet qui me tient particulièrement à coeur : l'État ne peut pas se considérer comme quitte de ses devoirs de solidarité à l'égard des allocataires du RSA juste parce qu'il verse une allocation, nous pouvons faire valoir ses droits ne pouvons faire valoir des devoirs pour les allocataires du RSA mais de toute façon préalables l'État aussi le devoir de leur donner une vraie chance, avec une offre d'insertion, une offre d'accompagnement partout sur le territoire et évidemment adapté personnalisable ne continueront aussi à transformer notre système de formation professionnelle pour accélérer la montée en compétence pour répondre aux besoins des actifs et des entreprises mais aussi pour faire face aux enjeux de transitions numérique écologique et démographique, nous travaillons en ce sens et avec ce projet de loi, nous vous proposons de donner une première impulsion en matière de validation des acquis de l'expérience, mais Carole Granjean ministre délégué reviendra sur ce sujet dans un instant, enfin la 3ème idée que je veux partager avec vous, c'est le fait que le thème emploi ce sont aussi de meilleures conditions de travail, nous avons des conflits, des conditions de travail en France qui sont parfois difficiles, des situations sociales sont parfois conflictuelles et nous savons avoir des marges de progrès en la matière, là aussi pour réseaux des tensions de recrutement, les entreprises devront aussi mieux intégrer mieux valoriser les métiers faire évoluer leurs salariés, nous les accompagnerons pour cela mais nous y veillerons aussi avec attention, car elles n'ont pas qu'un rôle de production mais aussi une part à prendre dans l'effort collectif à mener pour parvenir au plein emploi, le texte que je vous présente aujourd'hui vise donc à apporter un certain nombre de réponses et la première d'entre elles concerne l'assurance chômage, d'abord pour rappeler que cette assurance chômage est au coeur de notre modèle de sécurité sociale et professionnelle qu'elle a été bâtie au fil du temps par les partenaires sociaux pour devenir un outil puissant à la fois au service de la mobilité mais aussi de la protection des actifs au même titre que tous les autres axes que j'ai déjà mentionnée, nous devons la perfectionner pour parvenir au plein emploi, il faut garder son caractère protecteur, garder son universalité, nous avons d'ailleurs élargi son bénéfice à certains démissionnaires et aux travailleurs indépendants, mais il faut la mettre davantage au service d'un retour rapide à l'emploi à l'emploi durable car à nos yeux, nulle, nulle de la tête, condamné à une forme d'une employabilité, il faut aussi le rappeler, l'assurance chômage, nous avons déjà commencé à la réforme en 2000 19 et cette réforme de 2019 visait avant tout à répondre à l'explosion des contrats courts explosion depuis 20 ans, mais aussi à apporter une réponse définitive au déficit structurel de l'assurance chômage, déficit lié en partie justement à la prolifération des contrats courts entre 2009 et 2019, l'assurance chômage ainsi accuser systématiquement un déficit de 2,9 milliards d'euros en moyenne et c'est la raison pour laquelle nous avons apporté de transformation structurelle avec en 1er lieu un nouveau calcul des allocations pour garantir le fait que travailler soit toujours plus rémunérateur que le chômage mais aussi avec la mise en place d'un bonus-malus dans 7 secteurs économiques très utilisateurs de contrats courts et ainsi depuis le 1er septembre 2022, ce sont 6000 entreprises qui ont recours de manière plus importante que la médiane de leur secteur aux contrats courts qui paye une surcotisation chômage malus pouvant aller jusqu'à 1 point de cotisation supplémentaire sur l'ensemble de leur masse salariale et 12000 entreprises qui bénéficient en revanche d'un bonus pouvant aller jusqu'à 1,0 5 % de leur masse salariale j'entends évidemment que des critiques s'élèvent parfois de de Voiron à l'égard du bonus malus et vous avez d'ailleurs relayé ses critiques à travers une réécriture de l'article 2 du projet de loi à de telles qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale je veux cependant à cet égard rappeler quelques faits : les contrats courts coûtent structurellement à l'assurance chômage quelque 2 milliards d'euros par an et c'est pour cette raison que nous avons voulu réattribuer une partie de ce coup aux entreprises qui le faisait peser d'une certaine manière, sur l'ensemble de la communauté contributive et du même coup les responsabiliser le bonus-malus prendra évidemment du temps pour produire tous ses effets, et nous vous demandons de lui donner ce temps pour que les 7 secteurs aujourd'hui concernées en prennent la mesure mais aussi commencent à modifier plus profondément encore, le recours aux contrats courts, il y a de nombreuses alternatives possibles avec des CDI intérimaire des groupements d'employeurs, d'autres formes d'emploi que nous voulons promouvoir et accompagner pour revenir au calendrier d'examen de ce texte et répondre à la question pourquoi agir à nouveau aujourd'hui les les règles actuelles sont définies par le décret du 28 juillet 2019 10 décret de carence venu définir les règles de l'assurance chômage, puisque les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord, ce décret arrive à échéance le 1er novembre prochain et ce qui motive le principe d'urgence de ce projet de loi et le souhait que nous avons de prolonger les règles jusqu'au 31 décembre 2023 pour laisser le temps à la réforme de 2019 2 déployer tous ses effets, nous souhaitons aussi prolonger le bonus malus, jusqu'au 31 août 2024 ouvrir dès aujourd'hui un nouveau cycle de négociations n'aurait pas eu grand sens du fait de la crise sanitaire, les nouvelles règles ne sont entrées en vigueur, qu'il y a moins d'un an et ne paraît donc nécessaire de prendre un peu de temps pour que les partenaires sociaux puissent, à la fin de l'année 2023 se saisir à nouveau de ces questions relatives à l'indemnisation, vous souhaitons donc prolonger les règles, nous souhaitons aussi les nous souhaitons si travailler à les rendent plus réactif à la conjoncture économique, puisque le système telle qu'il existe aujourd'hui et finalement contre-intuitif avec des règles fixes celles existant, le système d'assurance chômage remplit en effet hein parfaitement son rôle, ainsi, sur les 15 dernières années, quand le chômage était supérieure à 10 % 55 % des demandeurs d'emploi étaient indemnisable alors que cette part de demandeurs d'emploi indemnisables est monté à 61 % fin 2019 le ce que le chômage a franchi à la baisse la barre des 8 % c'est le contraire qu'il faudrait observer si nous voulions que notre système soit plus protecteur dans des périodes de difficultés d'emploi, par ailleurs, la France se caractérise toujours par un taux de chômage structurel assez élevés malgré des tensions de recrutement et ce régime actuel de l'assurance chômage reste pensés, construit pour l'essentiel, pour répondre à un contexte de chômage de masse sans être suffisamment incitatifs au retour à l'emploi, cela explique notamment son caractère, pour qui le place parmi les plus généreux d'Europe, notamment pour la question de la durée d'indemnisation ou des seuils d'éligibilité, il est donc nécessaire de renforcer le retour à un emploi rapide lorsque les opportunités d'emploi sont dynamiques et, en revanche, quand il y aura moins d'emplois, il sera nécessaire que ces règles ne viennent plus protectrice, c'est ce principe de contrat cyclicité que nous sommes en train de discuter avec les partenaires sociaux, en précisant que nous sommes ouverts évidemment des aménagements sur les questions de durée d'affiliation sur les questions de durée d'indemnisation, mais une que nous ne souhaitons pas ouvrir une concertation ou une modulation de du montant des indemnisations dans la mesure où le montant des indemnisations, a déjà été modifiée avec la réforme de 2019, nous voulons donc réformer ce système pour qu'qui soit plus incitatif, mais nous ne voulons pas non plus que notre système deviennent aussi stricte que d'autres pays, je rappelle à ce propos, que la durée maximale d'indemnisation et par exemple en Allemagne en Suède de 12 mois dans des pays qui ne se caractérise pourtant pas par un manque de protection sociale, il faut aussi souligner et c'est une chance que nous avons, que le taux de conversion, c'est-à-dire le ratio entre la période de calcul des droits et la durée d'indemnisation et de un pour ce qui concerne notre pays alors qu'il est de 0 virgule cinq en Allemagne, en Italie, en Irlande ou encore de 0 virgule 4 aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal, nous travaillons donc un mécanisme de modulation des règles d'indemnisation en fonction, en fonction de l'état du marché du travail et la concertation ouverte avec les partenaires sociaux devraient durer 6 à 8 semaines pour aboutir d'ici à la fin de l'année, nous avons à répondre à des questions importantes sur les paramètres de modulation, mais aussi sur les indicateurs qui nous permette de rendre compte du cycle économique le plus fidèlement et le plus de la manière la plus réactif qui soit enfin je souhaite souligner mesdames et messieurs les sénateurs, qu'une fois que nous aurons fermé le chapitre de cette concertation autour de la question de la modulation des règles d'indemnisation, nous ouvrirons un nouveau chapitre de discussions avec l'ouverture d'une négociation interprofessionnelle et donc la recherche d'un accord national d'un d'un accord national interprofessionnel majoritaire en matière de gouvernance de l'assurance chômage, ce sera l'occasion de redonner, M. toute sa place au paritarisme en la matière, c'est la raison pour laquelle nous avons limité l'application du texte de loi que nous vous présentons à 14 mois et donc au 31 décembre 2023 je tiens enfin à préciser 2 choses pour terminer la première pour dire que d'autres dispositions du texte concerne la restauration de la définition du collège électoral aux élections professionnelles, pour tenir compte des conséquences d'une question prioritaire de constitutionnalité qu'il y a un article qui permet aussi la ratification d'ordonnances, que le Parlement habilité le gouvernement à prendre et des articles sur la formation professionnelle au sujet desquels Carole Grandjean on reviendra dans une minute, je termine en remerciant l'ensemble des sénatrices et sénateurs qui ont participé aux débats en commission des affaires sociales oh prend au 1er rang desquels les 2 rapporteurs, un certain nombre de dispositions ont été ajoutées au texte votre commission des affaires sociales, en matière de contrats cyclicité de sécurisation juridique de la procédure en matière d'abandon de poste qui sont des dispositions bienvenue et auquel le gouvernement apportera évidemment son soutien, vous le savez madame la rapporteure et monsieur le rapporteur, je suis plus réservé quant aux dispositions visant à sanctionner le refus de CDI ou encore en matière de déplafonnement de la durée maximale des contrats intérimaires et plus encore pour les restrictions apportées au système de bonus malus que votre commission a examiné, mais nous aurons tout le loisir d'en débattre plus longuement à l'occasion de l'examen des articles de ce texte, merci pour votre attention. La parole est La parole est maintenant à Madame Carole Granjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre du Travail du plein emploi et de l'assertion cher Olivier, madame la présidente de la commission des affaires sociales, même de roche madame et monsieur les rapporteurs chers Frédéric cher Olivier dames et messieurs les sénateurs, à la suite du ministre, j'ai le plaisir de vous présenter le projet que porte le gouvernement pour la validation des acquis de l'expérience, qui s'inscrit pleinement dans notre ambition collective de construction d'une société des compétences vers le plein emploi pour y parvenir, tous les outils à notre disposition doivent être mobilisés et René et rénové, lorsque cela est nécessaire, la validation des acquis de l'expérience fait partie de ces dispositifs connu de nombreux de nos concitoyens et pourtant très peu utilisé très peu utilisé au service de leur parcours professionnel, elle a pourtant toute sa place au service de la promotion des transitions et des reconversions professionnelles, elle doit redevenir un outil au service des trajectoires professionnelles de tous les actifs plus attractive, plus simple d'accès, plus moderne et plus valorisante, elle doit s'adapter aux expériences de plus en plus variés, de nos concitoyens, tantôt faite d'engagement associatif de bénévolat, de fonctions syndicales de salariat d'aide familiale parce que les compétences d'aujourd'hui s'acquiert dans de nombreuses situations ne politiques publiques doit s'adapter, c'est tout le sens de ce projet. Les dispositions de l'article IV entendent donc fonder une VAE de nouvelle génération, nous avons tous ici entendu les critiques portées à à la veille VAE d'aujourd'hui trop long, trop administrative, trop complexe, mal adapté à certains profils, un véritable parcours du combattant les Français salariés comme dirigeant d'entreprise ne s'y trompe pas, seulement 30000 parcours réalisé par an l'an dernier, 2 fois moins qu'il y a 10 ans, l'avait et donc source dans d'abandon et de trop nombreuses désillusions et pour cause, la durée moyenne d'un parcours est aujourd'hui de 18 mois au cours desquels le candidat d'A. devra franchir de nombreuses étapes évoluer dans un monde complexe fait de statuer et de financeurs de certificateurs et de référentiels de compétences visées de preuves administratives souvent seuls face à son à son projet, la validation des acquis de l'expérience et pourtant efficace à l'appui de la construction de véritable parcours d'accès à l'emploi pour donner du sens aux carrières de nos concitoyens, c'est pourquoi nous promouvons une approche universaliste de notre action dans une véritable logique de service public pour atteindre les 100000 parcours d'ici à la fin du quinquennat. Les dispositions qui vous sont soumises conduisent donc à lever les freins pour favoriser un plus large accès à la validation des acquis de l'expérience, nous souhaitons en 1er lieu comme vous le savez, permettre un plus large accès à la VAE des proches et dans le gouvernement est pleinement mobilisée pour permettre à celles et ceux qui interrompent leur carrière pour prendre soin d'un proche de faire reconnaître sur le marché du travail, les nouvelles compétences acquises en situation des danses lorsqu'elle relève de gestes professionnels ou de compétences transversales comme les savoir-être. La commission des affaires sociales de votre assemblée a souhaité fixer dans la loi le principe d'un accès universel à la validation des acquis de l'expérience si l'approche paraît évidemment séduisante à première vue, elle porte toutefois le risque déjà par par certaines associations d'aidants familiaux que ce public de soient pas clairement identifiées par le prochain service public ce à quoi le gouvernement veillera de manière très attentive, nous entendons également les craintes des associations, des dents relative à une approche adéquationnisme de la VAE des proches aidants je veux ici rassurer les aidant, comme toutes celles et ceux qui se lanceront dans une procédure de VAE pourront aussi s'il le souhaite, bien sûr, faire reconnaître leurs compétences en vue d'acquérir les des certifications relevant d'autres secteurs. Le texte qui vous est soumis vise également à simplifier la procédure de VAE ainsi que son environnement juridique tout en sécurisant le parcours des candidats, j'ai constaté avec plaisir que la commission des affaires sociales et les rapporteurs ont confirmé l'importance de ce mouvement de simplification en acceptant telles quelles sont les dispositions que nous avons introduites, il est question dans ce texte de simplifier le droit en posant dans la loi les fondamentaux d'une procédure de VAE et en renvoyant à la compétence réglementaire, les détails de mise en oeuvre d'une nouvelle procédure que nous voulons plus simple, plus rapide et surtout moins administratif qu'aujourd'hui cette simplification passe notamment par la possibilité de faire valider par blocs de compétences, la VAE afin qu'elle positionne au coeur les stratégies individuelles vers l'emploi, la VAE doit également maximiser les chances de succès de celles et ceux qui, candidate à une certification via un tel parcours. Le texte que vous allez examiner procède ainsi au doublement du congé VAE pour les salariés, afin de leur donner plus de temps pour préparer leur passage devant le jury, nous savons également que la durée des parcours est une source de réussite et il n'est plus acceptable que les candidats soient contraints d'attendre parfois jusqu'à 8 mois le leur passage devant un jury, c'est pourquoi le texte propose aussi de simplifier les règles relatives à l'organisation et à la composition des jurys. Le texte que nous vous soumettons aujourd'hui est enfin celui qui fera entrer la VAE dans la modernité, c'est une VAE plus digital plus accessible et mieux adapté aux enjeux du numérique que nous vous proposons c'est ainsi dans cette perspective que nous souhaitons créer un véritable service public national de la VAE qui aura la mission de mieux piloter cette politique publique en vue d'optimiser les parcours et donc la réussite des candidats c'est dans cet esprit que nous souhaitons doter la VAE d'un espace stratégique de coordination resserré autour des acteurs compétents car nous sommes convaincus que c'est en combinant les expertises de chaque acteur que nous parviendrons à redorer le blason de la VAE je tiens toutefois à dire que cet espace de coordination n'a de chance de réussir que s'il était à Gilles et adaptable, ce qui implique une gouvernance du groupement d'intérêt public, strictement limitée aux acteurs compétents, faute de quoi nous recréer Riom les conditions d'une politique publique trop complexe à mettre en oeuvre, je salue ainsi l'engagement à nos côtés, des régions qui auront leur rôle, bien sûr, a joué dans la mise en oeuvre de cette VAE moderniser au service des stratégies locales de développement de l'emploi et des compétences. Pour donner une assise à ce service public, le texte propose la création d'un espace numérique dédié pour entrée unique en matière d'information, de promotion et de conseils pour les usagers. Le gouvernement a également entendu la volonté des acteurs de l'accompagnement à la VAE d'expérimenter la possibilité d'une VAE dites inverser son principe rendre concomitant, le processus d'acquisition des compétences par l'emploi et la formation, et celui de la reconnaissance de ces mêmes compétences par la VAE afin de proposer des parcours individualisés d'accès aux certifications dans des métiers en tension de recrutement, elle permettra par exemple de valoriser enfin les contrats de faisant fonction en permettant de faire de ces périodes de véritable tremplin vers la certification et l'emploi durable. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, nous pouvons donner un nouveau souffle à laver avec cette réforme, nous allons mieux reconnaître les compétences de chacune et de chacun et permettre au plus grand nombre de s'émanciper, c'est un véritable progrès social et un grand rebond culturel pour notre pays, je compte donc sur vous, vous toutes et tous pour voter largement cet article et, au-delà, ce texte pour faire du droit à la reconnaissance permanente des compétences un droit réel et tangible : je vous remercie. Monsieur et Madame le Ministre. Monsieur et madame le Ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d'honneur, une délégation du Sénat de Côte d'Ivoire, conduite par son président, son excellence Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio, qui s'est entretenu avec le président Larché, hier soir, la délégation est accompagné à compte panier par notre collègue André Reichert, président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest et nous pouvons saluer je crois la grande qualité de nos relations inter-parlementaire. La Côte d'Ivoire a fait le choix du bicamérisme dans sa Constitution 2016, ce dont nous nous félicitons en 2 en 2020, le président Larché avait participé avec plusieurs de nos collègues au 1er forum du Sénat ivoirien avec les collectivités locales à Yamoussoukro, nos 2 Sénat sont engagés depuis dans une coopération étroite portant notamment sur l'évaluation des politiques publiques et la qualité des travaux législatifs oh là, permettez-moi de saluer l'action du président Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire, un pôle de stabilité dans un environnement régional troublé et ses efforts pour renouer le dialogue politique, cette voix n'est pas nécessairement la plus facile, mais elle est la plus prometteuse. Nos 2 pays sont par ailleurs engagés dans un partenariat étroit qui porte ses fruits dans tous les domaines et singulièrement en matière de sécurité et de défense pour mieux combattre le terrorisme, nous mesurons pleinement l'emploi l'ampleur, pardon, des mesures prises par les autorités ivoiriennes pour protéger les Ivoiriens de ce fléau, monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de salut de souhaiter à son excellence Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio et à sa délégation la plus cordiale bienvenue au Sénat français.

La parole est maintenant à Madame freiner puis ça, rapporteur de la commission des affaires sociales. Merci monsieur le le président monsieur le Ministre, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, l'ambition du projet de loi d'urgence que nous présente le Gouvernement est plus limitée que son intitulé ne le suggère, il s'agit pour l'essentiel, de proroger les règles actuelles du régime d'assurance chômage, ce texte soulève néanmoins des questions cruciales sur les objectifs, la gouvernance et le financement de ce régime, il semble en effet signer l'échec de la réforme de la gouvernance de l'assurance chômage, issues de la loi de 2018 puisque, alors que les règles d'indemnisation du chômage, Cissé par le décret de carence du vingt-six, cesseront d'être applicable à compter du 1er novembre 2022 aucun processus de négociation sorti d'un document de cadrage n'a été engagée pour définir de nouvelles règles afin de donner une base légale et réglementaire de fait à l'indemnisation des demandeurs d'emploi après cette date, l'article 1er autorise le gouvernement à prendre par décret en Conseil d'État, les mesures d'application du régime d'assurance chômage, jusqu'au 31 décembre 2023 ainsi qu'à prolonger l'application du bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage, jusqu'au 31 août 2024 attachée à la gestion paritaire de l'assurance chômage, la Commission considère que ces mesures dérogatoires ne doivent être applicable que pour une durée proportionné à la nécessité de l'urgence, d'autant que cette urgence résulte largement de l'abstention du gouvernement, en conséquence, elle a avancé au 31 août 2000 23 au lieu du 31 décembre la date limite d'application de l'ensemble des mesures qui pourront être prises par décret la période d'application de ce décret devrait Utri pour engager des concertations destinée à faire évoluer la gouvernance de l'assurance chômage, afin de tirer les leçons de l'échec de la réforme de 2018 à cette fin, la Commission a prévu d'abroger les dispositions du code du travail prévoyant la procédure de négociations des accords relatifs au régime d'assurance chômage, sur la base de la lettre de cadrage, elle a également défini une prostituée, une procédure transitoire, inspiré de l'Arctique L 1 du code du travail, faisant intervenir le gouvernement par le biais d'un document d'orientation en vue de la négociation d'un accord, parallèlement à la à cette restauration du paritarisme, la commission a souhaité renforcer à l'article 1er dix ah, ah, le cadre de l'indemnisation du chômage, elle a d'abord proposé que le droit à l'allocation d'assurance ne soit pas ouvert à un demandeur d'emploi ayant refusé 3 propositions de CDI à l'issue d'un CDD, au cours des 12 derniers mois, en outre, elle a jugé indispensable pour pouvoir mettre en oeuvre et mettre en place une indemnisation contracyclique d'inscrire dans le code du travail que les droits à l'allocation chômage peuvent être modulée en fonction d'indicateurs conjoncturels à l'article de la commission entendu modifier les paramètres du bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage en allant bien au-delà du dispositif proposé qui prévoit la transmission aux employeurs des données individuelles servant au calcul de la modulation en effet telle qu'il a été conçu le bonus-malus est inefficace car il ne cible pas réellement les contrats courts, les CDD ne représente que 2 % des fins de contrats prise en compte afin de recentrer ce dispositif sur sa vocation première de lutte contre la permittence, la commission a limité les fins de contrat prise en compte au seul CDD d'une durée inférieure ou égale à un mois à l'exclusion des cas de remplacements de salariés absents, excluant donc du dispositif, les fins de CDI et les fins de mission d'intérim, en outre, afin d'atténuer les effets du bonus malus pour les entreprises concernées, elle a limité la modulation du taux de du taux de 4 0 5 % % à plus ou moins 0 5 point au lieu d'un point, la commission a approuvé l'article 1er dix à insérer par l'Assemblée nationale qui prévoit que le salarié en abandon de poste est présumé avoir démissionné, notamment au regard des règles d'indemnisation du chômage, tout en veillant à présider, il a précisé la procédure applicable, elle a également adopté à l'article 2 bis qui prévoit la réactivation de l'expérimentation des CD, des multi-remplacement est inséré un article de terre qui supprime la durée maximale de 36 mois applicable aux missions d'intérim dans le cas d'un CDI intérimaires enfin la commission a adopté un amendement de notre collègue Philippe Bas, qui prévoit une procédure plus équitable pour les collectivités territoriales auxquelles il est demandé d'indemniser un ancien agent au chômage, monsieur le Ministre, Madame la Ministre, aurez compris notre commission a souhaité redonner l'initiative aux partenaires sociaux et rendre certains dispositifs plus juste et plus adaptée aux besoins des employeurs et des salariés dans un contexte de forte inquiétude mes chers collègues, nous invitons à adopter ce projet de loi modifié par la commission des affaires sociales, je vous remercie.

Frédérique Puissat, rapporteure pour son allant, son sens du collectif et et les dialogues que nous avons eu tout au long de de nos discussions et puis les administrateurs bien sûr les remercie aussi ils ont alimenté nos discussions et donc je pense que nous avons tous les ingrédients pour un bon texte, voilà, chers collègues, en plus des dispositions de l'assurance chômage, présenté par ma collègue rapporteur, ce texte vise également à développer la validation des acquis de l'expérience, la VAE troisième voie d'obtention d'une certification aux côtés de la formation initiale et de la formation continue, la VAE permet de renforcer l'employabilité des personnes concernées, Madame la Ministre a évoqué de favoriser la progression des carrières et de répondre aux besoins du marché du travail, elle permet aussi à ceux qui n'ont pas pu accéder à la formation initiale de faire reconnaître leurs compétences trop complexe, peu connu et insuffisamment valorisées la VAE est aujourd'hui très peu sollicité, on pourrait même dire que c'est une voix qui est parfois mal aimé, comme dit la chanson de Claude François, le recours au dispositif diminue d'ailleurs ces dernières années, le nombre de candidats diminue également à chaque étape du parcours du dossier du dépôt du dossier jusqu'à l'obtention de la certification, j'ai besoin qu'ont même dit la VAE mais personne ne me comprend alors on va essayer de la comprendre l'article IV propose donc de renforcer l'accompagnement des candidats et de faciliter l'accès à l'AVE l'éligibilité des proches aidants hein bien sûr prise en compte des périodes de mise en situation professionnelle, l'accompagnement des candidats dès la constitution de leurs dossiers, le financement du parcours par les associations de transition professionnelle ces différentes évolutions sont les bienvenues, elles ont été substantiellement complété à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement et nous les partageons il est ainsi proposé d'instituer un service public de la VAE dont la mission est d'orienter et d'accompagner tout demandeur d'un groupement public réunira ainsi notamment l'État et les régions, il sera chargé de mettre en oeuvre ce service public au niveau national, il devra favoriser l'information et l'orientation des demandeurs, promouvoir la VAE et contribuer à l'animation et à la cohérence des pratiques sur le territoire, la commission a souhaité s'inscrire dans la logique de cette réforme en complétant le dispositif sur 2 points : d'une part, elle a supprimé la longue liste des catégories de personnes et de type d'activité éligible à la VAE la nécessité d'y ajouter les proches aidants a montré qu'une telle énumération pouvait exclure certaines personnes dont l'expérience peut correspondre à des compétences professionnelles et mérite d'être reconnu, la commission est donc sorti d'une approche par statut en posant le principe selon lequel la VAE est ouverte à toute activité en lien avec la certification visée, cette approche nous semble plus conforme à la logique de la réforme engagée et puis c'est notre cap à l'image du modèle rhénan, le paritarisme comme dit Frédéric mais aussi l'heure aussi du corporatisme de tout corporatisme, d'autre part, la Commission a complété l'émission du GIP, afin que celui-ci prenne mieux en compte les besoins en qualification des territoires suivant cette approche, elle a prévu que le groupement serait présidé par un président de conseil régional, de plus, les ministères certificateurs devront déployer les moyens nécessaires au recrutement et à la mobilisation des jurys, les acteurs de l'accompagnement devront être soutenu, y compris financièrement et les démarches réellement simplifiées, la commission a approuvé l'article 3 qui sécurisent la définition de l'électorat et de l'éligibilité aux élections professionnelles pour tirer les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel, enfin, l'article 5 propose la ratification sans modification de 20 ordonnance portant mesures d'urgence en matière de droit du travail et d'emploi pour faire face à la crise sanitaire, ainsi que d'une ordonnance relative au recouvrement des contributions à la formation professionnelle, cette démarche est suffisamment rare pour être souligné, en effet, le précédent quinquennat était marquée par un Net recul dans la ratification des ordonnances, alors que 78 habilitation à légiférer par ordonnances ont été accordé en moyenne chaque année entre 2017 et 2022, contre une moyenne annuelle de 36 précédemment pour autant sur les 21 donnant qu'il est proposé de ratifier 14 ne sont plus en vigueur et une 15ème, a été annulée par le Conseil d'État, au motif que ces dispositions méconnaissait le Champ de l'habilitation qui avait été donné au gouvernement, a donc considéré qu'il n'était pas utile de ratifier ces 15 ordonnance CQFD. Une telle démarche n'ayant pour résultat que de gonfler artificiellement les statistiques, elle a donc limiter la liste des ratifications au 6 ordonnance dont les dispositions reste en vigueur et donc avec ma collègue, rapporteure, nous vous invitons à adopter le projet de loi issue de nos travaux, je vous remercie. Madame Cathy ah pour et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ont déposé une motion 73 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion, la parole est à madame ah pour ce pays pour la motion. Monsieur le président, madame et monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste a décidé de déposer cette motion tendant au rejet du projet de loi, mesures d'urgence relatifs au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, alors que le gouvernement a décidé de passer en force à l'Assemblée nationale en dégainant le 49 3 sur la loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, ce projet de loi habilite le gouvernement a fixé, seuls les conditions d'indemnisation des privés d'emploi, nous refusons cette remise en cause de la gouvernance de l'assurance chômage par les organisations syndicales et patronales, nous refusons de confier à l'article 1er les pleins pouvoirs au gouvernement jusqu'en décembre 2023, ce passage en force, marque une nouvelle étape du processus d'étatisation de l'assurance chômage largement entamé afin de servir plus directement les intérêts du patronat, l'étape suivante pourrait être la disparition de l'Unédic et de Pôle emploi avec la mise en place de France travaille. Ce projet de loi est une remise en cause du droit du travail au libre choix de son travail à des conditions satisfaisantes de travail et de l'assurance interprofessionnel et solidaire contre le chômage, alors que le Sénat débute l'examen de ce projet de loi, le gouvernement a déjà lancé les concertations avec les organisations patronales et syndicales pour moduler l'indemnité chômage. Ce mépris des parlementaires et d'autant plus inacceptable qui lors de ses réunions de concertation, le ministère du Travail a précisé que la modulation consisterait à allonger la période d'ouverture des droits au chômage, le relèvement de 6 à 8 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir les droits au chômage va priver 200000 personnes d'indemnisation et faire économiser 2 milliards d'euros sur le dos des jeunes qui seront les principales victimes de la modulation cette modulation ne serait donc qu'un moyen pour faire des économies en réduisant le nombre d'allocataires d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales de salariés ont renouvelé leur opposition à cette modulation même l'Union des entreprises de proximité qui n'est pas une officine du Parti communiste, pourtant, mais l'organisation des artisans, des professions. Si on libéral et des commerçants a critiqué, je cite, les doutes, notamment sur la corrélation entre la contrat cyclicité et la capacité à recruter plus facilement, il nous paraît plus important de travailler sur la formation, nous partageons totalement cette analyse les emplois non pourvus dans notre pays ne proviennent pas de la durée d'indemnisation chômage mais du manque d'anticipation et d'investissement dans la formation professionnelle si nous manquons d'ouvriers qualifiés dans l'industrie d'artisans dans le bâtiment de techniciens dans les services, c'est non seulement parce que les salaires sont trop faibles et les conditions de travail très difficiles mais encore parce que depuis des années, les gouvernements successifs ont cassé l'enseignement professionnel, la logique du gouvernement selon laquelle il faudrait réduire les droits au chômage pour inciter à la reprise du travail relève d'une vision archaïque de l'emploi le 14 juillet 2022 lorsque le président de la République a annoncé cette réforme, il a présenté l'assurance chômage comme un obstacle au bon fonctionnement du marché du travail, les parlementaires communistes sont particulièrement attachés à l'émancipation des individus dans leur travail, mais cette émancipation n'est pas possible dans la société capitaliste qui grignotent toujours davantage la vie personnelle au profit de la vie professionnelle, la dégradation des conditions de travail, les faibles salaires, les comportements toxiques qui a parfois des DRH conduise à un mal-être au travail et à une perte de sens si les infirmières démissionne, démissionne de l'hôpital, c'est justement parce qu'elle se plaignent d'une perte de sens et qu'elle ne supporte plus de trier les patients et de les laisser attendre des heures, l'émancipation par le travail est possible dès lors que les salariés participent aux décisions de l'entreprise avec une réduction du temps. Travail à 32 heures et avec une augmentation massive des salaires en attendant, nous refusons d'opposer les travailleurs avec les privés d'emploi les travailleurs et les les privés d'emploi sont de plus en plus dessaisi de leur droit à choisir librement un emploi en cohérence avec leur qualification ou leur formation, ils deviennent des variables d'ajuster. Seulement du marché du travail alors que moins de 4 chômeurs sur 10 perçoivent une allocation, et que la moitié d'entre eux, et sous le seuil de pauvreté, la réforme de l'assurance-chômage de 2019 a fait perdre 155 euros par mois à un 1000000 d'allocataires, elle a exclu 450000 paires. De toute allocation et à frapper les plus fragiles et notamment nos plus jeunes, cette baisse des droits s'est accompagné d'un Nevis évincement des privés d'emploi, l'allocation chômage ainsi en un an, les radiations administratives ont progressé de 40 avec ce projet de loi, le gouvernement reprend la main. Sur l'Unédic, qui depuis 1958 était géré conjointement par les organisations syndicales et patronales, plutôt que de s'engager à reprendre les 15 milliards de dette de l'Unédic générée par le recours à l'activité partielle durant la crise sanitaire, l'État veut transformer par décret, l'assurance chômage en simple filet de secours minimum cette réforme de l'assurance chômage est un déni de solidarité au-delà de la diminution des indemnités des plus précaires, le gouvernement veut transformer une assurance collective en épargne individualisé cette dénaturation de l'assurance chômage est un processus à l'oeuvre depuis plusieurs années et notamment depuis la substitution en 2018 de la CSG aux cotisations salariales et l'encadrement des négociations par le gouvernement, l'attaque contre les droits les plus des plus précaires cache des enjeux plus structurelle, où le chômage ne sera plus qu'à risque individuel, il est urgent de renouer avec la logique de solidarité salariale interprofessionnelle garantissant chacun contre le risque social du chômage entre 1992 et 2001 la dégressivité des allocations chômage n'a pas entraîné d'accélération de la reprise de l'emploi, de la même manière, les restrictions d'accès au droit des intermittents du spectacle et le doublement de leur taux de cotisation n'ont pas augmenté le nombre de CDI dans le secteur, en réalité, les chômeurs n'ont pas le choix de leur emploi et la restriction de l'accès aux indemnités chômage. Risque de les contraindre à accepter des contrats encore plus précaire contraindre à accepter des camps des contrats encore plus précaire la droite et le gouvernement semble d'accord sur de nombreux points sur ce texte et ma collègue Laurence Cohen, il reviendra dans son intervention, mais je tiens à dénoncer la suppression de l'indemnisation chômage pour les salariés qui abandonnent leur poste malgré les tentatives ne nos rapporteur de consolider le dispositif juridique la présomption de démission d'un abandon de poste est un recul considérable, le phénomène d'abandon de poste n'étant ni chiffré ni évaluer, il est largement précipité de légiférer dessus, d'autant qu'avec cette rédaction vous allez accentuer les risques juridiques nos juridictions prud'homales sont dans l'incapacité actuellement de répondre dans un délai d'un mois à une demande des salariés surtout c'est négliger le fait que l'abandon de poste est avant tout une porte de sortie en cas de conflit avec l'employeur, la création d'une présomption de démission va priver les salariés de toute indemnisation chômage et entraîner une explosion des arrêts maladie face au projet régressif du gouvernement, nous portons un projet alternatif d'une sécurité d'emploi et de formation pour sécuriser les parcours de vie en conclusion les sénatrices et sénateurs du groupe communiste serait Citoyen et écologiste rejettent ce projet de loi qui s'attaquent aux droits des salariés et à la gouvernance paritaire de l'assurance chômage pour toutes ces raisons, nous avons déposé cette motion tendant à opposer la question préalable que nous vous invitons à soutenir, je vous remercie. Que l'avis de la commission, monsieur le rapporteur sur cette question préalable. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, chers collègues, par principe. Je ne suis jamais favorable aux questions préalables et je pense que c'est souvent l'opinion du du Sénat parce que ça revient à à refuser de de débattre et débattre, discuter, c'est en quelque sorte ce que nous sommes, et donc une question préalable, c'est une forme de de négation de ce que nous sommes et puis il y a des arguments qui sont des arguments juridiques parce qu'il faut bien prolonger la convention de l'assurance chômage, sous peine de mettre en risque les les assurés et puis il y a de nombreux arguments politiques, ils ont été y a question du du taux d'emploi dans notre pays, hein, qui est une vraie question pour créer des richesses mais aussi pour financer notre il y a la question de la VAE hein les aidants et les proches aidants qui attendent, cher à Jocelyne Guidez qui attendent pour valoriser les acquis de de l'expérience la question des des contrats courts, qui sont nombreux dans notre pays et qui coûte 9 milliards à la totalité des des assurés, hein, des assurés sociaux, il y a la question de la gouvernance grosse question, hein, de l'assurance chômage, la place du paritarisme, donc vous voyez toutes des questions qui doivent être débattus ici et qu'il n'y aurait pas de sens de s'en exonérer alors c'est pas parce que le le match est difficile, on peut trouver le match et difficile, délicat, mais je crois que même dans ces cas-là, il faut pouvoir jouer le match et savoir jouer le match et donc je vous invite donc à rejeter cette question préalable et aborder le plus vite possible nos débats, merci à toutes et à tous. j'entends et je suis en tout cas je peux entend un certain nombre d'arguments qui font d'une opposition au texte sur des principes. ça a été rappelé par contre dans l'exposé de Madame la sénatrice, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites et et qui ne correspondent pas à ce que nous voulons faire, ni même pour une un événement particulier à à la réalité, vous dites, madame la sénatrice que France travail aurait comme objectif de faire disparaître, pôle emploi, ça n'est pas le cas et j'ai eu l'occasion de le dire devant la commission des affaires sociales de cette assemblée comme de l'Assemblée nationale, nous travaillons à une meilleure coordination mais en aucun cas la disparition de de Pôle emploi vous présenter comme acté le fait que la modulation amènerait à exiger six mois de cotisation sur les bancs huit mois pardon de travail sur les 24 derniers mois plutôt que 6, comme c'est le cas actuellement rien de tel n'est acté et si je ne veux pas préjuger des résultats de la concertation avec les partenaires sociaux, je peux d'ores et déjà vous dire qu'à titre personnel, si nous devons modifier les conditions d'affiliation, je préférerais et j'emploie volontairement cette formule que nous modifions la période de référence plutôt que la période parce que souvent l'entrée dans le marché du travail se fait sur la base d'un CDD de 6 mois et les CDD de six mois sont plus nombreux que les CD de 17 au ou huit mois, vous dites aussi que cette réforme a pour objectif de baisser le montant des indemnités, c'est faux, je l'ai dit, c'est précisé dans le document de concertation adressée aux partenaires sociaux la réforme de 2019 par la modification du hier à ramener le niveau de taux de remplacement de l'allocation chômage en France dans la moyenne européenne, c'est-à-dire 57 nous ne souhaitons pas le le modifier, enfin vous avez présenté le nombre de radiations administratives, comme il y a augmenté de 50 % en 2022 lorsqu'on regarde nombre de radiations administratives entre janvier et août 2022 par rapport à la période de janvier à août 2 1000 19 et en application des objectifs de de contrôle à la fois de contrôle de recherche d'emploi, mais aussi de qualité administrative des des fichiers, cette augmentation est de 14 %, nous sommes loin des 50 que vous avez évoqué donc pour toutes ces raisons, la vie est évidemment défavorable. en explications de vote sur la question préalable, j'ai d'abord Madame Rossignol la présidente Rossignol. Merci monsieur le président, le plus souvent mon groupe s'abstient sur les propositions de questions préalables s'abstient par amitié avec le groupe CRCE que rarement mais ne votent pas pour parce que le plus souvent nous pensons effectivement qu'il y a lieu à débattre et comme nous sommes des irréductibles optimistes, nous espérons même améliorer les textes à l'issue de ces débats, j'ai trouvé notre collègue Katia pour opposer extrêmement convaincante, d'autant que, on peut se poser la question de savoir s'il y a vraiment lieu à débattre sur ce texte, de quoi allons-nous débattre de vous représentation du chômage, des présomptions qui pèsent sur les chômeurs de l'idée selon laquelle, si les gens sont au chômage, c'est parce qu'ils le veulent bien, et qu'il suffirait de réduire l'accès à l'indemnisation pour qu'ils retrouvent. La voix de l'emploi, voilà de quoi nous allons discuter nos chances d'améliorer steaks sont à peu près nul puisque le gouvernement va trouver avec la majorité de droite du sénat beaucoup de points de convergences sur toutes ces analyses que vous partagez les uns et les autres, donc en l'espèce ce texte si voulez résumer, en fait, c'est la traduction législative et quand je dis je suis presque déjà pas tout à fait dans la vérité, parce que c'est la traduction d'un débat devant le parlement d'un texte qui est déjà en discussion devant les partenaires sociaux et de décisions qui finiront qui seront à la fin, prise par voie réglementaire, donc c'est à peine législatif, donc en fait, c'est la mise en oeuvre de la fameuse formule présidentielle, celle qui disait : il n'y a qu'à traverser la rue et du trash du travail, je vous en trouve comme je ne partage pas cette formule, nous voterons la question préalable. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame, monsieur le rapporteur, madame la présidente, hein, mes chers collègues, donc si vous voulez dans ce projet de loi, je n'ai rien vu de quelque 2 choses qui sont péjoratif pour les salariés d'abord si vous voulez, il est nécessaire que les règles d'indemnisation du chômage, ben, qu'ils soient poursuivis, puisqu'elle ça serait le 1er novembre il est bien sûr nécessaire que les partenaires sociaux participent avec le gouvernement sur les lois l'indemnité chômage, je pense que le gouvernement a tout tout loisir pour le faire et même bien sûr l'améliorer en ce qui concerne les autres. Trop d'emplois, elles sont importantes actuellement et ce qu'on fait 3 propositions de CDI après un CDD bon 3 propositions quand même c'est pas être contre la peine le bonus malus est amélioré et alors tout à l'heure, vous avez dit : si vous voulez, l'abandon de poste, il faut, il faudrait absolument pas revenir sur ce qui ce qui a été dit à l'au niveau de la commission, c'est vrai que pour moi, un abandon de poste ne doit pas être considérée et indemnisé comme un salarié licencié ou une rupture conventionnelle, ce n'est pas, ce n'est pas ça en fait, il le le salarié doit avoir les droits absolument,

elle doit répondre au marché du travail doit être valorisé, notamment pour les emplois à domicile et les emplois en pas d'où, dans le secteur médico-sociaux et c'est quelque chose qui va très important pour valoriser ces personnes qui en ont besoin, merci.

un affront au débat parlementaire et au paritarisme, nous sommes sommés donc de prolonger une réforme antisociale qui depuis l'étude d'impact alarmante de l'Unédic n'a pas été évalué tout cela pour permettre au gouvernement, en fait, c'est ça la véritable raison début 2023 de légiférer par décret lorsque les négociations avec les partenaires sociaux auront échoué car enfin, comment croire qu'ils pourront accepter une réforme qui prend comme modèle le système canadien qui a multiplié les radiations fait chuter le nombre d'allocataires, mais pas le Hal au chômage et approfondie, précarité et paupérisation des demandeurs d'emploi, votre gouvernement prend le problème à l'envers en ciblant essentiellement les demandeurs d'emploi en reportant sur eux la responsabilité de leur situation en fantasmant la figure d'un chômeur qu'il qu'on vient d'activer et qui profiteraient des prestations, vous faites l'économie de réflexion structurelle sur la qualité des offres d'emploi sur le marché du travail sur la nécessité de changer de travail et sur le nombre réel d'offres non pourvues qui tourne d'année en année autour de 6 % des offres sans compter que le texte, c'est un texte redessiné en commission en l'aggravant donc quand la réforme, vous avez un bonus malus qui est neutre : quand la réforme perd pèse essentiellement et pour des milliards sur les économies sur les chômeurs aussi, nous partageons le constat du groupe communiste et nous nous joignons à leur demande de Roger. bien entendu, nous avons pas du tout le le même point de vue que l'oratrice précédente puisque nous vivons dans nos territoires en permanence à la rencontre de chez entreprises de PME d'artisans qui nous explique au jeu des difficultés de recrutement pour trouver du personnel, des difficultés pour conserver, même le personnel avec aujourd'hui parfois des entreprises qui doivent modifier leur stratégie voire même ne peuvent même plus développer ou s'implanter dans les territoires, alors c'est pas vrai, sur la totalité de la France, il faut avoir une analyse qui soit plus précise, mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est un c'est une démarche généralisée en parallèle, nous voyons bien, de façon, alors on peut discuter du chiffre mais le nombre d'emplois dont pourvu est en augmentation, je crois qu'on doit à la fois regarder de très près cette réforme qui n'est pas seul nécessaire suffisante puisqu'il faut en parallèle travailler sur l'accompagnement voilà donc nous vous êtes nous avons plutôt un regard bienveillant sur ce texte,

qui a été vigilante, notamment dans le renfort de du paritarisme puisque nous sommes extrêmement vigilants sur cette démarche-là, nous savons que ça fonctionne, et donc là dessus, nous avons quelques points différence que le gouvernement, mais la commission a su corriger cette ces points divergence et donc, au regard de tout cela, nous voterons compte cette motion de censure.

entraînerait le rejet du texte en discussion. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 l'avis de la commission est défavorable celui le gouvernement également. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Donc, le scrutin Donc, le scrutin est clos. Il résultat votants 344 344 pour la motion 92 contre 252 la motion n'est donc pas adoptée et nous passons à la discussion générale. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Cohen pour le groupe CRCE. Et pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans la continuité de la motion présentée par ma collègue Katia pour je souhaite dénoncer la philosophie qui justifie ce projet de loi, à savoir que les chômeuses et les chômeurs ne voudrait pas traverser la rue pour trouver un emploi, vous considérez les privés d'emploi comme des fainéants et des profiteurs, alors même qu'un tiers d'entre elles et eux ne font pas valoir leurs droits, le chômage est source de souffrance, de mal-être et entraîne le plus souvent une perte de confiance en soi, ce que vous refusez obstinément de prendre en compte, faut-il rappeler ici que l'assurance chômage était un droit, les difficultés de recrutement invoqué par les entreprises ne justifie pas une remise en cause globale des droits de l'ensemble des salariés, ce n'est pas en modulant les indemnités chômage que vous allez trouver des électriciens, des couvreurs ou des aides à domicile pour y parvenir, il faut investir dans la formation professionnelle et améliorer l'attractivité des métiers notamment en revalorisant les salaires et en améliorant les conditions de travail, l'article 1er suspend la gouvernance paritaire du régime d'assurance chômage au profit du gouvernement qui pourra décider seul de moduler l'indemnisation chômage, la modulation de cette indemnisation selon la conjoncture et les territoires va entraîner une fracture géographique et une disparité temporel entre les droits au chômage au chômage ainsi les droits au chômage seront différents selon le lieu et la date à laquelle la locataire voudra y prétendre : la modulation est une remise en cause du principe d'égalité, le gouvernement peut donc remercier la majorité de droite au Sénat, jamais avare d'un recul social supplémentaire qui a inscrit dans le texte, le principe de contrat cyclicité comme la la niche, le journal Les Échos du 20 octobre les sénateurs LR ont-ils sauvé la mise à la réforme de l'assurance chômage, ils ont ajouté un article au projet de loi pour que les paramètres liés à l'ouverture des droits à la location et à la durée d'indemnisation puisse évoluer en fonction d'indicateurs conjoncturels sur le marché du travail, ce recul s'ajoute au vote de l'Assemblée nationale, sous pression du MEDEF et du groupe LR sur la présomption de démission pour les abandons de poste que le rapporteur de notre commission ont tenté d'encadrer sans s'attaquer aux problèmes de fond, en effet, en l'absence de données statistiques et d'études sur les abandons de poste en France, cette disposition repose sur une instrumentalisation de l'abandon de poste mais surtout créerait une procédure déséquilibré pour les salariés, totalement inadapté à la réaliser réalité de la justice prud'homale, non contente de régression ce projet gouvernemental, la droite sénatoriale a ajouté un article qui supprime l'indemnisation chômage des salariés en CDD, en cas de refus à 3 reprises d'un cours d'un contrat à durée indéterminée, autrement dit il faudrait accepter n'importe quoi, quelles que soient les conditions de travail, le trajet où les salaires proposés cette remise en cause des droits à l'assurance chômage n'est pas acceptable d'autant que ce sont les mêmes qui ont favorisé hier le développement des CDD et refuser l'augmentation des salaires qui souhaitent aujourd'hui pénaliser les salariés de la même manière, la majorité de droite de notre haute assemblée veut favoriser le recours à l'intérim, alors que ces contrats pèse lourdement dans le déséquilibre du financement du système et participe à la précarité dans notre pays, enfin, la droite a tué le dispositif de bonus-malus du gouvernement en limitant le malus, de sorte qu'il a quasiment disparu face au projet du gouvernement et de la droite sénatoriale, nous portons un projet alternatif qui passe par de nouveaux moyens de financement une lutte effective contre la précarité et les licenciements pour les salariés, il est indispensable de rétablir les cotisations sociales à l'assurance chômage en supprimant en contrepartie la CSG pour les salariés, il est indispensable de financer un service public unifié de l'emploi et de la formation professionnelle pour les privés d'emploi, il faut mettre en place une véritable sécurité sociale professionnelle qui repose sur l'universalité de l'ensemble des salariés afin d'acquérir des droits individuels entièrement transférables garantissant un montant d'indemnisation chômage sur 24 mois, bref un projet aux antipodes de celui proposé par la par le gouvernement et la majorité sénatoriale, autant de raisons pour lesquelles les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain citoyen écologiste voteront contre ce projet de loi, je vous remercie. La parole est à présent Monsieur Jean-Marie Vanlerenberghe pour le groupe centriste. Monsieur le Président, c'est le ministre, Madame la Ministre, mais j'espère la revoir madame et monsieur les rapporteurs chers Frédéric cher Olivier, bravo pour votre excellent travail avec la Commission et mes chers collègues, nous connaissons tous près de chez nous, un patron qui embauche mais ne trouve pas de personnel, nous entendons aussi tous les cancans contre le beau-frère de la copine du voisin qui profitent du chômage, voire du RSA et qui gagne plus que celui qui travaille. Ces faits existe, bien entendu, mais pensez-vous honnêtement que la vendeuse de chez Camaïeu, qui vient de perdre son travail pourra demain être serveuse chez Raoul le resto route question de profil, bien sûr, de salaire, peut-être, mais aussi de conditions de travail, vous l'avez évoqué, monsieur le ministre, de transport, de garde d'enfants, de formation, alors Monsieur le Ministre. Que faire. Plus qu'un objectif ou l'intitulé d'un texte ministériel je pense comme vous que le plein emploi est une réalité concevable et même atteignable, le travail est un droit, rappelons-le, voire institutionnel, le devoir de l'État et donc de donner à chacun et chacune, les moyens d'y accéder, mais quel chantier, le texte n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions, en réalité, il répond à l'urgence normative du régime d'assurance chômage plus qu'à cette urgence du plein emploi certes son adoption permettra de sécuriser l'indemnisation des demandeurs d'emploi, passé le 1er Legrand et aussi d'offrir un délai pour engager les concertations nécessaires. Mais ce délai doit surtout nous permettre d'engager le vrai chantier de l'assurance chômage, sa gouvernance. Sans réforme globale et profonde, le paritarisme aura vécu et vous y connaissait pourtant mon attachement comme celui de la commission et celui de notre groupe. Je crois sincèrement dans la capacité des partenaires sociaux à s'illustrer ailleurs que sur les dépôts pétroliers ou dans la rue. Il leur revient de trouver des solutions pour équilibrer les comptes, sinon l'État reprendra la main, nous pourrons le déplorer, il sera difficile de s'en étonner. Mais sur ce point, le texte en réalité n'est qu'une petite partie de la solution pour le plein emploi pour y prétendent nous devons changer de paradigme et c'est là qu'on attend France travaille. Je vous en conjure, Monsieur le Ministre, pas d'usine à gaz : pas de super structure miracle, pas de révolution, pas de fusion de tous les acteurs de l'emploi au fond. Nos attentes sont simples : ce sont celles des demandeurs d'emploi, un guichet unique, un accompagnateur unique et un parcours personnalisé jusqu'à l'entreprise, en passant par la case formation s'il le faut. Sans ça, sans cette capacité à mettre enfin sous le même toit avec un coordonnateur, la formation, l'insertion sociale et le recrutement économique, pas de plein emploi, les exemples sont nombreux : la Maison de l'emploi de l'entreprise, la formation de Vitré, m'apparaît comme la plus aboutie, la Maison des chômeurs d'Arras devenue Maison de l'emploi et des métiers en est un autre imparfait, certes, mais loin d'être isolé, je pourrais citer aussi Calais Saint-Quentin Bonneville et bien d'autres que je connais, voilà cet engagement suppose de ne plus fonctionner en vase clos de dépôt de dépasser la notion de chômage afin de permettre à chacun de trouver ou de retrouver le chemin de l'activité, alors seulement le plein emploi deviendra réalité d'ici là, l'Union centriste votera ce texte, merci à tous de votre attention. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Françoise Giroud a écrit le chômage et comme une marée noire qui recouvre l'herbe verte, là où elle a poussé à à teindre Le Pen emploi est un objectif que poursuivent tous les gouvernements, mais malgré un retour massif de personnes sur le marché du travail, le taux de chômage en France se maintient à 7 4 % alors que les entreprises n'ont jamais éprouvé autant de difficultés à recruter, la situation est inédite, nous connaissons bien les effets délétères du chômage, perdre son emploi revient à perdre une partie de son identité sociale vécu comme un échec le chômage peut être un vrai traumatisme pour tous ceux qui y sont confrontés, état, dans cet esprit que vous avez souhaité, Monsieur le Ministre, mettre en place une stratégie globale pour que le chômage de masse ne soit plus une fatalité, le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui en est la première étape et d'autres chantiers suivront à cette occasion, permettez-moi de saluer le travail des maisons de l'emploi qui constitue aujourd'hui l'un des dispositifs d'insertion professionnelle, le plus efficace, proposant de véritables politiques de l'emploi au niveau territorial, elle permet à de nombreuses personnes de retrouver une activité professionnelle et nous espérons donc qu'elles seront financées dans le cadre du projet de loi de finances dont nous débattrons prochainement, j'en reviens au au projet de loi au sein de ce texte particulièrement resserré, une mesure cristallise toutes les tensions : l'article 1er qui vise à prolonger les règles d'indemnisation de l'assurance chômage, adoptée en 2019, mais aussi et surtout à engager une concertation avec les partenaires sociaux pour établir de nouvelles règles d'indemnisation, bien que vous nous vous vous soyez engagés à ne pas toucher au montant des allocations, je ne vous cache pas que les sénateurs du RDSE sont partagés sur cette disposition, nous regrettons d'avoir à légiférer dans l'urgence sur l'assurance chômage, mais si nous ne faisons rien, des millions de chômeurs ne pourront plus percevoir leurs indemnités, les règles d'indemnisation fixée par le décret de carence, c'est sans d'être applicable après le 1er novembre 2022 surtout certains collègues, déplore que l'article 1er dépouiller les partenaires sociaux de leurs prérogatives de gestion paritaire, et nous demande de vous signez en quelque sorte un chèque en blanc, comme le souligne en effet le Conseil d'État dans son avis, le projet de loi ne comporte aucune limitation directe ou quant à l'objet ou à la portée des dispositions du futur décret, c'est pourquoi le groupe RDSE défendra plusieurs amendements visant à redonner toute sa place au dialogue social, nous regrettons également que la commission des affaires sociales est introduit un nouvel article pour priver les salariés d'indemnisation du chômage en cas de refus de CDI répéter cette remise en cause des droits à l'assurance chômage nous semblent particulièrement dangereuse, elle est de nature à modifier profondément les règles de l'assurance chômage, sans garde-fou et sans discussions préalables là-bas et n'a pas un autre avis, sa place dans ce texte d'urgence, nous regrettons enfin qu'à l'occasion de ce projet de loi nous ne puissions pas traiter du dispositif territoires zéro chômeur sous peine que nos amendements soit déclarée recevable otite au titre de l'article 45, c'était d'autant plus incompréhensible que l'Assemblée nationale a quant à elle, autorisée que ce texte soit le véhicule législatif pour réactiver l'expérimentation du CDD multi- remplacement nous avons pourtant été alertés sur la nécessité d'alléger la procédure pour habiliter de nouveaux territoires et pour permettre la poursuite du développement de cette expérimentation, fil s'il se félicite en revanche de la réforme de la validation des acquis de l'expérience qui permet à toute personne d'obtenir un diplôme grâce à son expérience souvent jugé trop complexe par les entreprises et et trop chronophages par les candidats, ce dispositif ne s'est pas imposé dans le paysage de la formation professionnelle, c'est pourtant un formidable outil qui prouve que l'on acquiert qu'on a en acquièrent des compétences tout au long de sa vie et que tout n'est pas joué à l'issue de sa formation initiale, Madame et messieurs les ministres, les sénateurs du groupe RDSE seront particulièrement attentifs aux débats et réserveront leur vote en fonction du sort qui sera réservé à leurs amendements, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, ce projet de loi répond avant tout, une fois n'est pas coutume à une véritable urgence il s'agit de prolonger les règles actuelles d'indemnisation du chômage, qui arrivent à échéance le 1er novembre prochain demain afin d'éviter un arrêt soudain du versement des prestations, ce point ne prête bien sûr pas à discussion, cependant, le texte va au-delà en accordant à l'État, à titre exceptionnel, la possibilité de définir de nouvelles règles du régime d'assurance chômage, au moyen d'un décret ainsi que la relever le Conseil d'État, le texte ne comporte aucune limitation directe ou indirecte, quant à l'objet ou à la portée des dispositions du futur décret outre le blanc sans demander aux parlementaires, le projet de loi reflète la sonde donc pris progressivement par l'État sur la gestion de l'assurance chômage, comme l'a souligné récemment un rapport présenté par notre collègue Frédérique Puissat le paritarisme recule depuis plusieurs années dans la gestion des dispositifs de protection sociale, que ce soit en matière de sécurité sociale de formation ou d'assurance chômage, notamment la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les règles de négociation des conventions d'assurance chômage, en permettant au gouvernement d'imposer les orientations et les objectifs financiers à atteindre par une lettre de cadrage très strictement défini l'échec prévisible des négociations conduites en 2019 a abouti finalement à l'adoption d'un décret la situation présente est comparable, mais cette fois-ci le gouvernement, arguant de l'urgence ne se soucie pas d'engager une négociation et précise, a d'ores et déjà qu'il définira les mesures d'application du régime d'assurance chômage, par un décret en Conseil d'État, nous savons quelles mesures introduira ce décret, il s'agit de réaliser l'annonce de campagne du président de la République de moduler les conditions d'indemnisation en fonction de la situation du marché du travail, qu'elle soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse, quand le chômage est élevé, une simple concertation avec les partenaires sociaux est prévue et qui vient d'être lancée de modulation, il n'est pourtant point question dans le texte, le gouvernement pourra la prévoir ultérieurement ou pas et décider seul de ses conditions d'application cet ensemble de dispositions s'éloignant du système paritaire que nous pratiquons me conduit à saluer les propositions formulées par nos rapporteurs qui sont venus modifier l'article 1er sur plusieurs points : 1er Point et cela me semble plus important, un amendement a introduit le sujet de la gouvernance de l'assurance chômage, dans le texte afin de rétablir le rôle actif des partenaires sociaux en effet puisque la procédure de 2018 s'est traduite par un échec, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à l'esprit de la loi, l'archer selon le cadre transitoire que nous avons adopté en commission, après la publication du présent texte une concertation sera engagée par le gouvernement en vue d'une vraie réforme de la gouvernance de l'équilibre financier de l'Unédic et des règles d'indemnisation de l'assurance-chômage, à l'issue de cette concertation, le gouvernement interviendra par le biais d'un document d'orientation et non d'une lettre de cadrage selon une procédure inspirée de l'article L 1 du code du travail donnant davantage de valeur à la négociation, second point, la commission a limité dans le temps la liberté laissée au gouvernement pour fixer les règles d'indemnisation des chômeurs en avançant le délai qui lui est accordée au 31 août 2023 cette situation étant exceptionnel, il n'est en effet pas souhaitable de la laisser perdurer plus que nécessaire 3ème point puisque cette faculté du gouvernement vise à créer un principe de modulation de l'indemnisation chômage, en fonction de la conjoncture, nous avons choisi d'inscrire en toutes lettres, ce principe dans le projet de loi nous considérons en en fait comme légitime l'objectif poursuivi s'attaquer aux difficultés de recrutement que connaissent actuellement les entreprises en dépit d'un taux de chômage réduit à 7,4 selon les chiffres du ministère du Travail 60 % des entreprises rencontre actuellement des difficultés de recrutement ayant terminé un tiers d'entre elles à limiter leur activité chaque jour dans nos circonscriptions des employeurs nous disent ne pas trouver de salariés les conditions d'indemnisation du chômage, selon diverses études, joue un rôle important pour la reprise d'emploi élaboré une règle d'ajustement, en fonction de la conjoncture semble donc souhaitable et jouerait dans les 2 sens, tenant compte des périodes de croissance mais également de récession il faut par ailleurs rappelé que même après le durcissement opéré en 2019, les conditions d'éligibilité à l'assurance chômage en France reste parmi les plus favorables de l'OCDE, cependant, en l'absence d'étude d'impact et de détails sur les modalités de la réforme, notre groupe émet les plus grandes réserves sur sa faisabilité, quelles seront les indicateurs permettant de déterminer si la conjoncture est bonne ou mauvaise ah quels intervalles, la situation économique sera-t-elle reconsidérer, vous semblez avoir rejeté Monsieur le Ministre, une appréciation par territoire, mais si l'on prend en compte la conjoncture économique nationale pourra-t-on appliquer les mêmes règles dans ma région, des Hauts-de-France grandement en intention que sur d'autres territoires, alors que le taux de chômage peut varier du simple au double, il serait préférable que l'analyse soit faite par bassin d'emploi, voire même parfois par quartier dans dans certaines villes, nous comptons sur nos débats pour obtenir des précisions de la part du gouvernement, d'autres sujets ont été introduits dans le texte à l'initiative de nos rapporteurs dont je tiens à saluer la démarche pragmatique, la qualité du travail et l'investissement sur des questions sensibles car d'ordre social, la question avait été posée à l'Assemblée nationale de restreindre les droits au chômage en cas de refus répétés de CDI suite à un CDD, situation qui nous est souvent décrite sur le terrain, notre commission a choisi d'intégrer cette disposition et a souhaité que ce refus d'un emploi stable soient particulièrement caractérisée en fixant la suppression du droit à indemnisation à partir de 3 refus, elle a par ailleurs répondu aux observations que vous aviez formulé à l'Assemblée, Monsieur le Ministre, en prévoyant une notification des refus à Pôle Emploi, je tiens à préciser qu'à titre personnel, je soutiendrai l'amendement de nos collègues, Laurent Duplomb et Bruno Retailleau, qui supprime l'indemnisation du chômage dès le 1er refus de CDI car à partir du moment où le CDI correspond même emploi exercé auparavant en CDD, il n'y a aucune raison d'attendre un 2ème ou un 3ème CDI, sauf bien sûr à ce qu'il ait trouvé un autre CDI dans un même esprit de justice vis-à-vis des autres demandeurs d'emploi et parce qu'il s'agit que d'une source importante de dysfonctionnement pour les entreprises, la commission a complété le dispositif introduit par les députés concernant les abandons de poste afin de sécuriser la procédure permettant de les assimiler à des démissions je dirais encore quelques mots sur les contrats courts, la commission a supprimé la durée maximale de 36 mois applicable aux missions accomplie en CDI, ce qui permet de sécuriser les parcours professionnels des intérimaires, tout en limitant le recours aux contrats courts, elle a également fixé pour 2 ans l'expérimentation autorisant la conclusion de CDD pour remplacer plusieurs salariés absents notre sentiment sur le dispositif de bonus-malus, créé en 2019 n'a pas changé, nous y voyons toujours un frein à l'emploi et une méconnaissance des impératifs de flexibilité auxquelles sont soumis certains employeurs le nous a donné l'occasion de revoir le dispositif afin de le recentrer sur les véritables cas de permittence et d'alléger son impact financier pour les entreprises, j'évoquerai enfin la VAE que nous avons à toute activité en lien avec une certification en dépassant l'actuel approche par statut afin de donner un nouvel élan à ce dispositif insuffisamment utilisée ainsi l'examen de ce projet de loi malgré son ambition très limité, nous a permis de traiter plusieurs difficultés rencontrées par les entreprises ou les demandeurs d'emploi et d'affirmer notre attachement au paritarisme, nous sommes dans l'attente d'autres mesures, que ce soit sur le plan de la gouvernance de l'assurance chômage ou sur le plan de l'emploi, car si le taux de chômage a baissé en France, il reste largement supérieur à celui de la moyenne européenne, sous réserve du maintien des dispositions dont nous avons enrichi le texte notre groupe votera ce projet de loi, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame et monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le président de la République a mis au coeur de son projet, une ambition forte, atteindre le plein emploi d'ici 2027 cet objectif de nous rassembler au-delà de nos sensibilités politiques et de nos appartenances partisanes. Atteindre le plein emploi, c'est permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société, quel que soit son origine sociale, c'est valoriser le travail, la création, les compétences et récompensé toujours les efforts, c'est enfin nous donner les moyens de financer notre modèle de protection sociale, mais comme souvent en politique, c'est moins l'objectif qui fait débat, que les moyens mis en oeuvre pour la table, je suis sûr que nos discussions au coeur des des prochains jours seront riches, je souhaite aussi qu'elle tienne compte de la réalité, et singulièrement du travail accompli depuis 2017 il y a 5 ans, on se demandait encore comment lutter contre le chômage de masse qui sévissait dans dans des décennies dans notre pays depuis des décennies, désormais nous entrevoyons l'espoir de vaincre pour de bon, en clair, nous sommes passés de N'objective négatif à un objectif positif c'est loin d'être anecdotique mais cela nous oblige à prendre des mesures courageuses, c'est déjà ce qui a été fait au cours des 5 années précédentes, j'espère que nous aurons de nouveau des échanges compte constructive dans cet objectif, voilà la mission qui nous échoit à nouveau aujourd'hui, avec ce projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ce texte vise essentiellement à réformer l'assurance chômage, afin de garantir l'efficacité et l'équité du régime lors du précédent quinquennat les principales réformes, que ce soit sur le marché du travail sur l'apprentissage sur la formation professionnelle, ou encore sur l'assurance chômage ont été engagées quand la conjoncture était plus favorable, mais ces réformes structurelles ont permis à notre pays de tenir bon par gros temps d'abord pendant la crise sanitaire maintenant, avec la crise énergétique et l'inflation malgré tout cela, le taux de chômage avoisine encore les

Bien sûr, on pourrait dire que la situation actuelle est nettement moins favorable qu'elle ne l'était avant la pandémie et pourtant, grâce aux réformes dont j'ai parlé et grâce aux mesures d'urgence et au plan de relance le marché du travail est très tendu, ce qui profite aux travailleurs malgré la situation leur pouvoir de négociation, hé bien réel, en conséquence, le régime d'assurance chômage se portent plutôt bien les nouvelles prévisions de l'Unédic, publiée jeudi dernier, montre que le régime pourrait dégager près de 13 milliards d'euros d'excédents sur la période 2022 2024, ce sont 3 milliards supplémentaires par rapport aux prévisions de juin dernier cette amélioration doit nous encourager à faire bouger les lignes sur ce sujet sensible, il nous faut à la fois mieux valoriser le travail et mieux protéger TG, pardon, les demandeurs d'emploi, mais je crois que nous pourrons trouver de nombreux consensus, la commission des affaires sociales a mené un travail sérieux, en validant la plupart des mesures du gouvernement et en y ajoutant d'autres mesures pour mieux valoriser le travail, je pense notamment à la notification à Pôle Emploi de tout refus de CDI au terme d'un CDD, nous avions proposé un amendement dans ce sens en commission, je me réjouis que nos rapporteurs est intégré une telle disposition au texte. Idem pour les abandons de poste, l'Assemblée nationale, a ajouté cette disposition et nous l'accueillons favorablement, il ne s'agit pas de lutter contre un phénomène majeur : le nombre de ces pratiques restent globalement stables, mais bien d'une question éthique, on ne peut pas octroyer une allocation, un salarié qui abandonne son poste et la refuser à celui qui démissionne en respectant les procédures, enfin sur la validation des acquis de l'expérience, nous soutenons la création d'un nouveau service public pourvu qu'elle se fasse à moyens constants, nous souhaitons que les départements puissent y être associés, si la formation est un volet de la politique sociale, alors ils ont toute leur place, les politiques de l'emploi doivent garantir la solidarité entre les actifs sans compromettre la compétitivité de notre économie, cette tension entre les objectifs apparemment opposés, nous oblige à trouver des des compromis, mais il y a là rien de nouveau sous le soleil, c'est le propre du dialogue social que de trouver des compromis en responsabilité pour conclure je souhaite évoquer le rôle des partenaires sociaux dans le régime d'assurance chômage, la commission a souhaité accélérer le retour au paritarisme de gestion c'est une question de fond, à laquelle nous allons répandre le groupe les indépendants et favorable au dialogue social, mais nous sommes aussi aussi attachés à pouvoir réformer le régime afin d'en préserver l'équilibre financier, je vous remercie.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous examinons ici le premier acte d'un vaste plan antisocial qui, de l'assurance chômage ou au RSA en passant par la retraite va émaillé notre session parlementaire sous l'égide ressusciter du travailler plus pour gagner plus en fait autant dans son discours de politique générale, madame Borne l'annonçaient leur serait à travailler plus, plus longtemps, pour atteindre un plein emploi 5 % et se conformer aux orientations de rigueur budgétaire du programme de stabilité aux recommandations du semestre européen et régulièrement du Conseil d'analyse économique, comme toujours, la doxa néolibérale did le gouvernement qui justifie sa politique de stigmatisation des chômeurs par la mise en avant d'un faux paradoxe entre les emplois non pourvus et le nombre de chômeurs déjà en 2003 François Fillon jugeait inacceptables les 300000 emplois non pourvus, chiffre sans cesse agitée depuis 20 ans jusqu'à récemment, sans analyse sérieuse de son contenu et de sa pertinence pour justifier ce prétendu paradoxe en regard du chômage, la réalité c'est que, selon les chiffres de Pôle emploi sur les 3 2 millions d'offres d'emplois recueillies et clôturé en 2018, seuls 157000 ont été non pourvus et guère plus en 2021, soit de 5 à 6 % du total des offres, la réalité c'est que même si ces Oeuvres trouvé preneur, elles sont largement insuffisantes pour combler le chômage endémique et offrir des opportunités, ne serait-ce qu'que 3 millions de chômeurs de la catégorie à la réalité, c'est que la majeure partie de ses offres d'emploi non pourvues ont reçu plusieurs réponses de candidature, mais qu'elles ont été rejetées par les employeurs et que, selon Pôle emploi, je cite, les 3 quarts des recruteurs d'une offre non pourvus, reconnaissent que les conditions de travail du poste proposé peuvent décourager le candidat les offres non pourvues résiduels ont donc à voir essentiellement avec la qualité de l'offre d'emploi et des conditions de travail et non du fait de chômeurs non-actifs dans leur. Recherche d'emploi, la d'Darès ce souligne dans une enquête sur les métiers en tension, en 2021 en expliquant que les difficultés d'embauche était lié aux conditions. Travail et aux salaires insuffisants, au point que, selon le l'OFCE 60 %. Des chômeurs non indemnisés ne les accepte pas non plus, de sorte que vous pouvez bien faire une énième réforme de l'assurance chômage, cela ne changera, je tiens à cette tension et vous le savez, le premier objectif, c'est bien la recherche d'économies en abaissant les droits des demandeurs d'emploi dans un pays toujours plus inégalitaire dans le partage de la richesse, ces réformes successives de l'assurance chômage, ciblant les demandeurs d'emploi sans s'attaquer aux problèmes structurels de la qualité des offres d'emploi entraîne le pays sur le chemin d'un plein emploi répressif où sont attaqués, les capacités d'arbitrage des chômeurs, les études sur le modèle canadien promu dernièrement le montre l'augmentation de la durée d'affiliation, la baisse de la durée d'indemnisation ou du taux de remplacement comme la territorialisation, on pourrait faire deux contraint d'une partie des chômeurs soit accepter des emplois mal rémunérés de moindre et de moindre qualité, soit à se voir radier, cela entraîne des externalités négatives car la baisse des indemnités chômage pèse sur le niveau général des salaires, vous vous attaquez au pouvoir d'arbitrage des chômeurs après avoir affaibli la capacité de négociation des salariés eux en poste, via les ordonnances Macron et les lois de travail antérieur, c'est la même politique et pour ce qui est des écologistes, nous ne ferons pas l'erreur de les opposer comme le discours ambiant nous y invite, vous défendez une société du travailler plus et et prétendument de la valeur travail, alors que l'avenir appartient au partage et à la baisse du temps de travail, d'abord pour une raison ancienne déjà par Marx, je cite : mais oui écoutez la condition essentielle de l'épanouissement et la réduction de la journée du travail, vous refusez de voir que la vague de démissions traduit une demande de transformation du travail de passage c'est bullshit jobs de David, 13 Treiber à des employes émancipateur à l'utilité sociale et environnementale, ensuite parce que votre modèle productiviste explose une à une les limites de la biosphère et qu'il nous faut urgemment ralentir, nous défendons la sécurisation du parcours professionnel, loin de la précarisation et de la paupérisation de ces réformes successives, le temps est venu non de travailler plus, mais de reprendre la marche vers la réduction du temps de travail que permet le partage des richesses et que, et qu'ils doivent respecter les limites planétaires, c'est pourquoi le groupe écologiste votera contre ce projet de loi, je vous remercie. La parole est à monsieur lévriers pour le groupe RDPI et pour six minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame et monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le plein emploi en France n'est pas une utopie, un simple Chypre factuel, le taux de chômage au sens du BIT a baissé de 2 2, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, à l'arrivée à l'Élysée, absolument, force est de constater que la réforme de 2019, engagé en 2019 porte pleinement ses fruits, la part des contrats courts dans les offres d'emploi disponibles diminue, plus de la moitié des embauches sont signés en CDI, contre 30 % en 2000 19 et au sein des 7 secteurs les plus exposés aux contrats courts 62 % des entreprises auront un bonus en 2022, ces chiffres montrent dans le contexte économique que nous connaissons une volonté des entreprises de préférer des contrats longs et des renouvellements aux contrats courts et précaire pour autant si l'amélioration est particulièrement marqué la France compte encore 7 3 % d'actifs sans emploi, c'est encore trop, et c'est la raison pour laquelle le président de la République et la première ministre oh mis l'objectif du plein emploi pour 2000 27 au coeur de votre feuille de route, le projet de loi que vous soumettez avec madame la ministre, Carole Granjean à la représentation nationale est une première étape vers cet objectif pour l'atteindre, vous prolonger les règles d'indemnisation de l'assurance chômage, issues de la réforme de 2019 en raison de la pandémie, ces règles sont entrées en vigueur il y a à peine un an, c'est trop peu pour en observer les premiers effets une série de travaux d'études et de recherches pour les évaluer, et d'ailleurs en cours, vous ouvrez une concertation approfondie avec les partenaires sociaux pour rendre les règles plus réactive à la conjoncture économique et à l'évolution du marché du travail, c'est un engagement du président, il est nécessaire d'avoir des règles incitative à la reprise de l'emploi quand les conditions économiques sont favorables, et inversement, de pouvoir compter sur un système plus protecteur quand l'économie va mal, quand des emplois sont détruits vous lancer une négociation pour redéfinir la méthode de gouvernance de l'assurance chômage, les partenaires sociaux et l'État partage le souhait de faire évoluer la gouvernance pour mémoire, les partenaires sociaux n'ayant pas réussi à trouver un accord majoritaire, l'État a dû reprendre la main, il a dû édicter des règles de l'indemnisation de l'assurance-chômage par décret de carence, celui-ci ne peut avoir une durée de vie supérieure à 3 ans ce décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi fixe jusqu'au 1er novembre 2022 les règles fixes, pardon, jusqu'au 1er novembre 2022, les règles d'assurance chômage, ce texte s'impose à nous d'un point de vue calendaire, vous proposez une clarification des dispositions du code du travail afin de rétablir la base légale relatives aux conditions pour être électeurs aux élections professionnelles, vous posez et c'est d'importance, les premiers jalons d'une réforme de la VAE qui va la rendre plus attractive et plus elle et plus accessible afin de parvenir à une a initié 100000 parcours de VAE chaque année d'ici la fin du quinquennat vous simplifier et moderniser les conditions d'accès a fait non afin d'en faire un instrument simple au service de tous les actifs qui souhaitent évoluer dans leur carrière, la VAE qui célèbrent cette année ses 20 ans constitue un dispositif pertinent et efficace de promotion d'évolution et de transition professionnelle, il est pourtant sous-utilisé et mal connue, donc compte de nos concitoyens, avec seulement 30000 parcours réalisé en 2021 contre 60000 il y a 10 ans. Fondée sur le principe de la reconnaissance des compétences acquises tout au long de la vie, cet outil permet d'accéder à une certification reconnue et développe ainsi l'employabilité de tous les actifs, en particulier les moins qualifiés et les plus éloignés de l'emploi, poursuivant cet objectif ce texte ouvre l'accès à la VAE pour des proches faisaient dans la reconnaissance des compétences acquises au contact d'un proche en situation de handicap, de perte d'autonomie ou accompagner à la fin de sa vie, leur permettra d'initier un parcours vers des certifications pour des métiers en forte tension de recrutement à l'instar des auxiliaires de vie, des aides-soignants, la majorité sénatoriale propose un amendement qui ouvrent des pistes, on est allé en élargissant le public cible, mais la réforme vient d'être amorcée et c'est sans doute prématuré pour conclure tous ces leviers précédemment cités doivent d'une part, permettre de répondre à la pénurie de main-d'oeuvre en augmentant le nombre de personnes aptes à occuper un métier en tension et accompagnée et valoriser les reconversions professionnelles des salariés si notre groupe mesurent la nécessité du projet de loi portant premières mesures d'urgences relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi et des modalités qui l'introduit il s'interrogent quant à l'intérêt de certains amendements rapporteur, notamment concernant le déplore plafonnement de l'intérim ou encore les modifications des paramètres du bonus malus, nous proposerons avec plusieurs collègues, un amendement visant à revenir sur la suspension des allocations chômage suite à 3 refus de CDI, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant madame Monique Lubin, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame et monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous émouvant, souvent sur les bancs de l'opposition de l'insuffisance des études d'impact accompagnant les projets de loi du gouvernement et nous nous inquiétons de sa propension à accumuler les réformes radicales en faisant fi du travail parlementaire, sans jamais se donner le temps de l'évaluation, le présent projet de loi ne fait pas exception, il se fonde sur une poignée d'idée hâtive et qui a malheureusement en partage avec la majorité du Sénat au titre de ses idées hâtive et les demandeurs d'emploi seraient largement indemnisés il faudrait inciter plus violemment les actifs en situation d'emploi discontinu à reprendre un travail pérenne, l'assurance chômage leur serait trop favorable, notre système d'indemnisation les inciterait à s'enfoncer dans la paresse et la fraude, une étude de Mathieu Grégoire et de clair Vivès ses idées en brèche publiée dans la revue de l'institut de recherche économique et sociale l'IRES, elle porte sur l'évolution des droits à l'assurance chômage de 1979 à 2021, elle établit qu'en matière d'indemnisation au chômage l'affirmation selon laquelle les droits des salariés à l'emploi discontinu a progressé jusqu'à dépasser les droits des salariés stables apparaît en complet décalage avec les résultats des simulations, mise en place, c'est le contraire qui se dessine l'indemnisation totale d'un salarié payé au SMIC à mi-temps subi une perte spectaculaire depuis 1979 en 2019 le montant perçu par ce salarié est inférieur de 50 % par rapport à ce à quoi il pouvait prétendre en 1979. La réforme de l'assurance-chômage, du premier quinquennat procédaient des préjugés ici battue en brèche, elle a toujours selon la même étude radicaliser l'évolution de l'assurance chômage vers une logique de comptes épargne, on y est indemnisé en fonction non pas du salaire mensuel, mais du salaire journalier, cela conduit, je cite, à inverser la hiérarchie des niveaux d'indemnisation entre eux alors que les plus exposés au chômage étaient les mieux indemnisées, ils sont des sont désormais les moins bien indemnisés le gouvernement avec le présent projet de loi promis de continuer sur cette lancée, Mathieu Grégoire vivait signale par ailleurs que les publications officielles tant de ta communiqué sur le taux de couverture de l'indemnisation du chômage pour définir ce taux ces publications renvoi non pas aux chômeurs indemnisés mais aux chômeurs indemnisables, ça fait une sacrée différence à partir de 2014 et jusqu'en 2019 le différentiel entre les indemnisables et ceux qui sont effectivement indemnisés s'accroît en effet de 5 4 points, c'est plus du quart des personnes dites couvertes par les systèmes d'indemnisation chômage qui ne perçoivent aucune indemnisation en 2018, comme le souligne l'IRES, on peut considérer qu'alors que le nombre de demandeurs d'emploi n'a jamais été aussi élevé avec près de 5 725 millions de personnes inscrites en catégorie ABC en janvier le taux de couverture, a atteint son niveau le plus bas de l'histoire et de l'indemnisation du chômage en juin 100 communiquer sur le taux de couverture en évoquant dans le sous-texte que les indemnisables c'est faire miroiter un système d'assurance chômage plus généreux qu'il ne l'est, ce n'est pas innocent cette insincérité dont fait preuve l'exécutif est l'une des raisons pour lesquelles nous nous opposons à l'article 1er du présent texte au nom d'une nécessité administrative exploité à des fins politiques, il prétend conférer au gouvernement toute latitude pendant de longs mois pour modifier les règles de l'assurance chômage, sans plus se soucier du Parlement ou des partenaires sociaux pour mémoire, comme le rappelait en 2001 Bruno Palier au moment de faire les choix d'orientation de la Sécurité sociale en 1945 une coalition d'intérêts se dresse contre l'intervention de l'État pour le dialogue social et une mise aux responsabilités des partenaires sociaux, c'était une demande des syndicats, elle a rencontré la volonté de Pierre Laroque, de mettre en place des corps intermédiaires dans lesquelles les représentants des salariés et des patrons auraient un rôle à jouer, ce choix de promouvoir les partenaires sociaux s'est accompagné de celui de reconduire la logique assurantielle pour les allocations chômage, le but était, selon Bruno Palier, d'intégrer les travailleurs en leur proposant de participer à la gestion du système de protection sociale, selon le principe si vous payez-vous gérer Pierre Laroque, ne voulait pas que le système de protection sociale soit financée par l'impôt, car alors les dépenses sociales seraient soumis à la contrainte budgétaire, c'était signifier que la demande sociale vient en 1er et le financement seulement ensuite dans un système qui privilégie d'abord les droits et envisage dans dans un 2ème temps l'ajustement financier. C'est dans cette logique que des tricots de votre politique et le présent projet de loi avec la désocialisation à marche forcée de notre système de protection sociale, vous ne réservé aux partenaires sociaux qu'un strapontin, voire un siège éjectable le choix fait, ici comme ailleurs, de ne pas parler de négociation mais de concertation illustre au demeurant la place que vous leur réserver l'introduction par la droite au cours de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale et au Sénat, de mesures de plus en plus restrictives concernant l'accès à l'assurance chômage témoigne par ailleurs d'un accord profond du gouvernement avec la supposée opposition de droite, la transformation de l'abandon de poste en démission attestent du choix de gouverner aux préjugés et d'une volonté d'incriminer le travailleur rien, je veux dire bien rien ne document, une pratique qui soit abusive massive illégitime de l'abandon de poste au contraire ceux qui recourent doivent pouvoir le faire pour se soustraire à toute configuration tels que de me à son poste, le travailleur mettrait en danger sa santé physique ou psychique ou se verrait victime d'abus, je ne sais pas, par ailleurs, je ne sais par ailleurs même pas s'il est nécessaire de commander, de commenter l'amendement introduit dans le texte par la majorité en commission des affaires sociales du Sénat, cet amendement crée en effet une possibilité supplémentaire de priver un demandeur d'emploi, de ses indemnités et il le fait sur une base nébuleuse, je serais très curieuse de savoir où il prend ses fondements, il part en effet d'une situation qui relève d'une exception, celle d'un demandeur d'emploi qui aurait refusé, sur une période de 12 mois, 3 offres de CDI à la suite d'un CDD, cette offre de CDI portant sur un emploi similaire et étant rémunérés au même salaire, quelles sont les études qui établirait que cette situation soit une donnée statistique critique justifiant la mise en place de cette mesure, on ne peut pas construire une loi à partir de considérations non documenté. Dans le même mouvement, vous avez inscrit la contrat cyclicité comme principe de modulation des indemnités chômage dans le code du travail, la conjonction de ces 2 innovations dispensable a pour résultat que nos concitoyens dans la perspective de recharger leurs droits à indemnisation et pour survivre, pourront être amené à accepter un CD des sous-qualifiés ou sous-payés et se voir obligé de rester dans cet emploi, c'est déguisé sous peine d'être radiés, vous semblez tenter d'instituer un droit de réquisition des travailleurs banalisé dans notre code du travail. Mise en avant par le gouvernement pour promouvoir son projet de loi, la promotion de la validation des acquis de l'expérience comme voie d'accès aux proches aidants et aux aidants familiaux à une professionnalisation suscite quant à elle des réserves, comme l'expliquera ma collègue Michèle Meunier au moment où l'on parle de sens du travail de grande démission de souplesse et de qualité de vie de juste rémunération, le gouvernement et ses alliés répondent rétorsion suspicion et incrimination des travailleurs, loin de ces dérives, j'ai déjà eu l'occasion de rappeler qu'il ne peut y avoir de valeur travail sans valeur de son travail de valeur, rien ne peut se faire en réduisant les travailleurs au statut d'unités de production dépouillé de droit Robert Castel rappelle que le salarié n'a pas gagné sa prime n'a gagné sa prééminence que parce qu'à partir de la condition salariale par la mise en place de droits étant attaché un État social a été mis en place avant cela on était salarié lorsqu'on était rien et que l'on n'avait rien à échanger, hormis la force de ses bras, notre système social, notre assurance chômage ont été mises en place pour nous permettre de faire société et intégrer les travailleurs, le gouvernement et ses alliés choisissent de les maltraiter, de faire taire leurs représentants à coups de 49 3 et de lois dont la sincérité interroges, renforcer la cohésion sociale et plus que jamais nécessaire, nous sommes à un moment de notre histoire, nous avons besoin de refaire société et ce besoin le gouvernement le prend complètement à rebours idée, il n'y a d'équations fondamentales avec les besoins du pays, nous voterons contre ce projet de loi qui tourne le dos aux fondements de notre démocratie sociale. Et Madame avec : Annick Jacquemet, conclut la discussion générale, pour l'Union centriste. Monsieur le président, monsieur le ministre madame et monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, comme nous le savons, le droit du travail est un domaine plus que complexe, en effet, il organise les droits et devoirs de l'ensemble des employeurs et des travailleurs, afin de garantir l'équilibre entre les parties et de protéger, chacune d'entre elles, l'enjeu qui est le nôtre et de faire évoluer notre droit pour rester au plus près du fait social sans entacher les acquis passer à ce titre, nous devons également garantir l'application des protections sociales associent nos rapporteurs, dont je salue l'excellent travail l'ont assurément menée en suivant ses objectifs de bon sens, c'est pourquoi ce projet de loi s'attache dès son article 1er à donner une base légale et réglementaire à l'indemnisation des demandeurs d'emploi à compter du 1er novembre 2022, il autorise le gouvernement à prendre par décret, les mesures d'application du régime d'assurance chômage, jusqu'au 31 décembre 2023 cette mesure dérogatoire et proportionnée à la nécessité de l'urgence permettra au paritarisme de signer un accord portant sur l'assurance chômage, dans un délai rapide mais suffisamment importants pour le bon déroulement des échanges par ailleurs il prolonge jusqu'au 31 août 2024 l'application du bonus-malus à l'article de la Commission a précisé utilement le Champ d'application et c'était nécessaire le bonus-malus permet de dissuader de dissuader la généralisation des contrats précaires et à l'inverse de récompenser les entreprises plus vertueuse sur ce sujet l'article aménage le dispositif en permettant la transmission aux employeurs de la liste des anciens salariés pris en compte pour le calcul du bonus-malus attendu par le secteur cette mesure semble de nature à améliorer la transparence du dispositif, l'article IV porte sur la validation des acquis de l'expérience cet article concernée d'abord le secteur médico-social et en particulier celui de la danse, notre groupe se réjouissait déjà de cette bonne évolution en faveur des aidants cet article largement con con complété réforme désormais plus profondément la la validation des acquis de l'expérience tout en sécurisant le dispositif la création d'un Jeep devrait contribuer à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours à la promotion de la VAE ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur le territoire. Par ailleurs, la navette parlementaire a enrichi ce texte de plusieurs dispositions notable. La présomption de démission en cas d'abandon de poste s'il convient de remarquer que certains abandons de poste sont totalement justifiée, il est aussi vrai qu'un fort dévoiement du principe est observée dans les fêtes, or il n'est plus souhaitable qu'un salarié licencié à l'issue d'un abandon de poste, dispose d'une situation plus favorable en matière d'assurance chômage qu'un salarié qui démissionne en faisant présumer la démission de l'intéressé, l'article tend à sécuriser le bon usage du droit en fin de relations contractuelles toutefois sans la soupape de sécurité du dispositif, ce nouveau principe aurait pu être largement critiquable requins au regard des abandons de poste justifiée par des situations parfois dramatiques. L'expérimentation du CDD multi-remplacement a été réactivé, cela était nécessaire dans la mesure où l'expérimentation a été peu contributive en raison de la crise sanitaire, les conclusions de celles-ci permettront je l'espère, aux employeurs de recruter avec un seul contrat une personne pour remplacer plusieurs salariés d'une même entreprise pour conclure et malgré que le titre de ce projet de loi semble plus ambitieux que les mesures qui le composent le groupe Union centriste votera en faveur de ce texte, je vous remercie. Merci madame la présidente. Merci madame Monsieur le Ministre, vous souhaitez conclure la discussion générale, vous avez la parole. apporte un certain nombre de mesures en matière de réforme des règles de l'assurance chômage en matière de validation des acquis de l'expérience, mais qui, évidemment, ce texte ne peut pas être le seul, en matière d'emploi, ça ne peut pas être le seul outil les questions relatives à la formation à l'accompagnement des hommes et des femmes les plus éloignés de l'emploi, les questions relatives à la formation initiale, je pense à la à la réforme de la voie professionnelle, ou encore au développement de l'apprentissage, sont autant de sujets qui nous permettront d'aller vers le plein emploi et j'aurais pu ajouter en écho à des concertations menées actuellement les aspects relatifs. Au travail des des seniors au taux d'emploi des seniors pour reprendre le terme consacré ou encore aux conditions de travail et donc nous irons évidemment plus loin, nous aurons d'autres occasions de discuter d'outils permettant d'aller vers le plein emploi au-delà des seules dispositions de ce texte, il ressort, monsieur le président des des discussions en tout cas les interventions 4 thèmes qui je crois vont peut être structuré nos nos débats nous échange le 1er concerne la la place du paritarisme et nous y reviendrons dans dans un instant avec un amendement du gouvernement que je proposerai à votre assemblée pour établir la rédaction de l'article 1 la la commission des affaires sociales, sur proposition de de madame la rapporteure, je crois, à modifier cet article, hein, en limitant la durée et la date butoir d'application du texte et en prévoyant une prochaine une forme dérogatoire pour organiser le dialogue social autour de la gouvernance de l'assurance chômage, je suis assez convaincu qu'au-delà des des choix faits par la commission des Affaires sociales et de ceux du gouvernement, une forme de de consensus fenêtre autour de ce sujet-là, nous n'avons effectivement pas ouvert de négociation interprofessionnelle autour des questions d'indemnisation au moment où nous aurions dû le faire, c'est-à-dire au moment de l'élection présidentielle pour respecter les délais, propre à la recherche d'un Annie, ce qui nous amène dans la situation d'urgence que nous connaissons et ce qui nous amène donc à à demander une prolongation possible des règles jusqu'au 31 décembre 2023, de manière à ce que cette date soit cohérente avec d'autres éléments de calendrier, j'y reviendrai par contre sur les questions de gouvernance, le rôle du paritarisme, je me suis engagé, c'est l'occasion pour moi de le répéter devant vous auprès de tous les partenaires sociaux à l'ouverture d'une négociation et d'une négociation qui soit une négociation très ouverte il y a 4 grandes familles de scénario pour la gouvernance de l'assurance chômage, un seul ne recueille pas l'assentiment du gouvernement, c'est celui de l'étatisation de l'assurance-chômage, mais pour les autres, le document sur lequel nous engagerons cette négociation sur un document ouvert permettant justement à la négociation d'aller au bout de, de tous les aspects 2ème sujet qui peut faire débat concerne. L'abandon de poste, la sénatrice Cohen qui a Madame la sénatrice, vous avez raison sur le fait qu'il n'y a pas d'agrégats statistiques précis permettant de mesurer le nombre d'abandons de poste les abandons de poste donne lieu à des licenciements pour faute grave et donc ce que nous pouvons mesurer, c'est l'évolution du nombre de licenciement pour faute grave, quand on regarde le nombre de de CDI, faisant l'objet d'une rupture pour licenciement pour faute grave, une augmentation est est assez conséquente, mais elle est proportionnelle à l'augmentation du nombre d'emplois en CDI dans le pays et donc on peut considérer qu'il n'y a pas d'évolution majeure par contre est ce qu'on regarde le nombre de licenciements pour faute grave concernant des employées en CDD, il y a un doublement du nombre de licenciements et je fais procéder ainsi, de recherche, mais il paraît très vraisemblable que ce soit cette vague de d'abandon de poste que nous connaissons notamment sur des CDD, en particulier dans des secteurs comme l'les le riz, les cafés et les restaurants qui explique cette augmentation par contre là où nous aurons un débat, c'est que nous considérons effectivement que l'abandon de poste lorsqu'il n'est pas justifiée par une mise en danger et c'est en cela que j'accueille très favorablement les évolutions apportées par la commission des affaires sociales, l'abandon de poste, il n'est pas justifiée par cette mise en danger est une rupture d'un engagement contractuel qui doit s'apparenter à une démission, ça n'est pas un droit que d'obtenir une indemnité Unédic après avoir procédé un abandon de poste si celui-ci n'est pas motivée par un danger ou des questions liées à la à la sécurité, y compris parfois des formes de de maltraitance 3ème sujet qui va je crois occuper beaucoup de nos débats, la question du du bonus malus, j'ai, j'y reviens, pas simplement pour dire que certain nombre d'arguments dont j'ai été évoquée pour justifier du maintien de cette procédure, nous vous proposons de le faire avec un horizon au 31 décembre 2024 pour respecter les cycles d'observation, une mise en oeuvre de trois ans, telle que prévue pendant la loi de 2019 mais je, je m'arrête là pour ne pas être trop long, nous y reviendrons, et enfin la question des refus de CDI, elle a, à l'issue d'un d'un d'un ou de plusieurs CDD j'ai j'ai dit mais plus grandes réserves sur l'amendement adopté en commission, elles sont par définition encore plus importante pour l'amendement qui vise à appliquer une forme de sanction dès le 1er refus d'un CDI, il y a plusieurs raisons à cela des raisons très pratique, mais aussi les raisons de fond, je considère que lorsqu'un salarié embauché pour une durée déterminée, est allé au bout de son engagement contractuel sans à aucun moment, revenir sur l'engagement qu'il a pris, il n'y a pas de de raisons de de le sanctionner si ils refusent de continuer ou de prolonger dès lors que lui-même a tenu l'intégralité des engagements pris initialement j'ajoute par ailleurs que le code du travail prévoit d'ores et déjà en cas de proposition d'un CDI dans les mêmes termes que le CDD et il faut souligner cette cette égalité des termes la possibilité pour l'employeur de ne pas verser la prime de précarité, si l'employeur démontre qu'il a proposé un CDI dans les mêmes conditions que le CDD qui qui s'achève enfin beaucoup de d'intervenants ont évoqué la la validation des acquis de l'expérience, je n'y reviens pas les débats sur l'article 4 permettront à même à Ministre délégué Carole Granjean, dont je précise qu'elle nous a quittés pour assister et me représenter aussi aux questions d'actualité au gouvernement de l'Assemblée nationale, aura l'occasion de de s'exprimer devant vous et de répondre à l'ensemble de vos questions. Merci, monsieur le Ministre, donc nous. Tous vont clore pardon à la discussion générale et nous passons à la discussion du texte de la commission et à l'article 1er Monsieur mouillé la parole. Merci monsieur le président, monsieur ministre, mes chers collègues, à l'occasion de l'examen de ce premier article, je tiens à prendre la parole pour me faire l'écho de l'expérimentation territoire zéro, chômeur de longue durée, cette expérimentation Monsieur Ménez qui fonctionne bien et de nombreux territoires français souhaite adhérer de nouveau la loi du 14 décembre 2020, a donné la possibilité à 50 nouveaux territoires de s'engager dans ce processus, le chiffre est atteint et de nombreuses collectivités et de nombreux partenaires sous les sites l'organisation pour continuer à adhérer pour aller plus loin et augmenter le nombre de territoires. Dans l'état actuel, seul un décret au Conseil d'État peut permettre l'habitation de nouveaux territoires, il semblerait plus simple et cohérent de modifier la loi et de conserver la procédure en vigueur pour aller au-delà de 50 territoire un amendement sénatorial allant dans ce sens ont été déclarées irrecevables, c'est pourquoi je profite de cette prise de parole pour connaître, Monsieur le Ministre, votre point de vue pour la suite de l'expérimentation, remercie pour votre écoute. soulever quelque part à un problème de méthode avec avec ce gouvernement qui en dit long finalement sur sur une pratique politique, c'est-à-dire que vous proposer une loi pour détricoter l'assurance chômage qui vient en aide aux plus fragiles, un projet que vous dites s'inspirer du du Canada, vous n'avez fait aucune consultation dans le pays concerné pour étudier les impacts des réformes que vous souhaitez vous inspirer, vous n'avez pas consulté, le gouvernement canadien, vous n'avez pas consulté les syndicats, mais ça, je ne vais pas vous jeter la Pierre, vous voulez consulter pas en France non plus, un peu trop vous demander de faire ça, donc c'est quand même problématique de comme démarche politique quand on propose un texte que qui est censé s'inspirer d'un autre pays, je vous dis ça parce que je reviens justement d'un déplacement au Canada, ou j'ai pu, moi, faire ce travail d'échanges avec les personnes qui sont directement concernés par ces réformes et ça a été très bien dit par mes collègues auparavant les conséquences et diminution de pension précarisation précarisation accrue et mon d'ailleurs remis un livre que je vais vous donner tout de suite après, comme ça vous pourrez vous même l'étudier sur le Mouvement action chômage de Montréal, une petite histoire des luttes pour le droit à l'assurance chômage, comme ça, vous allez vous apercevoir, c'est quoi les réformes Nello néo-libérale que vous promeuvent promeuvent en France ce que ça donne concrètement sur la situation des gens et plus moi je, je souhaiterais que vous inspirer de d'autres choses qui se passent dans ces pays-là, par exemple, il y a des réformes qui sont faites dans les provinces canadiennes pour faire face justement en pénurie d'emplois, ça s'appelle la semaine des 4 jours dans un pays libéral, ça c'est bizarre, rien n'est évoquée par rapport à par rapport à ça, donc moi ce que je vous appelle, c'est plutôt de, de, de, de revenir bien sûr de d'accepter les amendements que nous, nous proposerons pour améliorer ce texte qui va précariser un peu plus déjà les gens qui sont les plus vulnérables, dans notre société. Madame Benbassa. Est inscrite sur l'article. vous attendez que l'on vous donne tout pouvoir d'agir sur les règles qui régissent l'assurance chômage, vous nous dites, Monsieur le Ministre vous soucier des actuels bénéficiaires car sans ce texte, il ne pourrait plus percevoir leurs droits, l'urgence dont vous nous faites part n'impose nullement que l'on vous donne une telle liberté d'action, d'autant plus que cette urgence relève de votre responsabilité de votre incapacité de concertation, de votre inaction, vous nous dites, Monsieur le Ministre, vouloir dynamiser le marché de l'emploi, votre solution Andy guillemets inciter je vous cite les demandeurs d'emploi à accepter tout top, parce qu'il ne serait pas assez motivés, or pour les organisations syndicales et patronales qui, pour vous, non, visiblement pas leur mot à dire l'état du marché du haut trop bas niveaux de rémunération aux conditions de travail non adaptés ou encore en manque de qualification, vous devriez aller écouter davantage et prendre en considération leur évaluation de l'état du marché encore une fois, vous leur répondez hors sujet pour preuve selon le Pôle emploi 92 % des demandeurs cherchent activement un travail, parmi eux, plus d'un quart ne demande pas leur droit à l'indemnisation, la réalité est que tant de personnes se trouvent en situation de grande précarité, monsieur le Ministre, on attend de l'exécutif des solutions pratiques et non des constatations théorique, qui ne sont pas celles du terrain et qui risque d'aggraver davantage la situation du marché du travail et des travailleurs au chômage, merci. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, ce cet article 1er nous nous pose on pose problème et nous pose question, vous avez lancé des concertations avec les partenaires sociaux, bon déjà je je ne comprends pas très bien, vous m'avez donné une réponse en commission mais qui ne m'a pas convaincu, pourquoi vous avez attendu vraiment la fin le dernier jour le le danger pour les demandeurs d'emploi de ne plus être indemnisés pour relancer la machine, vous avez lancé des concertations avec les partenaires sociaux, mais dans un cadre extrêmement strict et à nous, parlementaires, finalement, vous nous demandez de vous signer un blanc-seing une fois que ce texte sera voté, il y aura quand même beaucoup de zones d'ombre et et et nous ne pouvons pas finalement vous donner, donner la possibilité au au au au gouvernement d'ériger des règles

une bien évidemment aux partenaires sociaux la 2ème chose que je voudrais dire, c'est que dans une des motivations que j'ai entendu ici ou là pour faire une réforme à marche forcée, on nous dit que l'Unédic, les finances de l'Unédic serait en danger, or le dernier rapport qui nous a été envoyé, la semaine dernière par l'Unédic, nous dit que les comptes de l'Unédic sont excédentaires à cette année le seront l'année prochaine et le sera encore l'année d'après,

et enfin sur un sujet différent, mon collègue, le sénateur Mulligan a parlé, je fais partie de ceux qui ont déposé un amendement pour territoire zéro chômeur, je ne comprends pas très bien pourquoi il a été déclarée recevable puisque le titre du projet de loi, c'est le fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi et nous avons beaucoup de gens qui attendent donc effectivement, effectivement, comme mon collègue, je vous demanderai de de nous dire ce que l'on peut envisager, merci. Merci monsieur le président, pardon pour mesdames et messieurs les sénateurs, si je ne répond pas dans l'ordre des des interventions mais je voudrais simplement dire, en écho à ce que dit Madame lui ben à l'instant que si nous avons fait le choix du calendrier qui qui ont réuni aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure parce que si nous avions respecté parfaitement. L'enchaînement des négociations et de la recherche d'un accord national interprofessionnel, il aurait fallu ouvrir cette négociation sur la base d'une lettre de cadrage, comme prévu par la loi de 2018 au moment de l'élection présidentielle et nul doute Madame Lubin que vous nous auriez reproché dans cette période là, de ne pas être suffisamment légitime pour ouvrir une telle négociation sur un sujet aussi important, c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix que nous assumons, de ne pas ouvrir cette négociation et donc aujourd'hui de vous proposer de proroger pour 14 mois et 14 mois seulement les les règles en ajoutant la la question de de la modulation c'est ça qui qui motive ce calendrier et qui motive cette remarque, j'en profite pour vous remercier, madame l'humain puisque vous l'avez dit à l'instant, les résultats, l'Unédic sont bons et c'est tant mieux, c'est à la fois le fruit de la reprise de l'emploi, c'est aussi le fruit de la réforme de 2002 2019, et je n'ose pas voir une forme de satisfecit de votre part à la réforme de 2019, mais comme l'objectif était de sortir d'une période où le déficit structurel de l'Unédic était de 2009 par an la perspective un excédent à 4 milliards IV est plutôt une très bonne nouvelle et de, je crois, nous nous rassurer toutes et tous un un mot pour dire en en écho à ce que disait madame la sénatrice Benbassa que que je ne vois plus, je crois qu'elle est partie, dire que, évidemment, que nous cherchons à être pragmatique, nous cherchons à apporter des solutions les plus concrètes possibles, c'est la raison pour laquelle quand Madame la rapporteure propose de mieux encadrer, de mieux sécuriser le dispositif d'abandon pour permettre à à telle ou telle salariés en situation de maltraitance en situation de harcèlement, de pouvoir faire valoir ce droit et ainsi de pouvoir procéder à un abandon de poste de manière protégé nous souscrivons au Cadre qui est ainsi mis qui peut ainsi protéger tous tous types de de salariés, enfin sur les questions relatives à territoire zéro chômeur évoqué par Monsieur Mounier, madame la sénatrice, je n'ai pas à me prononcer sur la recevabilité d'un amendement devant le Sénat de la même manière que je n'ai pas à me prononcer, je ne, je ne me suis pas prononcé sur la même recevabilité opposée au même amendement par l'Assemblée nationale, que ce soit au titre de l'article 40 ou de l'article 45 pour ce qui concernait l'Assemblée nationale, ce que je peux dire, par ailleurs, c'est que le projet de loi de finances pour 2023 prévoit un budget pour territoire zéro chômeur qui passe de 29 ans, pardon, de nous augmentons les crédits consacrés à cette expérimentation pour suivre le rythme de la labellisation par ailleurs l'intégralité des territoires qui m'ont été proposées, la labellisation par le comité scientifique présidé par Louis Schweitzer, ont fait l'objet de cette labellisation j'ai encore signé un arrêté il y a quelques semaines, voire même quelques jours pour se faire, et nous ne sommes pas encore au soixante, nous sommes plutôt autour de 39 peut-être 42 parce que les 3 derniers que j'ai signé, je ne sais pas s'ils sont dans les 39 en plus des 39 nous avons dans la loi de 2020 une disposition qui prévoit une une une évaluation de cette expérimentation, et c'est aussi à cela que l'année 2023 de têtes consacré cela d'ores et déjà fait l'objet d'échanges entre mon cabinet, les équipes de l'association d'autres partenaires comme France Stratégie et donc nous devons procéder à cette évaluation pour faire en sorte que si cette évaluation est concluante, nous puissions continuer à la développer si elle nécessite des ajustements que nous puissions procéder aux ajustements mais aujourd'hui nous avons encore un peu de marge entre le nombre de territoires labélisés et le nombre plafond qui est fixé à 60, dispute cinquante et nous avons par ailleurs au budget 2023 les crédits pour accompagner cette expérimentation. Merci, Monsieur le Ministre, donc nous commençons les amendements et nous avons pour démarrer 2 amendements de suppression, les 12 et 46 qui vont être présenté d'abord par Madame Merci monsieur le président, dans l'esprit de, de, de ce que je viens de vous dire, cet amendement vise à abroger la précédente réforme de l'assurance chômage et à supprimer l'article 1er de ce projet projet de loi, la réforme de l'assurance chômage s'est fait contre les partenaires sociaux, les syndicats engageant même des contentieux devant le Conseil d'État et la publication par l'Unédic d'une étude d'impact des décrets n'est pas de nature à apaiser les relations entre les partenaires sociaux et le gouvernement, qui s'était bien gardé de communiquer ses évaluations des effets de la réforme qui entre en vigueur au fur et à mesure, baisse de l'allocation journalière de 17 % en moyenne, la première année pour un 1000000 150000 allocataires les conditions d'affiliation sont durcies, avec notamment l'alignement du rechargement des droits sur les entrées dans le régime, les modalités de calcul de la durée du montant de l'indemnisation sont remises à plat une dégressivité remis en place pour les chômeurs de moins de 57 ans, percevant précédemment au moins 4500 euros brut par mois, une taxe forfaitaire est prévu pour les CD CDD et un bonus-malus sectorielles instauré, elle a touché les territoires les plus défavorisés de notre pays, 30800 personnes à la Réunion dans 9200 jeunes de moins de 25 ans 33000 personnes en Seine-Saint-Denis, dont 8100 jeunes de moins de 25 ans 50400 personnes dans le nord, dans 17300 jeunes de moins de 25 ans, et elle est budgétairement inutile puisque le le jour, je ne vais pas redire ce que je viens de dire sur les comptes de l'Unédic.

fait perdre 155 euros par mois à plus d'un 1000000 d'allocataires et qui a exclu 450000 personnes du bénéfice de l'allocation chômage surtout l'article 1er confie les pleins pouvoirs à l'État sur la définition des règles d'indemnisation chômage, jusqu'au 31 décembre 2023 la commission des affaires sociales a effectivement avancé la date au 31 août mais cela demeure néanmoins sur le fond, une reprise en main par l'état d'une compétence délégué réservé depuis 58 aux organisations syndicales et patronales d'ailleurs l'article près ne prévoit pas seulement la prorogation des règles d'indemnisation chômage de 2000 19 mai ouvre aussi la possibilité de modifier les critères d'indemnisation, ce qui ne peut que nous inquiéter le gouvernement a tenté de ma de de le masquer, mais finalement, a été contraint d'afficher son projet de moduler à la baisse l'indemnité chômage selon la conjoncture économique, l'ensemble des organisations syndicales rejettent ce projet, vous le savez, la CGT, la CFDT, Force ouvrière, la CFTC et la CFE-CGC, mais également l'association patronale des entreprises de proximité vous mes chers collègues, droite de l'hémicycle, qui était très sensible à la voix des entrepreneurs, vous devriez les écouter parce que nous rejetons cette OPA de de l'État, nous demandons la suppression de l'article premier, je vous remercie. Merci monsieur le le président donc, effectivement, ce sont des Allemands de suppression de l'article premier simplement rappeler que cet article 1er a 2 objectifs : le 1er objectif c'est de donner une base légale et réglementaire à l'indemnisation des demandeurs d'emploi à compter du 1er novembre 2000 22 et le 2ème article effectivement ses d'autoriser temporairement temporairement, le gouvernement a fixé par décret, décret, les règles d'assurance chômage en dérogeant à la gouvernance prévue par le code du travail, alors nous avons fait un autre choix, hein, vous le savez, chers collègues, nous avons fait le choix en ce qui concerne la commission effectivement de d'accepter que le gouvernement proroge le décret de carence de 2019 pour sécuriser les règles de l'assurance chômage à compter du 1er novembre 2022, mais nous avons aussi fait le choix de déroger à titre temporaire à la loi de 2018 pour qu'effectivement redonner la main aux partenaires sociaux et c'est le le choix que nous avons fait en l'occurrence de quoi c'est un avis défavorable pour ces 2 amendements. Madame Lienemann, demande la parole pour une explication de vote. j'ai pas l'impression que vous nous ayez donné de réponse sur la manière dont le gouvernement souhaitait traiter cette expérimentation on veut aller vers le plein emploi, il y a des choses qui marchent et on dit nous ça, j'ai même pas comprendre, deuxièmement dans dans le le dans cet article, et d'ailleurs dans la précédente réforme qui est ainsi validée, on peut quand même remarquer l'obsession de toujours faire pression sur les salariés et sur les chômeurs, et dès qu'il s'agit d'obtenir un comportement correct des chefs d'entreprise et des entreprises, alors là on est mou du genou, on donne des délais on exonère plein de gens, on nous a expliqué que c'était un des arguments que madame Borne donner en permanence ici, c'est que cette réforme allait refaire reculer les CDD de courte durée, or on vient justement au mois d'actes d'octobre d'avoir le bilan, on se rend compte que pour les CDD d'un mois d'un mois, hein, c'est pas le Pérou, ils ont augmenté de plus de 5 % en un an, et deuxièmement dans l'hôtellerie restauration. Les CDD de moins d'un jour fada jour quoi de moins d'un jour explose augmente à nouveau, alors on ne peut pas nous dire faut faire des efforts, d'un côté et de l'autre, il y a des droits et des devoirs, là le devoir du chef d'entreprise n'est pas respectée et vous continuez à avoir comme seule solution un déséquilibre entre les efforts demandés aux ça et se demander aux autres. Le monsieur le ministre, avant le vote. Merci monsieur le président, juste pour dire à Madame la Ministre que regarder le nombre de CDD proposés d'un mois ou plus d'un mois, est une chose, il a augmenté de 5 % le nombre de CDI par rapport à 2019 a augmenté de 50 % et c'est aussi cet accroissement très différenciées entre le nombre de CDI proposés à l'embauche pour les contrats de moins d'un mois de plus d'un mois, pardonnez-moi, et le nombre de CD qui compte et c'est ce qui explique que nous sommes passés pour les embauches sont des contrats de plus d'un mois de 46 à 52 % CDI dans la part des embauches, je pense qu'on peut aussi se féliciter de de ces résultats là. Bien donc je mets aux voix les 2 amendements de suppression qui est favorable.

Merci monsieur le président, c'est l'amendement que j'évoquais tout à l'heure, en réponse à la discussion générale qui permettrait de revenir à la fois des délais d'application de la loi allant jusqu'au 31 décembre 2023 je m'explique, en un mot sur ce point, nous avons au cours de l'année 2023 à mettre en place France travaille la préfiguration a été lancée, nous avons aussi à renégocier la convention tripartite entre l'État, l'Unédic et Pôle Emploi pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 et nous souhaitons dans le même temps hein mener la la la négociation tout cas ouvrir et permettre aux partenaires sociaux de mener la négociation sur la question de la gouvernance de l'assurance chômage, tout converge au 31 décembre 2023 et à une application au 1er janvier 2024 c'est la raison pour laquelle nous nous ne sommes pas favorables à la modification de la date butoir d'application du décret que nous sollicitons du Parlement la 2ème chose, c'est que nous sommes convaincus de la nécessité d'une négociation sur la gouvernance, mais dans le cadre prévu par les lois qui encadrent aujourd'hui actuellement, plus exactement, le dialogue social, donc c'est un rétablissement de la rédaction de l'Assemblée nationale que nous sollicitons par cet amendement. Merci Monsieur le Président, alors je vais me poser un peu sur cet cet amendement proposé par le gouvernement, voilà 60 ans, Monsieur le Ministre, que l'assurance chômage et géré par les partenaires sociaux, c'est un principe qui a plusieurs intérêts, entre autres, de dépasser aux réduire les antagonistes entre les partenaires sociaux, de rendre plus consensuel, le choix et surtout de donner du poids à la démocratie sociale, souvent un certain nombre de partis se pose la question de la différence entre le gouvernement, la majorité gouvernementale et la majorité du Sénat. La différence, elle est la suivante : vous dites être pour la gestion paritaire mais vous faites la loi de 2018 : que fait la loi de 2018, on l'a annoncé un certain nombre et un certain nombre de, de, de, de collègues l'ont dit tout à l'heure au perchoir que fait la loi 2018 : elle corps cette la négociation au travers la lettre de cadrage qui du coup a été un échec, immédiatement, on en a vu effectivement le résultat du reste, vous ne l'avez pas utilisé, même si il y avait effectivement un certain nombre d'enjeux calendaire qui ne vous ont pas permis de le faire, mais vous ne l'avez pas utilisé, donc vous-même vous avez considéré que la loi de 1018 ne permettait pas effectivement de donner donner la main aux partenaires sociaux. Et de surcroît vous supprimez la part sociale de la cotisation salariale ce qui, d'ores et déjà au sein de l'Unédic donne moins de poids aux représentants des partenaires sociaux au sein de la gestion de l'Unédic, qu'est ce que nous faisons, nous nous redonnant la main aux partenaires sociaux au travers un dispositif qui est un dispositif transitoire qui est très simple, qui s'inspire, qu'on ne l'a dit Pascale Gruny tout à l'heure de l'Arctique L 1 du code du travail sur un principe de concertation concertation d'orientation négociation c'est la seule façon de donner pleinement la la parole aux partenaires sociaux et de redonner la gestion de l'Unédic aux partenaires sociaux de la gestion de, de, de, de l'assurance chômage, je dirais que l'assurance chômage aux partenaires sociaux, voilà la différence entre vous et nous vous vous dites nous, on fait et voilà pourquoi nous sommes défavorables à votre amendement. Mais pour ce opposer parole sur cet amendement du gouvernement. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, l'amendement du gouvernement vise à rétablir, donc l'article 1er qui a été adopté par l'Assemblée nationale, je voudrais profiter de cet amendement pour rappeler à monsieur le ministre du travail que dans la présentation de la motion j'ai cité les pistes du gouvernement sur les critères de la modulation de l'indemnisation chômage, s'il est vrai que vous avez exclu jusqu'à présent de moduler le montant de l'indemnisation, et c'est heureux, vous avez présenté aux organisations syndicales et patronales l'option qui consiste à moduler les conditions d'accès à l'assurance chômage ainsi dans un article du journal Le Monde en date du 19 octobre 2022, le document de concertation et cité joli une modification du seuil d'éligibilité à l'assurance chômage ou de la période de référence de la filiation a un effet immédiat et rapide sur les entrées ainsi le gouvernement pourrait modifier ses critères en les passant à 6 mois travailler

Et ce qu'il y a d'autres demandes d'explications de vote, donc je mets aux voix l'amendement du gouvernement, l'amendement 94 avec un avis défavorable de la commission qui est. Qui est contre. Il y en a un peu plus, donc il n'est pas adopté alors de ce fait, je vous signale mes collègues un tunnel de 22 amendements en discussion commune, ce qui va demander un petit effort de concentration et de d'efficacité du dialogue madame mon je commence avec l'amendement 85. Merci monsieur le président, et la conclusion de la négociation, au mépris des principes du paritarisme, cette méthode anti-démocratique est permise depuis 2008 par le décret de carence qui donne au gouvernement des marges considérables au point que nous sommes ici à discuter du prolongement d'un décret qui ouvrent sur un autre où nous n'aurons pas plus que les organisations syndicales véritablement voix au chapitre, le régime logistique de l'assurance chômage s'apparente en conséquence, hein. 49 3 permanent pourtant profondément atteinte à la démocratie, nous refusons cet cet état de fait, c'est pourquoi cet amendement propose de supprimer la possibilité de légiférer par décret en cas d'absence d'accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux réinstaurant pleinement le paritarisme dans la gestion de l'assurance chômage, en conséquence, il se propose de revenir automatiquement à la dernière convention conclue par les partenaires sociaux, lorsqu'un régime de carence expire le temps d'organiser de nouvelles négociations donc. Le risque de vide juridique et donc résolu et le paritarisme réaffirmé en cohérence et en complément des ajouts de la commission des affaires sociales sur il y a peu, Emmanuel Macron, annonçait dans un discours fleuve l'urgence pour le gouvernement d'adopter une nouvelle méthode, plus respectueuse de la négociation et de la démocratie, nous vous donnons ici, Monsieur le Ministre, l'occasion de passer du discours aux actes.

lorsque le régime de carence aujourd'hui utilisée par le gouvernement, expire en fait le but c'est de revaloriser le dialogue social et empêcher le gouvernement de détricoter l'assurance chômage, nous proposons que lorsqu'un régime de carence arrive à expiration sans qu'une nouvelle convention n'ait été agréé l'assurance chômage soient régis par la dernière convention ayant donné lieu à un accord entre les partenaires sociaux, ainsi dans le cas présent, cela signifierait de revenir sur la réforme ayant diminué l'indemnisation de 1 15 1000000 d'allocataires pour cent cinquante-cinq euros en moyenne par mois par locataire et retarder l'ouverture des droits de près de 500000 assurés les estimations des économies générées par cette réforme avoisine les 6 5 milliards d'euros au détriment des salariés et des chômeurs. Madame Maryse Carrère. Merci monsieur le président, cet homme demain est quasiment identique au tout au moins il a le même objet, donc il sera défendu merci. Ensuite, madame mange reprend avec l'amendement 84. Merci monsieur le président, l'article 1 du projet de loi met le pied dans la porte d'une dérive anti-social au long cours, programmée par le gouvernement des réformes de l'assurance-chômage jusqu'à celle de la retraite, en passant par le RSA, je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil d'État lui-même nous alarme en rappelant, je le cite, que le projet de loi ne comporte aucune limitation indirect ou un ou Direct quant à l'objet ou à la portée des dispositions du futur décret en tant que législateur vous nous invitez à signer un chèque en blanc, sans qu'aucune étude évaluatif n'a été réalisée sur la réforme que nous sommes censés prolonger et sommes l'étude d'impact de l'Unédic, ça a été dit, qui veut, qui prévoyait que plus d'un 1000000 de personnes verraient leurs indemnités baisser et ce malgré le retard dans l'ouverture des droits pour des centaines de milliers de personnes malgré la pénalisation injuste et abrupt provoquée par le nouveau calcul du salaire journalier de référence pour tous les travailleurs, les saisonniers comme pour ceux qui bloqués dans la précarité, enchaîne les contrats courts, vous nous avez dit que vous venez tous sauriez plus le taux de remplacement a tellement baissé que vous pouvez effectivement ne plus le toucher la promulgation de ce texte permettra, après une concertation sans négociation une refonte unilatérale de l'assurance chômage, sur le modèle antisocial du Canada, donc on vous invite aussi à lire le livre, qui a eu pour effet sinon pour objet de faire chuter drastiquement le nombre d'allocataires dans ce pays et selon de nombreuses études de forcer les chômeurs à accepter des emplois aux conditions de travail dégradées et aux salaires bas, voire indigne la prise en tenaille entre la prolongation d'une d'une réforme antisociale et inefficace pour pousser au retour à l'emploi, quelle que soit sa qualité et le chèque en blanc d'une 2ème réforme n'est pas acceptable tant pour les partenaires sociaux que pour le Parlement, en conséquence, nous proposons la suppression de cet alinéa.

la réforme menée à l'heure à partir de 2019, c'est fait, je viens de le dire, contre les partenaires sociaux qui n'ont cessé d'alerter sur ses conséquences sociales, alors qu'une évaluation de l'impact de cette réforme n'est promise que pour fin 2020, 2024 les premières données font apparaître un une augmentation des chômeurs en catégorie B, C, D et une de une tension inédite sur le marché de l'emploi saisonnier provoquées par l'allongement de la durée d'affiliation soit un effet contre-contre-productif de votre réforme sur la tension du marché du travail une baisse des indemnités, faisant basculer, de nombreuses personnes dans la pauvreté, même sous l'angle de la réduction des emplois vacants, la réforme semble un échec puisqu'entre le 2ème trimestre 2021 et le 2ème trimestre 2022 les emplois vacants ont augmenté, passant de 264000 à 362000 selon l'adresse ne permettant pas de lutter contres les tensions sur le marché de l'emploi qui ont bien d'autres causes, malgré cela, le support de concertation que vous avez envoyé aux partenaires sociaux et clair dans l'intention du gouvernement d'intensifier la réforme en envisageant un nouvel allongement de la durée d'affiliation, une diminution de la durée d'indemnisation, accompagnant la baisse, on l'a dit, du taux de remplacement de la réforme précédente, voire une territorialisation de l'assurance chômage, sur le modèle du Canada, de plus en plus inacceptable, ce qui explique le refus d'une négociation préalable dans le respect du paritarisme et de la démocratie donc avec cet amendement, en conclusion, nous rétablissons l'obligation d'une négociation avec les partenaires sociaux incluant cette fois les associations représentatives de chômeurs et précaires, premiers concernés par les effets des réformes successives et qu'une démocratie vivante devrait intégré comme partie prenante, je vous remercie. Il y avait la parole pour l'amendement 77. Merci monsieur le président, donc il s'agit d'un amendement de repli, attachée à la gestion paritaire de l'assurance chômage, nous proposons de proroger les mesures actuellement en vigueur dans l'attente de la concertation avec les partenaires sociaux sur la gouvernance d'équilibres financiers et les règles d'indemnisation de l'assurance-chômage. Merci ensuite Madame Lubin, vous avez l'amendement 19 monsieur Jean 13. La hier. Oui, il s'agit d'un amendement de repli qui vise à rétablir la compétence des partenaires sociaux pour la période de carence que le gouvernement a lui-même créée en laissant filer les délais, comme l'a rappelé l'avis rendu par le Conseil d'État le 5 septembre 2022, le projet de loi ne comporte en effet aucune limitation directe ou indirecte, quant à l'objet ou à la portée des dispositions du futur décret et si les rapporteurs ont introduit un dispositif plus favorable au Paris paritarisme concernant la nécessaire évolution de la gouvernance de l'assurance chômage, ils n'ont pas touché à celui régissant le décret sauf pour réduire la durée durant laquelle le gouvernement pourra agir de son propre chef sur les règles d'indemnisation par l'assurance chômage, cela s'apparente donc toujours à la signature d'un chèque en blanc au gouvernement en piétinant le paritarisme, ainsi que le Parlement pour mémoire la réforme menée pendant le précédent quinquennat fut la première réforme menée contre l'avis des partenaires sociaux depuis 1971 le gouvernement ne peut pas, une nouvelle fois contourner le dialogue social par cet amendement, le groupe socialiste, écologiste et républicain entend redonner la main aux partenaires sociaux, y compris sur la période transitoire post-première novembre 1er novembre 2022 merci. La parole, mon cher collègue, pour présenter l'amendement 20 ou c'est madame. Notre amendement vise à conditionner la prise du décret en Conseil d'État à la transmission au Parlement et aux partenaires sociaux d'un rapport sur la gestion de l'assurance chômage, la loi du 5 septembre 2018 prévoit normalement que le gouvernement transmettre chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux, gestionnaires avant le 15 octobre un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, mais depuis 2018, ce rapport n'a pas été transmis le Parlement légifère, donc sans même qu'un bilan officiel de la précédente réforme de l'assurance chômage ait été réalisée et rendue publique, c'est sur la base de résultats factuels que de nouvelles règles d'indemnisation doivent pouvoir être réfléchie et mise en place, nous devons savoir précisément l'impact des règles d'indemnisation que le gouvernement a décidé par décret en 2019 sur l'accès à l'indemnisation, sur le retour à l'emploi sans bilan chiffré étayer, il n'est en effet pas possible de justifier de nouvelles règles, ce projet de loi en déplaçant le problème à l'échelle de la pseudo-responsabilité individuelle culpabiliser attriste du demandeur d'emploi réactif, tous les vieux stéréotypes sur le chômeur qui ne veut pas travailler qui refusent un CDI, ce faisant, il ouvre la voie à des mesures encore plus régressive de la part de la majorité sénatoriale. Merci monsieur le président, la droite sénatoriale se pose en défenseur du paritarisme, de l'assurance chômage, face au gouvernement qui souhaite décider seuls des règles d'indemnisation, mais prévoit une simple concertation entre les organisations syndicales cette concertation est une mascarade, comme le décrit bien le ministre du Travail, qui la voit comme un échange, une discussion, ce sont des propositions des contre-propositions et à la fin, le gouvernement prend les les décisions qu'il doit prendre le gouvernement invoque l'urgence de mettre en place un cadre juridique pour l'indemnisation des chômeurs, alors que c'est lui qui n'a pas envoyé avant le 29 juin la lettre de cadrage aux organisations syndicales, c'est lui qui décide de ne pas simplement prorogée, la réforme de 2019, c'est lui qui a fixé au 31 décembre 2023 l'habilitation à décider seul des règles d'indemnisation chômage, le président de la République avait annoncé, revenir à un fonctionnement plus horizontal et moins vertical notre amendement remplacer la concertation prévue à l'article 1er pour discuter de la modification des règles d'indemnisation chômage par une véritable négociation sociale ou la vie des partenaires sociaux, n'est pas simplement consultatif mais obligatoire avant de réformer l'assurance chômage, le gouvernement se comporte comme un banquier qui déciderait de venir s'installer dans notre maison et de fixer les règles sur l'utilisation de la température des radiateurs, je vous remercie.

Ah pardon, pardon, je je sautais une ligne le le vingt-et-un donc chez Madame fournir le pardon. Merci Monsieur le Président, cet amendement va effectivement dans le même sens et les termes de sémantique ayant leur importance il cet amendement vise à remettre au centre de la démocratie sociale, la négociation avec les partenaires sociaux plutôt que de mettre l'accent, comme le fait le gouvernement sur une concertation qui n'a pas du tout le même sens : le paritarisme et le dialogue social implique un cadre d'échanges, tels que les partenaires sociaux via leurs prérogatives reconnues et c'est cela la négociation, il en va donc du respect de la philosophie qui a présidé à la mise en place de l'assurance chômage, les rapporteurs sont d'aller en ce sens en supprimant la lettre de cadrage dans la procédure de négociations des accords sur l'assurance chômage et en fixant un cadre transitoire discussion plus favorable au paritarisme, nous leur proposons d'aller plus loin, en exigeant une négociation également pour cette période de carence à venir. madame Monge maintenant pour l'amendement 90 avec mes excuses. Oui, merci Monsieur le Président, alors c'est un peu redondant, mais c'est quand même très, très important ce passage des amendements, car le gouvernement temps peut-être faire de la concertation, le principe qui devraient guider la construction de toutes ces politiques publiques mais le droit du travail n'est pas une affaire de concertation, c'est une question de négociation. Les partenaires sociaux ne sont pas des instances à seulement consulter ce sont les interlocuteurs privilégiés de la négociation collective, garante du paritarisme, d'une connexion réel avec les personnes concernées et de la protection des droits des personnes en recherche d'emploi, comme nous l'avons dit en s'autorisant à prendre par décret sans réelles négociations avec les partenaires sociaux, de nouvelles règles pour l'assurance chômage, le gouvernement peut facilement outrepasser le gouvernement peut facilement outrepasser tant les oppositions à sa lettre de cadrage que demain à son support de concertation et imposer une réforme sans respecter les principes du débat démocratique et du dialogue social, c'est inacceptable en démocratie, comme l'écrivait Rousseau dans le contrat social, le Peuple soumis aux lois doit en être l'auteur de sorte qu'un régime n'est démocratique que si les personnes concernées par les lois n'en sont pas exclues et ne sont pas exclus de la fabrique de la loi, la prise en compte par des procédures démocratiques des positions des travailleurs, qu'ils soient actifs ou privés d'emploi, des agents de Pôle dans emploi et donc primordial pour la mise en place de réformes efficace et protectrice, dès lors, les modifications envisagées par décret dans cet article doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation, je dis bien une négociation avec les partenaires sociaux, c'est l'objet de l'amendement.

ne pouvons pas évaluer objectivement et de manière exhaustive la précédente réforme puisque nous n'avons pas reçu les éléments. ensuite l'amendement 93 de Madame Poncet mon jeu. Il la parole. Merci monsieur le président, alors dans son support de concertation envoyé aux partenaires sociaux le ministère, le ministère du Travail envisage la possibilité d'appliquer une régionalisation du régime d'assurance chômage, en prenant l'exemple du Canada où un tel dispositif a été introduit en 1977 amplifié depuis l'heure au Canada est corrélée à une augmentation de la durée d'affiliation à une baisse de la durée d'allocation le modèle canadien n'a eu pour effet que de faire chuter continuellement le nombre de personnes éligibles, assurance chômage, écoutez bien, qui est passé de 87 % en 1989 à 42 % en 1997 son instauration en France, couplé aux mesures de durcissement, d'accès à l'assurance chômage ne manquera pas d'avoir les mêmes effets, la régionalisation est vertement critiqué comme inéquitable au Canada, en France, le dynamisme de l'emploi n'a rien à voir entre les différentes régions, mais le nombre d'offres d'emploi doit pour doit, pour doit, pour chaque territoire et rapporté à celui des demandeurs d'emploi de plus, sauf à ne pas tenir compte des compétences et des qualifications, les offres comme les demandes d'emploi peuvent nécessiter d'ampleur reconversion et formation avant de s'appareiller, rien ne devrait justifier une inégalité de traitement entre les demandeurs selon les régions et ne devrait même pas être à l'étude, compte tenu des conséquences négatives qu'ils ont eu au autant au Canada d'ailleurs qu'aux États-Unis et qui par ailleurs n'ont rien résolu, je l'ai déjà dit des tensions sur le marché du travail mais multiplié par contre oui, les employes de mauvaise qualité et de piètre productivité du travail, sauf à introduire un nouveau parrain maître durcissant les droits encore et toujours pour les chômeurs, donc, cet amendement vise à exclure la possibilité pour le gouvernement d'inclure la régionalisation par décision unilatérale dans le nouveau décret prévu dès début 2023. Ensuite, nous l'écoutons l'amendement numéro 50 présenté par Madame hein, pour se et Madame Cohen, présentée par Marie-Noëlle Lienemann. au décret enfin que le décret s'arrête le 31 décembre au 31 août nous, nous proposons que ce soit le 1er février en fait, c'est pour dire que nous ne souhaitons pas je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que c'est pas une petite décision vous l'avez dit madame la la rapporteure, c'est notre modèle social issu de l'après-guerre. Qui est petit à petit des tricoter dans ses fondements, pas seulement dans les mesures mais dans ses fondements, c'est le : la démocratie sociale, c'était la réponse française à une meilleure association du monde du travail et des entreprises aux décisions qui les concernent, c'est une certaine vision de la société et là maintenant c'est fini ça, l'État reprend la main et l'État avait quand même beaucoup la prérogative financière philosophiquement la cotisation le l'indemnisation est un droit lié à la mutualisation des cotisations, ça n'est pas une aide sociale qui est donné au de la solidarité nationale et ça change beaucoup parce que tout le discours sur l'assistanat et cetera vise à tout confondre : non, il y a des droits acquis par les salariés dont le cadre est décidée par la négociation sociale entre partenaires sociaux, ça n'est pas une assistance versés par la solidarité nationale et c'est à force de faire ses petites réformes ont fini par glisser vers tous ceux-là qui finit par trouver illégitime, ce qui est un droit et qui fait reculer l'idée même que les salariés se font de la reconnaissance de la société française. L'amendement numéro 7 c'est Madame Mellow qu'il présente. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, là le l'amendement que je vais vous présenter de mon collègue Emmanuel Capus est une version de compromis, en effet, en commission, le délai limite au terme duquel les règles actuellement en vigueur, devront être révisés a été ramené de fin décembre 2023 à août 2023, or le rallongement de ce délai, telle que prévue par le gouvernement, a pour objectif de mieux prendre en compte les les effets, les effets de ces règles ainsi indépendamment du mode de détermination des futures règles qui succéderont aux règles actuelles, il apparaît judicieux de conserver un délai suffisamment long pour permettre la collecte des données ces données permettront de mieux évaluer l'efficacité de ces règles et donc de prendre des décisions plus éclairées le moment venu, c'est l'objet de cet amendement.

pour les entreprises recourant excessivement aux contrats courts et précaire, c'est un amendement important et nécessaire au vu de la refonte du bonus-malus déjà engagés par les rapporteurs, il est d'ailleurs le pendant de la suppression de ce dispositif de minorité de minoration introduit à l'article de. Merci l'amendement 108 et présenté par Madame Poncet mon jeu. Merci monsieur le Président, c'est un amendement relatif aux saisonniers, car depuis la mise en place de la dernière réforme de l'assurance chômage, prolongeant notamment la durée d'affiliation les constats se multiplient, montrant l'impact négatif de la réforme de l'assurance chômage sur les saisonniers, dont les emplois sont par définition plus court, voire discontinue si la modification de la durée minimale d'affiliation requise pour ouvrir des droits à indemnisation, passant de 4 à 6 mois a profondément amoindri leurs droits, le support de concertation envoyé aux partenaires sociaux, poursuit cette fuite en avant de la réduction des droits puisqu'un allongement de la durée d'affiliation et de nouveau évoqué et envisagé cet allongement et la prise en compte des jours non travaillés entre 2 emplois saisonniers dans le calcul, dès lors, forcément à la baisse du salaire journalier de référence s'est avéré contre-productif pour l'attractivité de secteurs concentrant les emplois saisonniers et accru leur pénurie cet été ça été documenté et donc la tension sur le marché du travail, ces emplois sont déjà caractérisé par une intensification massive du travail de dures conditions de travail très très mal très mal pris en compte dans les rémunérations, donc la réforme de l'assurance chômage introduit donc une double peine pour les travailleurs saisonniers beaucoup de travailleurs ont vraisemblablement été contraint de se réorienter vers d'autres activités et cet amendement vise donc à la prise en compte des spécificités de ces travailleurs et oblige à des négociations entre les représentants des salariés concernés et le gouvernement afin d'aboutir à un accord spécifique et mieux adapté pour les travailleurs saisonniers. Merci monsieur le président, le fonctionnement donc actuel de l'assurance chômage permet au gouvernement et au patronat de se passer des organisations syndicales, en effet, si les négociations entre les partenaires sociaux pour définir une nouvelle convention a chope le gouvernement peut imposer par décret les réformes que le patronat, lui souffle évidemment à l'oreille, ce texte n'est que l'aboutissement depuis 2018 de la loi avenir professionnel, contre laquelle nous avions voté après avoir déduit réduit les capacités des de décisions des organisations syndicales, en encadrant toujours davantage les prérogatives du paritarisme, ce projet de loi transfère directement à l'État, la gestion de l'Unédic, nous pensons à l'inverse, que les syndicats de salariés ont toute leur place dans l'élaboration des normes régissant l'assurance-chômage, notre amendement propose de revenir automatiquement à la dernière convention conclue par les organisations syndicales et patronales lorsque le régime de carence expire cette disposition empêchera les gouvernements de jouer la montre pour justifier la reprise en main des règles d'indemnisation chômage, je veux remercier. Vous avez à nouveau la parole, cher collègue, pour présenter l'amendement numéro 49. Merci monsieur le président, donc, selon le maître de conférences en sociologie de l'Université Lorraine Jean Pascal il gelait la réforme de l'assurance chômage est un déni de solidarité au au-delà de la diminution des indemnités des plus précaires, le gouvernement vise à transformer une assurance collective en n'épargne individualisé notre amendement vide un vise à inscrire dans la loi le caractère assurantielle de l'assurance chômage et sa vocation à sécuriser le revenu des travailleurs et des travailleuses en imposant des taux de cotisation différent selon les entreprises et les secteurs et en différenciant les règles d'indemnisation pour les plus hauts salaires la réforme détricote la solidarité interprofessionnelle selon les laquelle les employes se payent pour ceux qui subissent le chômage, de même la dégressivité des allocations des chômeuses et les chômeurs les mieux payés, sépare les intérêts des plus aisés et des autres, le risque est donc que les particularités de chacun finisse par des délégitimer toute solidarité que finalement les mieux rémunérés et les plus stables ne veuille plus payer pour les plus précaires, le chômage ne devrait donc qui a risques individuels face à cela, il est urgent de renouer avec la logique de solidarité salariale interprofessionnelle garantissant chacun et chacune, contre le risque social du chômage telle et le sens de notre amendement, je vous remercie. Entendu Madame Monge présente l'amendement 87. Merci monsieur le Président, alors l'article 1 du projet de loi telle que modifiée par la commission des affaires sociales du Sénat présenté une avancée pour le paritarisme au milieu d'un vaste projet antisocial en ce qu'elle supprimait la lettre de cadrage instaurée en 2018. Celle-ci avait pour effet de contraindre le dialogue social avec les partenaires sociaux et de décider du périmètre des thématiques à aborder lors des négociations, dès lors, les partenaires sociaux ne pouvaient plus décidé des règles de l'assurance chômage, mais simplement de leur modulation à la marge de quelques paramètres cela permettait au gouvernement de faire échouer les négociations afin de légiférer par décrets sans contrôle des partenaires sociaux, comme ce fut le cas en 2019 pourtant, la suite de cet article reste flou puisqu'elle instaure en lieu et place de la lettre de cadrage, un document d'orientation aux objectifs mal définis et qui, bien qu'elle puisse être utile, hein, l'information du Parlement arrive bien tard puisque le support de concertation indiquant avec précision les projets de réforme du gouvernement, a déjà été envoyée aux partenaires sociaux la concertation et non la négociation est donc déjà lancée et les orientations du gouvernement sont déjà connus, si donc nous partageons la suppression de la lettre de cadrage instaurée par cet article et que nous défendons la mise en place immédiate de réelles négociations et non de concertation avec les partenaires sociaux, il semble que le document d'orientation, instaurée par le 3 de l'article 1 arrive un peu tard et qu'ils sont trop similaires à la l'aide de âge donc ce que cet article supprimé à juste titre et nous proposons donc aussi de le supprimer. Merci, cher collègue, il a, c'est à nouveau à Madame pour ce polie pour la présentation de l'amendement numéro 48 ou de Madame Lienemann qui a la parole. Oui ben c'est un amendement qui reprend des thèses développées par d'autres collègues, puisque nous refusons la modulation entre territoires et entre régions car nous considérons que c'est une remise en cause fondamentale de l'égalité républicaine, d'autant plus que comme on l'a dit, c'est une question de cotisation globale sur les sur l'État-Nation puis alors. Où va-t-on s'arrêter parce qu'alors on va dire : ah ben non, mais dans la région, c'est pas homogène ah donc le taux de chômage, il n'est pas le même en Seine-Saint-Denis que dans le centre de Paris, donc on va encore modulée des sous, modulation décider au nom de quoi bref, je crois que dans cette période où nous avons besoin d'une République solide où nous avons besoin que nos concitoyens, ce sont tous traités à égalité cette régionalisation de la d'amnistie chômage est totalement inacceptable, injuste et inefficace, on ferait mieux de réinventer des politiques d'aménagement du territoire pour créer de l'emploi, de manière plus équilibrée sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, le dernier de la série et présentée par nos collègues du groupe indépendant Monsieur Lagourgue un peu la parole. Merci monsieur le Président, en commission, le rapporteur en propose une nouvelle rédaction de l'article 1er qui accélère le retour à une gestion paritaire du régime, cette option a le mérite de mettre les partenaires sociaux en situation de responsabilité puisqu'ils redeviendront décisionnaire concernant le pilotage du régime concrètement ce retour au paritarisme de gestion se matérialise par le retour à un document d'orientation par opposition au document de cadrage cependant une telle option ne suffit pas à résoudre le problème, les problèmes qui se poser aux partenaires sociaux avant que le gouvernement ne décide lors du précédent quinquennat de reprendre la main sur le pilotage du régime, notamment pour ce qui concerne la capacité à prendre des décisions responsables pour garantir l'équilibre financier financier du régime, or l'avenir du paritarisme de gestion dépend de la capacité des partenaires sociaux à assurer l'équilibre financier des organismes dont ils ont la gestion, c'est pourquoi cet amendement vise à préciser que le document d'orientation prévue par la nouvelle rédaction de l'article 1er indique que les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options possibles transmis par le gouvernement doivent également visé à garantir l'équilibre financier du régime. Merci, cher collègue donc madame la rapporteure, vous avez la présentation de la ville, la commission sur l'ensemble des amendements. Merci monsieur le président, leur si si mes collègues en sont d'accord, je vais ramasser les amendements par sujet parce qu'il y a beaucoup de sujets qui se recoupent je je ne citerai pas tous les collègues qui ont déposé des amendements, hein, c'est pas irrespectueux, mais c'est plutôt pour, par souci d'efficacité et et du coup peut être aussi que je serais pas dans l'Ordre des amendements mais chacun réussira ah si, à s'y retrouver, sous les rédactions différentes des amendements 85 18 76 et 67 propose qu'un accord continue d'être applicable, même après son expiration jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu l'amendement 85 supprime le décret de carence ces 4 moment ces quatre amendements aurait pour effet de rendre la procédure inopérante permettant le maintien d'une convention d'assurance chômage, sans limitation de durée, s'il n'y a pas de conclusion d'un nouvel accord ce qui ce qui aboutirait à l'heure à un blocage de la gouvernance et priverait de toute possibilité de fixer des règles par décret par décret de carence en cas d'échec des négociations, ce qui présente un risque pour l'indemnisation des demandeurs d'emploi en l'occurrence c'est un avis défavorable de la commission pour les 85 18 76 et 67, l'amendement 84 supprime la ligne A or l'intervention d'un décret est rendue nécessaire pour sécuriser dès le mois de novembre, le versement des allocations chômage, nous en avons déjà parlé en ce qui concerne la position de la commission, c'est donc un avis défavorable sur le 84, les amendements 77 et 19 souhaite que le décret ne puisse prolonger que les règles déjà en vigueur, c'est-à-dire celles issues du décret de carence de juin 2019, il ne faut toutefois pas exclure que certaines évolutions des règles d'indemnisation soit nécessaire dès l'intervention de ce décret par exemple l'introduction des des règles contracyclique dont nous avons déjà parlé, c'est donc un avis défavorable sur les 77 et 19 l'amendement propose que le décret prévu à l'article 1er soit pris après la transmission au Parlement et aux partenaires sociaux du rapport élaboré par le gouvernement sur la situation financière de l'assurance-chômage, le code du travail prévoit déjà que ce rapport soit transmis annuellement Parlement et aux partenaires sociaux, c'est donc une demande de retrait, comme nous l'avons proposé en commission ou à défaut un avis défavorable sur le vin sur les amendements, amendements identiques 21 et 90, ainsi que sous des rédactions différentes les amendements 86 47 et ils ont tous pour objectif que les règles fixées par décret soit précédé d'une négociation et non d'une concertation, je rappelle qu'une négociation doit se conduire pour la conclusion d'un accord, elle est donc pas adapté au recueil de l'avis des partenaires sociaux avant de prendre un décret, c'est pourquoi l'article 1er prévoit une concertation préalable à la prise du décret, c'est donc un avis défavorable sur les 21 90 86 47 et 108 concernant l'amendement 22, il est sans doute pas nécessaire d'ajouter la transmission d'un rapport aux partenaires sociaux et Parlement avant la prise du décret sur les règles d'indemnisation, les effets de la dernière réforme qui n'est pleinement entré en vigueur qu'en 2021 sont encore partiellement connus le cadre de négociations qui a été fixé par la Commission pour l'année 2023 sera sans doute plus approprié pour recueillir via le document d'orientation du gouvernement un diagnostic, un diagnostic sur la réforme, c'est donc un avis défavorable sur le vingt-deux l'amendement 93 exclu la possibilité pour le décret de prendre des mesures qui créerait une différence de traitement entre allocataires en fonction de leur lieu de travail ou de résidence, nous pensons notamment notamment que le principe de contrat cyclicité des règles d'indemnisation est souhaitable et que ses modalités pour être dès le décret prévu à l'article 1er c'est donc un avis défavorable sur le 93 sur l'amendement la commission a déjà avancé au 31 décembre du 31 décembre au 31 août 23 la date limite pour l'application des règles qui seront fixées par décret, avancer cette date au 1er février ne laissera pas le temps suffisant aux partenaires sociaux d'engager une concertation sur la nouvelle gouvernance du régime puis de négocier un accord, c'est donc un avis défavorable sur le à contrario, l'amendement 7 rétabli la date du 31 décembre alors que la commission a avancé au 31 août la date de fin d'application du décret ne souhaitons pas que le gouvernement s'écarte pour une durée excessive de la gestion paritaire du régime, j'ai eu l'occasion d'en parler, l'horizon du 31 août 23 nous semble donc suffisant pour qu'une une concertation puisse être engagée sur la gouvernance avant une négociation en vue de la conclusion d'un accord, c'est donc un avis défavorable sur le site sur l'amendement 23 qui exclut la possibilité pour le décret de fixer des règles relatives au bonus-malus qui aurait pour effet de réduire les recettes de l'Unédic, le dispositif est actuellement neutre financièrement, la commission a limité la durée d'application des mesures prises par décret, il a souhaité recentrer le bonus malus sur les contrats courts, la précision proposé ne nous semble donc pas nécessaire, c'est donc un avis défavorable sur l'amendement 23 sur l'amendement 49 qui supprime le quatre transitoire de concertation et de négociation des partenaires sociaux, qui a été introduit par la commission et qui souhaite également ajouter des dispositions de portée déclaratoire visant à inscrire un principe de solidarité face à la privation d'emploi, ce dispositif ne semble être très générales et ne pas apporté ni ne retirer aucune garantie aux demandeurs d'emploi, c'est donc un avis défavorable sur le quarante-neuf sur l'amendement 87 qui supprime aussi le cadre transitoire de concertation et de négociation des partenaires sociaux, qui a été introduit par la commission, c'est donc un avis défavorable sur cet amendement 87 quarante-huit, il ne ne semble pas utile de préciser que le document d'orientation, élaboré par le gouvernement en vue de la négociation ne pourra traiter différemment les demandeurs d'emploi en fonction de leur lieu de résidence ou de travail, nous considérons que le document d'orientation, poser des éléments de diagnostic et identifier des pistes possibles mais pas de contrat à la négociation, c'est donc un avis défavorable sur le 48 enfin l'amendement huit complète inutilement utilement, il nous semble le contenu du document d'orientation qui sera transmis aux partenaires sociaux afin qu'il présente les options possibles pour garantir l'équilibre financier du régime sans revenir à la contrainte du budget de cadrage, il nous semble donc que cette proposition est de nature à éclairer la négociation des partenaires sociaux en en vue de la conclusion d'un accord, c'est donc à l'avis favorable sur le huit. Donc, maintenant, il nous faut l'avis du gouvernement sur cette série. Merci monsieur le président le l'avis du gouvernement sur cette série d'amendements et est le même que celui de la commission, à une exception près. Nous avons un avis défavorable sur la totalité des des amendements pour des raisons parfois convergentes avec celles exprimées par Madame la rapporteure parfois différente puisque nous considérons que certains des amendements vont plus loin que ce que la commission a adopté, dans la mesure où le gouvernement ne partage pas l'option de la commission sur l'organisation de la discussion, nous ne pouvons donner un avis favorable et cela explique que la vie soit aussi défavorable sur l'amendement numéro 8 telle qu'il a été présenté et auquel Madame la rapporteure, a donné un avis favorable à l'instant

du choix que nous avons fait pour accompagner la mise en place de la contrat cyclicité entre concertation et et négociations pour dire que l'avis du Conseil d'État a rendu le 5 septembre précise que dans la mesure où nous proposons la suspension de la compétence des partenaires sociaux tels que prévu à l'article L-1 du code du travail pour 14 mois le gouvernement peut, par décret, définir les règles d'indemnisation de l'assurance chômage, dans le même avis : le gouvernement dit que, en application de l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 le Conseil d'État dont enjoint le gouvernement conseil au gouvernement plus exactement d'organiser une concertation autour de la question de la modulation et de la préparation du décret, il précise, de manière très explicite, que le gouvernement est ainsi exonérés d'une obligation de négociation mais doit consacrer la consultation nécessaire des partenaires sociaux otite du préambule de 1946 c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de cette concertation concertation qui doit permettre, nous le souhaitons tout cas d'aboutir avant la fin de l'année 2022 pour que l'application des règles de contrat cyclicité que nous appelons de nos voeux puisse intervenir dès début 2023 sur la la question relative à l'évaluation de la réforme de l'assurance chômage, telle que définie en en 2019, cette réforme a été défini par le décret de 2019 est entré en vigueur le 2 novembre 2019, mais la réalité de son application a été décalé au au second semestre 2021, du fait des périodes de confinement et des périodes de Covid ça explique cette période courte que nous n'ayons pas procéder à une évaluation en tant que telle manière tout à fait consistant, ça explique aussi pourquoi nous proposons la prorogation pour 14 mois, considérant que les premiers éléments dont nous disposons sur la diminution de la part des contrats courts sur le rétablissement des comptes de l'Unédic nous engage à poursuivre et à aller au bout de du délai qui était ainsi prévu je précise par avance que la la direction de l'analyse et de la recherche, des études statistiques du ministère du Travail a d'ores et déjà mis en place des procédures d'évaluation qui auront lieu au cours de l'année 2023 lorsque la réforme suffisamment d'ancienneté pour pouvoir être ainsi évaluer deux 3 remarques pardon, enfin la première pour dire, mais je fais quoi, une intervention de Madame la Ministre, Lyman qui faisait référence à l'héritage de la Libération, c'est vrai pour le préambule de 46 et la consultation des salariés, sur les conditions de travail, ça allait un peu moins mais ce n'est pas ce que vous avez dit, je tenais simplement à le préciser, sur la question de l'assurance chômage en tant que telle, puisque le régime que nous connaissons, a été défini en 1958 de manière un peu décalée, je le dis par précision et une et pas par contradictions Madame Madame la Ministre, la 2ème chose pour dire que je ne sais plus si c'est Madame Lubin en monsieur Chantrel qui l'a évoqué, vous m'avez dit à un moment que c'était la première fois que les règles d'assurance chômage était défini par décret et non pas en application d'un accord national interprofessionnel, ça n'est pas le cas il y a un précédent en novembre 2000, ou un décret a été pris pour pallier ou en tout cas, prendre des dispositions différentes de celles de l'accord majoritaire, qui était intervenu et, enfin, il a été posé la question par dame madame mange des saisonniers, ce que je peux vous dire madame la sénatrice, c'est que, à l'été 2022 par rapport à l'été 2019, donc avant la crise du Covid, le secteur de l'hôtellerie, des cafés, des restaurants qui est le plus fort pourvoyeur d'emplois saisonniers affiche 5 % d'emplois de plus qu'en 2019, donc il n'y a pas de grande démission des saisonniers et nous sommes loin de de la fuite ou de la désertion des saisonniers, que l'on entend ou que l'on voit évoquée

et donc nous commençons par le, 85 qui a fait l'objet la double avis défavorable. Et ce qu'il y a des explications de vote si il y en a pas, je consulte, qui est pour cet amendement.

monument 77 même vote Monsieur Chassaing pardon.

engager une conversion une concertation avec les partenaires sociaux sur la gouvernance et à conclure un accord de l'assurance chômage sur indemnisation bien sûr et sur un document d'orientation je voterai cet amendement parce que je ne vois pas pourquoi il est contre la la l'article 1 de la commission.

moment 19 double avis défavorable qui est pour. Contre n'est pas retenu l'amendement vingt même votre

Non, alors donc on va voter séparément, qui est pour l'amendement de Monsieur kaput. Qui est contre.

Donc il a fait l'objet d'un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement, donc il est favorable. Alors qu'il est contre. Il est adopté. Nous restons sur l'article 1er et nous examinons l'amendement 51 présenté par Madame ah, pour s'opposer. Merci, merci Monsieur le Président, le présent amendement vise à revenir sur la réforme de 2019 de l'assurance chômage qui a modifié les règles d'indemnisation et entraîner une baisse de 17 % en moyenne de l'allocation chômage pour 1,15 1000000 d'allocataires et jusqu'à 40 % pour près de 400000 d'entre elles et eux la réforme de 2019 a modifié la formule Duc de calcul du salaire journalier de référence et notamment la prise en compte des périodes non travaillées, les allocations chômage versées aux demandeurs d'emploi ne sont donc plus lié aux salaires, il convient donc de revenir sur la loi de 2019 qui a contribué à la précarité de milliers de chômeurs alors que, selon le ministère du Travail, entre 25 % et 42 % des privés d'emploi ne demande pas la location à laquelle ils ont droit, le durcissement des règles d'indemnisation renforce le non le non recours la lisibilité du système d'assurance chômage pour les allocataires est remise en cause par ces réformes successives qui complexifie les règles de l'assurance chômage, jusqu'à présent un jour travaillé ouvraient droit un un jour d'indemnisation, l'ensemble de ces principes sont remis en question avec les projets du gouvernement auquel nous nous opposons fermement, par conséquent, nous demandons l'abrogation de la réforme de 2019 je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, leur effectivement un autre collègue souhaite au travers cet amendement, remettre en cause la réforme de l'assurance chômage, alors c'est vrai que nous, nous avons fait le choix plutôt hein de proroger le décret de carence, mais au-delà de ça, chers collègues, je pense qu'il y a une un problème d'imputation d'articles sur cet amendement et en fait entre l'objet recherché et l'amendement telle qu'il est posé, il doit y avoir une erreur donc au-delà de cet aspect-là, la commission a émis un avis défavorable. Le gouvernement. Pour le matin, madame. Donc je mets aux voix cet amendement numéro 51 avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est pour. Qui est contre. Il est pas adopté, nous avons ensuite 2 amendements identiques numéro 52 et numéro 88

en cas d'écarts significatifs entre la trajectoire financière du régime d'assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l'accord, en fait, on est, on est là typiquement dans la situation de déresponsabilisation des partenaires sociaux avec le gendarme qui serait la puissance publique éternel. Ce qui d'ailleurs entre nous soit dit, ah plutôt la de ne pas inciter à la responsabilité, parce que quand vous savez qu'in fine et et ben les les sujets difficiles qui suppose un compromis équilibré, vous pouvez vous dispenser d'avoir assumé ce compromis est laissé à l'état l'arbitrage final ça finit par tuer le fondement même de la démocratie sociale qui est effectivement d'arriver à un équilibre dépositions des compromis équilibrés et globaux non seulement c'est un recul du paritarisme ont seulement, c'est une vision de l'État surveillant général des finances, mais en plus je ne crois pas que ça concourt à la responsabilisation collective.

sur l'écart sur la loi avenir professionnel de 2018 et de cet écart, et du fait que le 1er ministre du coup demande aux organisations d'employeurs et de salariés de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l'accord et ainsi négocier des mesures d'économies, mais enfin, encore faudrait-il savoir d'où vient le déficit, le déficit de l'Unédic a été largement causée dans le passé par le désengagement progressif de l'État et sa participation de plus en plus importante au film et la qui correspond quand même désormais à 11 % de ces retraites qui désormais dépasse celle de l'État et qui a provoqué hier un déficit artificiel, de ce fait, amplifiée par la suppression des cotisations chômage des salariés via l'instauration de la C. donc sensible, fluctuant au gré des dynamiques de l'emploi, la santé financière de l'Unédic ne peut constituer le critère pertinent à court terme pour la négociation des accords sans faire cette cette analyse des causes des de l'écart qui a été pointé et dont l'objet doit rester la protection des droits des demandeurs d'emploi dans le cadre d'une sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie, donc par conséquent, nous proposons de supprimer ces dispositions de rationnement budgétaire prétexte à imposer de nouveaux décrets contre l'avis des partenaires sociaux, je vous remercie. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements. Merci monsieur le Président, effectivement, on a 2 amendements qui sont identiques à qui vise à supprimer le mécanisme de suivi financier de de l'assurance chômage, alors il leur il faut alors je partage un certain nombre de propos qui ont été énoncés par Madame mangent c'est vrai qu'il y aurait effectivement du ménage à faire, hein, sur le budget de l'Unédic, hein, qu'est-ce qui relève du paritarisme et qu'est-ce qui relève effectivement des décisions du gouvernement, mais au-delà de ça, des gouvernements, devrais-je dire, mais au-delà de ça, c'est pas parce qu'on a une gestion paritaire que au final ne l'État ne garde pas l'ultime droit de regard sur la gestion de l'assurance chômage et en l'occurrence ce mécanisme financier permet quand même d'avoir à un moment donné, ce qu'on appelle, nous, la règle d'or, c'est-à-dire à un moment donné, se dire : si on s'échappe d'une trajectoire financière à un moment donné l'état doit intervenir, c'est pourquoi nous sommes défavorables à ces deux amendements parce que nous avons, nous, souhaité conserver cet aspect de mécanismes financiers dans le texte de loi. Monsieur le Ministre, même avis donc je soumets au Sénat, les 2 amendements 52 et 88 qui est pour. Qui est contre. Ils ne sont pas adoptés et donc nous en venons au vote sur l'article 1er. Modifié par un seul amendement est ce qu'il y a des explications de vote sur ce sur cet article. S'il y en a pas jeune soumis à l'approbation du Sénat qui est pour l'article 1er. Qui est contre. Il est donc adopté après l'article 1er nous sommes saisis d'un amendement numéro 13 de Madame Lubin, il le présente. Actuellement, Pôle emploi né destinataire que de 15 % des offres d'emploi diffusées par les employeurs, notre amendement vise à rétablir l'obligation de diffusion des offres d'emploi via le service public de Pôle emploi, cette obligation est un préalable à la mission de placement des demandeurs d'emploi par Pôle emploi, surtout depuis l'application de la procédure de refus d'offres d'offres dites raisonnables dont la définition a été largement restreint dans 2019 qui peuvent aboutir à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi : Pôle emploi peut donc radier des chômeurs pour avoir refusé une offre mais n'est pas destinataire de l'ensemble des offres d'emploi, ce qui est un non-sens. Et ce qui était le cas auparavant, hein, il faut dire qu'auparavant, Pôle Emploi été destinataire de toutes les Offres d'emploi. mais entre temps, les plateformes se sont développés, Le Bon Coin est arrivé à un certain nombre d'outils ont été mis à disposition d'un certain nombre de chefs d'entreprises et d'ailleurs du reste aussi d'un certain nombre de personnes qui qui recherchaient un emploi et, effectivement, si cet amendement vise à obliger les employeurs à transmettre leur leur offre d'emploi, pôle emploi ce n'est plus le cas aujourd'hui, dire que Pôle emploi ne nous a pas attendu pour finalement aller récupérer les Oeuvres qui sont sur ces plateformes, si je prends l'exemple de l'Isère lisière agrège 100 plateforme et va chercher sans opérateur qui déjà mettre en ligne un certain nombre d'offres d'emploi, donc en agrégeant ses 100 plateformes et y compris les Oeuvres qu'ils reçoivent, je crois qu'on a un panel des des offres d'emploi qui sont mises à disposition, je crois que c'est plutôt quelque chose qui est vertueux cet amendement étant un peu péremptoire et à mon avis n'est n'étant pas utile, compte tenu du fait que, de façon opérationnelle choses se font déjà, la commission a émis un avis défavorable. Eh bien, c'est l'avis du gouvernement également. Je le mets donc aux voix, quels sont ceux qui sont favorables à cet amendement numéro 13 pardon. Qui est contre.

Oui alors, cet amendement vise à inscrire dans la loi les objectifs mêmes de l'assurance chômage qui a date en sont totalement absents, il s'agit ici de, de, de contrer une dérive insidieuse orchestrée par le gouvernement, tels que de décret en projet de loi qui modifie profondément la philosophie même de l'assurance chômage, alors il convient donc d'inscrire dans la loi le caractère assurantielle de l'assurance chômage et sa vocation à sécuriser le revenu d'des travailleurs.

Entendu, avis de la commission sur ces deux amendements. Oui, merci Monsieur le Président, effectivement, ce sont des amendements identiques, hein, qui est non, c'est un principe de solidarité face au risque de privation d'emploi c'est un dispositif et un énoncé qui me semble très général, qui n'apportent il ne retire rien et aucune garantie aux demandeurs d'emploi, c'est donc un avis défavorable sur ces deux amendements, monsieur le président. Même avis du gouvernement, je les mets aux voix, y a-t-il des voix pour.

mes chers collègues, la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 proclame le le droit au travail, qu'a évoqué le ministre-tout à l'heure en discussion générale et l'objectif du gouvernement et si la courbe du chômage évolue plutôt positivement, il y a encore beaucoup trop de gens qui sont malheureusement loin de l'emploi, afin de les soutenir, les guider dans leur recherche, a été mis en place, instaurer voici quelques années le le parcours personnalisé d'accès à l'emploi avec, notamment, ça a été évoqué par Madame Lubin tout à l'heure, l'offre raisonnable d'emploi qui est basée sur 3 critères donc la zone privilégiée géographique où doit se situer l'emploi le salaire attendu et, évidemment, la nature et les caractéristiques de l'emploi aujourd'hui, la législation fait que la radiation d'un demandeur d'emploi peut être prononcée pour 2 offres raisonnables d'emploi refusé, se pose le cas d'une offre raisonnable d'emploi qui est refusé, sans motif valable l'objectif de cet amendement, c'est d'inciter le demandeur d'emploi à revenir à l'emploi en réduisant de moitié au cas où les refuser une offre raisonnable d'emploi l'indemnité perçue ça agit pas du tout de stigmatiser, il s'agit pas du tout de punir le demandeur, il s'agit de l'inciter, de valoriser le travail avec d'abord une logique de cohérence puisque l'offre d'emploi raisonnable, c'est lui-même qui l'a défini, donc c'est un petit peu étonnant de refuser ce qu'on veut, et puis la 2ème chose, ça a été évoqué tout à l'heure par Philippe mouiller c'est la problématique de besoin sur le marché du travail, nous rencontrons tous quasi quotidiennement des chefs d'entreprises qui sont en recherche de personnel, il faut répondre aussi à cette attente. Merci madame la rapporteure sur l'amendement de. avoir un moment donné, une réduction de, de, de l'allocation de retour à l'emploi, bon, j'avoue que ce problème de l'offre raisonnable d'emploi et est en l'occurrence un problème, ça semble être du bon sens, d'ailleurs, la loi de 2007, je vois Catherine Procaccia, qui là, elle avait descendu en son temps, en 2007 ou en 2008, on est effectivement sur un principe de bon sens, mais force est de constater aujourd'hui que ça ne marche pas, on est, effectivement, on a d'abord été sur 3 refus d'offres raisonnables d'emploi on est aujourd'hui sur 2 refus d'offres raisonnables d'emploi, on pourrait passer à un refus d'offres raisonnables d'emploi mais moi quand je regarde les statistiques, qu'est ce que je vois, alors on avait les statistiques, les seules que nous avions effectivement à l'époque quand on était sur la loi de 2018 nous avions les statistiques de 2016 les offres raisonnables d'emploi ne représentait que 0 0 2 % du total des radiations notre collègue, Laurent Somon, qui n'est pas là mais, mais il était aussi de déposer le même type d'amendements, il est allé voir Pôle emploi de la Somme et il a effectivement regarder en quoi effectivement les offres abominable d'emploi était un facteur qui permettait à un moment donné de dire on va pousser des gens à reprendre une activité quand on a effectivement un refus d'offres raisonnables d'emploi hé bien effectivement là sur la somme, ah si on regarde effectivement le chiffre les offres raisonnables d'emploi ne représente, en l'occurrence j'ai vous retrouver ce chiffre-là que cette motif de refus, alors que quand on est effectivement sur une absence de rendez vous, on est à 2383 refus, donc on s'aperçoit quand même qu'on a une vraie difficulté, donc moi ce que je voulais vous proposez, cher collègue, c'était de dire renvoyons-nous à l'article 6 l'article 6 qui a été introduit par nos collègues députés qui précise effectivement que nous souhaitons un rapport alors c'est suffisamment rare pour le préciser, madame la présidente, nous avons laissé cet article aussi dans ce, dans le texte de loi alors que systématiquement on refuse des rapports et la demande qui est faite par nos collègues de l'Assemblée nationale et que nous avons proposé de garder, qui est l'article 6 qui précise qu'effectivement, nous avons besoin d'un rapport sur les offres raisonnables d'emploi pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas à hauteur de ce que ça devrait fonctionner parce que vous avez raison de le dire, c'est du bon sens, mais dans les faits, ça ne s'apparente pas effectivement comme un motif pour une reprise d'activité, donc c'est plutôt un avis défavorable ou alors une demande de retrait en attendant qu'on ait suffisamment d'et d'éléments de ce que va nous apporter l'article 6 qui est dans ce texte de loi. Ce ministre. monsieur le président, comme Madame, la rapporteure de manière assez, assez exceptionnel en tout cas pour ce qui me concerne, le gouvernement a donné un avis défavorable à l'amendement qui proposait d'inscrire un article 6 et donc une demande de rapport sur l'offre raisonnable d'emploi madame la rapporteure là dit la radiations pour refus de 9 raisonnable d'emploi d'une 2ème offre raisonnable d'emploi est un phénomène qui, en réalité extrêmement marginal, d'un point de vue statistique, on parle de quelques centaines, parfois même de quelques dizaines d'unités par an parce que la définition de l'offre raisonnable d'emploi est difficile à établir, que ce soit sur le critère géographique ou sur les équivalences de qualification, c'est la raison pour laquelle je m'associe à la demande de retrait de l'amendement et que je renvoie moi aussi à cet article si ce qui permettra par le rapport demandé et auquel l'ensemble des administrations évidemment concourir de mieux préciser les définitions, la manière dont on appréhende ce qui est 9 raisonnable d'emploi pour que ce qui peut être effectivement un principe de de un principe de bon sens en tout cas une clé d'explication puis c'est applicable en l'état, ça ne nous paraît pas l'être, d'où la demande de retrait à des fois, ça sera un avis défavorable. monsieur, madame Dumas d'abord demandé la parole et ensuite monsieur Richard. je pense que nous avons eu à peu près tous des témoignages, moi j'en ai eu mais je suis convaincu que je ne suis pas la seule, de personnes qui vous disent mais on m'a proposé, Pôle emploi m'a proposé un emploi mais dans des conditions dans lesquelles je ne peux absolument pas le pourvoir aller travailler à mi-temps quand on est dans un département rural, par exemple, les faire 100 kilomètres aller-retour par jour pour un emploi à mi-temps est-ce que c'est une offre raisonnable d'emploi oui, mais c'est une question de bon sens, mais il y a des gens qui considèrent que, hé bien, lorsqu'on n'a pas d'emploi on doit accepter une offre d'emploi, point barre, et pour qui l'offre raisonnable d'emploi ben si celle-là, donc on est dans le subjectif et une fois n'est pas coutume je partage assez ce que vient ce que vient le l'idée d'un rapport après tout on en demande de nous des rapports qu'on obtient jamais d'ailleurs, soit dit en passant, dont quelques-uns aurait je pense pourtant leur utilité, mais bon, j'attends de voir ce qu'il y aura dans un futur rapport je pense que la subjectivité de l'offre raisonnable d'emploi rapport ou par rapport demeurera.

et elle est pour moi frappé au coin du bon sens, madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, j'ai bien compris que vous nous disiez que ça ne marche pas, la notion, le concept de d'offre raisonnable d'emploi ne marche pas.

c'est assez clairement expliqué qu'est ce que c'est qu'une offre raisonnable d'emploi c'est une offre dont la nature et les caractéristiques de l'emploi, rechercher la zone géographique privilégiée le salaire attendu ont été déterminées au sein du projet personnalité d'accès à l'emploi du chômeur un accord sur toute une série de de critères, c'est la nature, excusez-moi de le répéter les caractéristiques de l'emploi, la zone géographie il va vous dire quelle zone il va vous dire le salaire attendu et on dit que ça marche pas et et et et donc on va faire un rapport pour savoir ce que c'est qu'une offre, mais c'est clair, ça c'est clair, moi je franchement je pense que il il est temps de prendre des mesures à l'égard de, de, de personnes qui, qui indique une chose un jour et qui, après, il se contente de dire non, non, ça m'intéresse pas, ces critères ne correspondent à rien et je ne suis pas prêt à accepter cette offre, franchement, je crois que on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, voilà et ce qu'il faut un rapport pour ça non, moi je veux le faire fonctionner, il y a un projet personnalisé, le chômeur indique ce qu'il veut, lorsqu'il a dit que ce qu'il voulait, si c'est si c'est effectivement à ça, dit à sa disposition qu'il l'accepte, merci. Je voudrais juste apporter une précision, ça existe déjà le conseiller Pôle Emploi a la possibilité de suspendre les allocations 15 jours pour défaut de recherche d'emploi. Madame Lienemann. Ne nous approuvons l'idée de rapport parce que comme vous l'avez dit madame la rapporterait, en fait, on a l'art de se focaliser sur des sujets qui ne sont pas les sujets prioritaires et du coup, hé ben on ne s'occupe pas de regarder tous les autres sujets, alors l'obsession, c'est d'aller chasser la masse des chômeurs tricheur qui ne voudraient pas travailler qui se débinent devant des les opportunités de travail et caetera moi j'avais une formule un peu provocatrice quand on aura plus que le les fainéants au chômage en France, on peut, on saura résoudre les problèmes, je rappelle qu'il a quand même 5 millions de chômeurs non indemnisés. nous ne souhaitons ce rapport et nous souhaitons qu'au contraire, au lieu de se focaliser sur des sujets qui vise sans arrêt à culpabiliser une infime minorité de chômeurs en discréditant les autres nous nous occupions des sujets massif, par exemple, le gouvernement pendant des années, en tout cas depuis Monsieur Macron a voulu tuer globalement les négociations de branche au profit des négociations d'entreprise si nous revalorisation le travail des branches le pouvoir qu'elles ont sur la formation, sur la définition des nouveaux métiers sur l'amélioration des codes du travail, quitte à être accompagnés par l'État dans certains dans certaines branches, nous aurions certainement un rapport au travail, améliorer des opportunités et de de retrouver un lien entre la formation, la volonté des jeunes et des salariés et les opportunités des différentes branches.

madame le rapporteur, et je voterai votre demande de rapport, peut-être qu'il faut effectivement clarifier les choses et peut être et même sûrement que sur le territoire, les conseillers Pôle Emploi n'agissent pas forcément partout de la même façon, néanmoins, je suis convaincu que autour de vous, vous avez rencontré des demandeurs d'emploi qui ont bien co-construit entre guillemets leur offre raisonnable d'emploi et ce qu'il souhaitait figurer bien précisément dans les offres qu'on leur a proposé, moi j'ai beaucoup d'exemples à partir de là, ça me semble vraiment illogique de ne pas les mettre en face de leurs responsabilités, il y a des droits, il y a des devoirs après Madame Lienemann mes propos ma proposition a été légèrement caricaturer par vous-même, vous vous parlez de chasse aux méchants of chômeur fainéant, excusez-moi, ce n'est pas du tout l'objet et avec une malice gentille, permettez-moi de vous dire que je suis plutôt du côté de votre leader Fabien Roussel qui préfèrent la France du travail à la France du chômage et qui n'aime pas trop la gauche des allocs et qui n'aime pas trop le droit à la paresse, dont certains d'entre vous se prévalent. Bien, je pense qu'on doit pouvoir voter mais hein pour se Poli ne nous privons pas. Nous aussi, monsieur, nous approuvons les propos de Fabien Roussel je vous rassure, et Fabien Roussel ne remet absolument pas en cause le droit à des personnes à être indemnisés aux allocations chômage, oui, nous défendons le travail mais nous défendons aussi ces gens qui sont victimes du chômage, qui ont cotisé quand même pour la plupart, et qui ouvre droit à des allocations chômage, voilà, je voudrais vous juste vous faire cette précision parce que comme vous parlez de mon secrétaire national, hé bien, je me sens en droit de vous répondre, merci.

Qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous passons à un amendement quatorze de Madame Lubin toujours après l'article 1er. Par un arrêt du 30 mai 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la caractérisation de la négligence fautive de l'organisme chargé de servir les allocations d'assurance chômage emportait un droit pour le demandeur d'emploi, obligés de restituer des sommes indument versées de solliciter réparation de son préjudice et que le juge du fond avait souverainement apprécié le montant du préjudice causé par cette faute en lui allouant une somme correspondant au montant des allocations litigieuse nous proposons simplement de fixer cette jurisprudence dans la loi la défenseure des droits est en effet encore saisi de dossiers pour lesquels Pôle emploi n'assure toujours pas la réparation du préjudice subi en raison de ces manquements pour éviter des démarches lourdes, voire des procédures parfois coûteuses pour le bénéficiaire. Quel est l'avis de la commission du 30 mai 2000, alors nous nous considérons, on en a déjà discuté en commission, hein, nous considérons qu'il n'est pas utile d'inscrire cette jurisprudence dans le code du travail, car le principe de la responsabilité civile qui est reconnu par la loi et d'application générale et que l'Arctique 1240 du code civil, posant en effet le principe de la responsabilité du fait personnel, donc ça en mettre effectivement un amendement qui est satisfait, donc, c'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable de la commission. Monsieur le Ministre, mais ma vie vous le maintenez Madame. Je le mets aux voix qui est pour. qui est pour. Il n'est pas adopté, nous poursuivons les articles additionnels après l'article premier, donc c'est l'amendement 31 également de Madame Lu Cet amendement vise à donner des garanties procédurales, lorsqu'un demandeur d'emploi une décision administrative le concernant suite à différentes réformes, le demandeur d'emploi se retrouve facilement dépourvu quand une décision administrative est prise à son encontre radiation sanctions changement de catégorie rattrapage d'indus, il ne sait pas à qui s'adresser, dans quel délai et ce d'autant plus avec la numérisation de l'accès au service public, s'il arrive tout de même à formuler un recours, ce dernier n'est pas suspensif, ce qui peut entraîner parfois de graves conséquences économiques pour son ménage à l'opposé de cette maltraitance administrative institutionnalisé, nous proposons de garantir des droits procéduraux basique aux demandeurs d'emploi, la possibilité d'aller devant le juge et le médiateur en même temps le caractère suspensif du recours et la nullité des décisions ne respectant pas ces garanties. Ces garanties seraient de nature à favoriser un meilleur traitement administratif des demandeurs d'emploi à réduire ainsi leur anxiété administratives et à améliorer leur insertion professionnelle et sociale, j'avoue que, d'ailleurs, ce genre d'amendements, ça vaut pour des demandeurs d'emploi, mais ça, ça peut aussi valoir dans d'autres situations. Entendu Madame la rapporteure. parce qu'ils ont des difficultés sur le montant qui qui qui est proposé, néanmoins nous considérons quand même qu'il y a déjà un certain nombre de procédures de contestation qui existe, il y a déjà des possibilités de faire des réclamations à Pôle emploi il y a des médiations qui sont possible, il y a des instances paritaires régionales qui veillent en outre à l'application des règles de l'assurance chômage et pour lequel, qui peuvent être saisis qui peuvent être saisis par les demandeurs d'emploi et puis avoir des recours de justice qui sont également possibles, donc il ne me semble pas nécessaire d'introduire de nouvelles mesures, même si on est bien d'accord, on aura peut-être toujours un certain nombre de personnes qui seront dans la difficulté, on en connaît tous mais en tout cas alourdir ce processus, nous ne nous semble pas souhaitable, c'est donc un avis défavorable de la commission. Avis partagé par le gouvernement, je mets aux voix l'amendement numéro 31 avec double avis défavorable et pour. Contre. La population. Nous avons ensuite l'amendement numéro 15, également du groupe socialiste. C'est un amendement qui vise à instaurer un versement automatique par Pôle emploi des moins perçus aux allocataires, selon un dispositif miroir de celui appliqué pour les trop perçus. Madame le rapporteur. amendement qui précise qu'il faut que les allocations soient versées, ce qui est un peu une lapalissade : il faut que les allocations soient versées, il faut que nous le réaffirmons nous pour pas qu'on connaît ces difficultés que j'ai annoncé tout à l'heure, mais de la même façon il viserait effectivement à ce que Pôle emploi puisse anticiper ses propres erreurs ou celle des demandeurs d'emploi, donc c'était un amendement qui ne paraît pas très opérationnel, c'est donc un avis défavorable de la commission. une indemnité n'est pas totalement versées du fait d'une pièce manquante, la fourniture de la pièce compte entraîne automatiquement le versement, donc c'est la pratique de Pôle emploi, c'est en cela que votre amendement est satisfait et s'il fallait le rappeler au banc pour qu'il y a un caractère officiel à la déclaration s'est ainsi fait donc c'est une demande de retrait ou défavorable. Vous avez ensuite prononcer sur l'article l'amendement numéro 26 de Madame Rubin, qui va le présenter. Cet amendement vise à créer un conseil d'orientation de l'assurance chômage, nous constatons en effet que le débat public sur la réforme de l'assurance chômage, objet du présent projet de loi est excessivement par le manque de données publiques sur l'assurance chômage public perspectives financières impact des précédentes réformes, cela conduit à considérer des propositions infirmée par la recherche économique, exemple la dégressivité de l'allocation, la hausse de la durée d'indemnisation, la baisse des montants de l'allocation comme efficace pour inciter le demandeur d'emploi à trouver un emploi, le fleurissement des amendements anti-indemnisation alors que seuls 40 % des demandeurs d'emploi sont indemnisées en sont une illustration supplémentaire, nous proposons donc la création de ce conseil d'orientation à l'assurance chômage qui pourrait prendre modèle sur le conseil d'orientation des retraites et qui serait une instance indépendante du pouvoir exécutif qui fournirait un rapport annuel, appuyé sur des données publiques, de manière à éclairer le débat public. l'avis de la commission madame la rapporteure. Merci monsieur le président, donc, effectivement, cet amendement vise à la création d'un Conseil non permanent d'orientation de l'assurance chômage, alors c'était un principe qu'une qu'ne nous semble pas souhaitable pour un certain nombre de raisons, d'abord parce que

et enfin les concertations et les négociations en matière d'assurance je me chômage ont vocation à se tenir dans le cadre du paritarisme et le Parlement peut être informé grâce à ses prérogatives d'évaluation et de contrôle, donc, c'est donc un avis défavorable sur cette proposition. monsieur le président je considère l'idée intéressante hein intéressante parce que lorsqu'on parle de de mesures y compris dans le cas de la compta cyclicité vous contestez mais le ce qu'on parle de mesure des indicateurs économiques et la mise en oeuvre de mesures de modulation, avoir un conseiller d'orientation, un conseil scientifique peut être utile et lorsqu'on parle de perspectives financières pour l'Unédic, avoir aussi un avis d'expert peut être utile, par contre, l'avis est défavorable à ce stade, pour une raison pour moi, cela relève véritablement d'une négociation entre les partenaires sociaux, dans le cas de la négociation sur la gouvernance de l'assurance chômage, que j'ai annoncé pour le 1er semestre 2023, donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Madame Hubert. Entendu, donc nous le soumettons aux voix, sauf s'il y a des demandes d'explications non donc l'amendement 26 avec double avis défavorable qui est pour. Contre n'est pas adopté. Dernière amendement dans cette série d'articles additionnels Madame Carrère vous Monsieur Merci monsieur le président, donc la la loi du 5 septembre 2018 prévoit un rapport sur les conséquences du non-recours aux droits d'assurance chômage, visait à apporter un éclairage quantitatif au phénomène de non recours à caractériser la population nous recourant et à proposer des pistes d'explication explication il ressort de cette étude que l'estimation du taux de non recours des personnes non inscrites à Pôle Emploi dans l'année qui suit leur fin de contrat varient entre 25 et 42 % selon le chant les hypothèses retenues, cela représente environ entre 390000 690000 personnes essentiellement des salariés en contrats courts, ces chiffres sont édifiants, aussi, il nous semble important qu'au vu de cette étude, le gouvernement puisse proposer des pistes d'amélioration qui permettrait d'assurer un meilleur recours au droit en matière d'assurance chômage. Oui, merci Monsieur le Président, alors c'est vrai que je, je, je reconnais que l'étude de la Dares, est ce qui nous a été proposé un peu une extrémiste par le par la d'arrêt je vais pas dire que c'est pas le gouvernement et par la Darès lors de la séance à la nationale et est plutôt intéressante et et forcé de constater quand même Monsieur le Président, comment quand même d'un certain nombre de données sur l'assurance chômage et qu'on a besoin effectivement de pouvoir à un moment donné, et faire un état des lieux d'un certain nombre de mesures qui sont prises et également avoir des chiffes qui nous permettre d'éclairer les débats chers collègues, nous avons fait déjà des efforts considérables, nous avons maintenu de rapport dans ce texte de loi, l'article 6 et l'article 7 c'est pour ça je je vous propose, puisque là, c'est encore une demande de rapport là par contre, de vous donner un avis défavorable sur cette proposition de demandes de rapport, même s'il faut quand même bien le dire, tous les suivis relatif au non-recours sont quand même intéressant, et communiqué loue des chiffres, nous en avons besoin pour effectivement avoir des informations sur la gestion du ludique et au-delà sur la façon dont le marché de l'emploi se passe dans notre pays. Merci monsieur le président, effectivement le le rapport sur le non recours a été rendu avec du retard, il a été transmis au Parlement le le 29 septembre c'est une vraie base de travail, il a un aspect rassurant si je puis dire, mais je mais ce n'est pas parce que c'est rassurant que c'est satisfaisant parmi les causes non recours il y a parfois une volonté quand je dis une volonté, c'est le cas d'un demandeur d'emploi qui termine un contrat mais qui ne s'inscrit pas auprès de Pôle emploi parce qu'il sait qu'une note période d'activité va sourire dans un délai relativement court, et il a un autre aspect rassurant mais qui n'est pas satisfaisant, c'est le fait que le taux de non-recours semble à peu près identiques à ce que l'on connaît sur d'autres prestations sociales, ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant, mais ce n'est pas pire au plus mauvais qu'ailleurs, il faut qu'on puisse continuer à travailler sur l'information sur l'accès au droit, dans l'attente, c'est une demande de retrait plutôt qu'avoir un second rapport sur les mêmes raisons. retraites entendu. Donc, nous arrivons à l'article 1er bis à pour lequel nous avons au départ quatre amendements de suppression identiques et nous commençons par le 33 présenté par Madame Merci monsieur le président, notre groupe est est fermement opposé à la philosophie de culpabilisation des chômeurs, porté par par ce projet de loi nous ne souscrivons donc pas à l'agrégation de de cette logique introduite par les rapporteurs en commission avec la suppression de l'indemnisation chômage au bout de trois Offres d'emploi en CDI refusé à l'issue d'un CDD, de même pour le principe de contrat cyclicité inscrit à l'initiative des rapporteurs dans le code du travail et qui vise à faire varier à la baisse ou à la hausse les indemnités des chômeurs en fonction de la situation économique du pays, c'est pourquoi notre amendement vise bien évidemment à supprimer cet article. Madame Lienemann, pardon, donc ça allait bien, l'amendement 70. Oui, et cet amendement si peu demande la suppression de cet article et en particulier parce qu'il prévoit qu'en cas de refus de trois reprises un CDI, le salarié de CDD n'aura plus d'indemnisation du chômage, nous considérons que cette mesure est totalement absurde et en tout cas, injuste, parce que vous êtes prompt à nous expliquer que les chefs d'entreprises ont besoin des CDD, nous vous nous avait vanté la précarité tellement à l'excès d'ailleurs que l'on on en voit maintenant les effets négatifs, en revanche, le salarié, lui, il sera obligé d'accepter dit personnellement, si je devais avoir le choix, je choisirais le CDI mais au nom de quoi alors que nous avons des gens qui cotisent nous imposerions salariés de prendre un CDI, tant les CDD existent 2ème chose monsieur, monsieur le préfet, nommé ministre, je voulais vous indiquez que vous m'avez bien donné le chiffre de 40 % pour les créations de CDD mais vous comparez l'année 2022 à l'année 2021, or il serait plus juste de prendre comme base, février 2020, c'est-à-dire avant la pandémie premiers mois avant la pandémie et à ce moment-là, on a une augmentation des CDI qui n'est de 12 % toujours mieux que rien, mais c'est en tout cas ne tombons insuffisant, il ne fait pas la preuve d'une efficacité du bonus malus. L'amendement 79 et présentée par Monsieur Gold je suppose. nous considérons ce dispositif ne contient aucun garde-fou permettant de vérifier si le refus du salarié est justifiée ou non. Et toujours dans la série des amendements identiques Madame poncer monde avec l'amendement numéro 103.

retourner au travail et vraiment à contre-courant des analyses et des enseignements qu'il faudrait tirer quand même de phénomènes sociaux observé récemment et notamment c'est vrai après suite au confinement comme la vague de démissions qui révèlent quand même une une aspiration à des emplois de qualité et le refus d'un travail dépourvue de sens ou mal rémunérés aux conditions de travail dégradées s'étale c'est à heure. Si ne fait que prolonger la politique quand même de du soupçon permanent envers les demandeurs d'emploi allergique au travail addict aux prestations et qui refuseraient délibérément les offres, les Oeuvres pour se complaire au chômage et qui vivrait donc aux dépens des travailleurs qu'ils ont un temps été quand même puisque cela leur a permis d'ouvrir les droits qu'gaspillent aurait ce récit a une fonction quand même essentiellement idéologique qui malheureusement progresse à force d'être martelé ce qui n'en fait pas pour autant une vérité hein, même si on peut regretter de l'avoir quand même quelques fois complaisamment reprise selon le l'OFCE, faut-il vous le dire, vous le martelez 8 % seulement des allocataires de l'assurance chômage n'aurait chercherait pas vraiment d'emploi, or ces personnes-là, selon Pôle emploi sont le plus souvent déjà rattrapés par les contrôles par les radiations en cas de non recherche d'emploi ou de refus de ces offres d'embauches prétendument raisonnables de plus la temporalité de 12 mois semble ignorer que, selon l'Unédic cette locataires sur 10 sont indemnisés, moins d'un an cet article poursuit donc je suis désolé de le dire, un bug d'affichage politique et idéologique, n'ajoutant rien passé la la oui, oh la la, oui, c'est nous qui devrions dire oh là là, hein, depuis 2 heures n'ajoutant rien au dispositif il n'ajoute rien au dispositif déjà fourni des sanctions pour les demandeurs d'emploi, mais ajoute à l'entreprise visant toujours à faire de ces chômeurs, les responsables de leur situation et c'est amendement donc vise à la suppression de cet article. Quel est l'avis de la commission sur les quatre amendements madame là. Oui, merci en CDI au terme d'un CDD, et le deuxième inquiétant effectivement à inscrire dans le code du travail, l'aspect contracyclique, tels qu'il a été effectivement énoncé à plusieurs reprises dans cet hémicycle alors je je passe sur le côté contrats cycliques parce que je crois qu'on a déjà dit un certain nombre de de choses en la matière, je vais revenir sur cet aspect qui concerne effectivement le le principe qui tend à priver les salariés de la en cas de refus répétés d'offres d'offres d'emploi en CDI moins chers collègues, je vais vous répéter une phrase à plusieurs reprises dans cet hémicycle s'agissant effectivement de ce principe là, je voulais simplement vous ramener à l'essence même du droit de l'allocation chômage, quel est, ils ont droit à l'allocation d'assurance chômage, les travailleurs aptes au travail d'emploi est un volontaire et dont la privation d'emploi est involontaire, que dit le code du travail aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous l'avez effectivement et Nancy il dit effectivement qu'un salarié qui refuse au terme d'un CDD, un CDI sur un même emploi dans une même rémunération n'a pas droit à la prime de précarité qui est de 10 % je rappelle que 10 % du salaire brut, donc on a déjà un 1er pas qui nous permet, à un moment de dire qu'il n'y a peut-être pas de privation involontaire d'emploi. Parce que la vraie question : quand on est effectivement en CDD et qu'on refuse un CDI est-ce qu'on peut considérer que on est en privation d'emploi involontaire. Est ce qu'on peut considérer qu'on est en privation d'emploi volontaire non, on fait un choix de vie, mais cet amendement ne vise pas effectivement à dire un certain nombre de concitoyens fait les choix de vie que vous voulez, les personnes qui veulent, à un moment donné, à avoir des CDD et les enchaîner sans prendre de CDI bien entendu que jamais nous ne permettrons de dire : nous refusons ce principe là, simplement, nous disons qu'à partir du moment où on fait ce choix là, on n'a pas le droit à l'allocation de retour à l'emploi, on ne peut pas faire des choix de vie chère collègue, on ne peut pas faire des choix de vie qui sont payés par les système assurantiel, voilà l'objet de cet amendement, voilà pourquoi nous l'avons défendu, c'est donc un avis défavorable. Merci monsieur le président, madame la rapporteure là dit là, l'article 1er bis de a une particularité, c'est qu'il a 2 objets très distincts, premier objet d'apporter une base légale, en tout cas d'inscrire dans la loi le principe de la Contra cyclicité en fonction de la conjoncture économique, j'ai dit dans mon intervention avant la discussion générale, que le gouvernement est favorable et considère que c'est une piste intéressante, ça ne m'amène à ne pas souhaiter la suppression pure et simple de l'article 1er bis de par contre, je l'ai dit aussi : nous ne sommes pas favorables, mais j'y reviendrai dans un instant à la à l'occasion de la présentation de l'amendement 95 à la disposition adoptée par la commission des affaires sociales relatives à la privation de la en cas de refus de deux à 3 reprises d'un CDI à la fin d'un CDD, mais j'aurai l'occasion de m'en expliquer sur le 95 dans l'attente et et indépendamment de ce désaccord sur la 2ème partie de l'article je je ne souhaite pas sa suppression pour préserver la question de la contrat cyclicité introduite par la commission des affaires sociales, donc c'est défavorable. Madame avait a demandé expliquer son vote. Après, elle passe son tour Madame Lubin souhaite expliquer son vote. non, non, la réalité c'est quoi la réalité, vous la voyez depuis votre siège et là chers collègues et la réalité non je, non mais je, je l'ai déjà dit effectivement lors d'un lors d'un de notre

donc nous ne pouvons pas légiférer et inscrire dans le marbre des choses que nous avons en tête parce que nous l'avons entendu comme ça, de ci de là parce que, comme le disait je ne sais plus qui, ce matin, ou ou comme le disait tout à l'heure d'ailleurs Monsieur Vanlerenberghe dont j'ai apprécié l'intervention tout à l'heure en en discussion générale, je trouve que là, ça n'est pas sérieux, on va inscrire dans le même dans le marbre des choses qui peuvent pénaliser durablement, je vais vous citer un exemple, vous prenez un demandeur d'emploi qui a perdu un emploi sur l'entreprise a fermé c'est arrivé dans tous nos coins de France et c'est arrivé, particulièrement chez moi des gens qui ont cinquante ans qui avait 30 ans de carrière donc un salaire qui allait à peu près avec leur carrière et ainsi de suite, qui au bout de quelques mois n'ont pas retrouvé un emploi qui entraîneur dans une industrie à côté, je peux citer l'agroalimentaire par exemple parce que ils ils arrivent en fin de droits, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas trouvé d'emploi qui correspondait à ce qu'ils avaient auparavant et je trouve qu'à cet âge-là, c'est normal de vouloir avoir un emploi qui correspond à ce qu'on avait au minimum auparavant et donc ils prennent un emploi moins bien rémunéré moins intéressant peut être un peu difficile pour eux, hé oui, on va leur proposer un CDI et non, ils vont pas l'accepter parce que décidément, ils aimeraient bien retrouver ce qu'ils avaient avant et ils aimeraient bien travailler en fonction de leur état de santé de leur âge et ainsi de suite : qui sommes-nous, qui sommes-nous pour aller inscrire dans le marbre des choses qui interdiront ces choses-là et qui mettra en difficulté des gens dont nous ne connaissons pas la vie, qui sommes-nous. Monsieur Richard ensuite a demandé, a expliqué son vote. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi j'ai naturellement voté contre ces différents amendements mais permettez-moi un petit clin d'oeil à destination de Madame le rapporteur tout à l'heure, vous nous avez dit que le la proposition qui était faite par l'amendement Paco sur l'offre raisonnable d'emploi n'avait pas marcher enfin vous donniez un avis défavorable, parce que ça marchait pas, vous pouvez me certifier que cette proposition introduite en commission visant à supprimer l'ARE à des personnes qui refusent 3 fois un CDI à l'issue d'un CDD va mieux marcher que l'offre raisonnable d'emploi, permettez-moi d'en douter, parce que ça me paraît être autant une bouteille comme dit une usine à gaz, je vais lire que l'offre raisonnable d'emploi. Madame mon jeu. Oui, et puis peut-être qu'on pourrait renverser la situation, c'est-à-dire quand même ce que cette personne ne s'est vu proposer 3 fois un CDD, c'est quand même à l'origine cela et je rappelle que ce qui coûte quand même à l'assurance chômage, ça a été dit, alors on a parlé de milliards je crois mais je crois que c'est beaucoup plus, ce sont les contrats courts, ce sont les séparations comme ça qui coûtent à l'assurance chômage, donc moi ce que je propose, c'est qu'on oblige les employeurs à proposer trois fois un CDI. et de la Commission et du gouvernement, quels sont ceux qui y sont favorables, qui votent pour ces amendements. Quels sont ceux qui y sont opposés.

Merci monsieur le président, à l'inverse de l'eau, donc de l'objet de l'objectif de l'article 1er à qui veut pénaliser les salariés en CDD, cet amendement vise à encadrer les contrats de travail à durée déterminée afin qu'il cesse d'être utilisé comme un mode de gestion de la main-d'oeuvre des entreprises pour qui les CDD constituent parfois des variables d'ajustement, il est ainsi prévu de limiter le nombre de personnes en contrat à durée déterminée à 10 % de l'effectif global dans les entreprises d'au moins 11 salariés, je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, effectivement, c'était un amendement qui réécrit les dispositions du code du travail relatives au cas de recours aux contrats à durée déterminée de manière à les limiter en particulier prévoit que le nombre de salariés occupés en CDD pour cause d'accroissement temporaire ne peut excéder 10 % de l'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année précédente, bon c'était un amendement qui nous paraît être excessivement rigide et, de surcroît, de surcroît, il supprime l'article permettant de conclure des CDD au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, privant ainsi de base juridique certains contrats aidés pour tout ça, c'est donc un avis défavorable, monsieur le président.

Quels sont ceux qui sont contre. Et il n'est pas adopté, nous avons ensuite cet amendement en discussion commune, donc c'est un peu moins dur que la dernière fois nous commençons par l'article l'amendement 95 du gouvernement. Merci Monsieur le Président l'amendement 95 et celui que j'ai évoqué il y a un instant, il vise à proposer au Sénat, supprimer la disposition adoptée en commission des affaires sociales qui permettrait le retrait de du droit à l'ère en fonction du refus de trois CDI au cours de la même année, je m'explique, en un mot, nous avons une première difficulté qui est une difficulté pratique cela signifie malgré les efforts de la commission des affaires sociales du Sénat, une procédure de notification par les entreprises de croisement des systèmes d'information qui rend assez hasardeux et en cela je rejoins ce que disait monsieur le sénateur Richard sur la mise en oeuvre d'un tel, dispositif qui plus est, à l'échelle d'une seule année et et je pense véritablement que le dispositif peinerait malgré toutes les bonnes volontés exprimées sur le côté pratique à être opérationnel, sauf au risque de créer une procédure extrêmement lourde pour les entreprises en terme de déclarations et pour Pôle emploi de suivi des déclarations de CDI puisqu'on pourrait aussi imaginer qu'un même demandeur d'emploi

mais au-delà de la difficulté pratique au-delà des procédures, au-delà de la quasi-incapacité à mon sens de nos services à assurer rapidement le suivi d'une telle situation, cette disposition pose aussi un problème de principe, problème de principe car sans forcément reprendre les choses avec la même verve que Madame tout à l'heure, je considère que lorsqu'un un salarié recruté en contrat à durée déterminée va au bout de l'engagement qu'il a signé, tiens, la totalité des engagements contractuels sans les rompre sans faillir à l'engagement qui est le sien, il n'y a pas lieu de de le sanctionner, c'est une situation très différente à nos yeux de l'accession de l'abandon de poste, l'abandon de poste, c'est une rupture unilatérale d'un engagement contractuel sans crier gare, si vous me permettez cette expression en mettant le chef d'entreprise dans l'embarras par une disparition du jour au lendemain, le fait de ne pas souhaiter poursuivre à l'issue d'un contrat à durée déterminée, quand bien même, et ça fait d'ailleurs partie de la difficulté que de garantir l'équivalence des conditions proposées dans le CDI par rapport au CDD, mais le fait de ne pas souhaiter continuer alors qu'on a tenu l'intégralité de ses engagements contractuels ne me paraît pas de nature à constituer une forme de fautes ou d'erreurs et donc ne pas devoir être sanctionné, je précise que nous avons un travail à réaliser, cela a été dit tout à l'heure sur la question de l'eau et des possibilités de sanctions en cas de refus du neuf raisonnables d'emploi mais je renvoie là à l'article 6, telle que cela a été évoqué, et donc dans l'attente et qui plus est, pour une période d'application qui serait une période de 14 mois je sollicite d'adoption de cet amendement et donc la suppression de ces dispositions, privant de l'accès à l'ARE les titulaires de CDD, refusant à 3 reprises dans une année, l'accès un CDI. Nous avons un amendement identique présentée par notre collègue Martin lévrier. Merci monsieur le président, je ne vais pas redire ce qu'a dit brillamment de notre Ministre je vais poser quelques questions qui qui moi me soucie à travers à travers la logique que propose l'amendement de l'amendement de de la commission, pardon, si on se met du côté de l'employeur, l'employeur doit donc ne notifier à Pôle emploi mais notifié quoi et comment c'est le 1er sujet qui me paraît très important parce que, est ce qu'il doit notifier la raison du refus du salarié et ce qui doit donner toutes les pièces justifiant qu'il a proposé un CDI ou juste informé,

pour que des gens en CDD, ils ont des bonnes raisons dans 90 % donner un chiffre, c'est idiot parce qu'il y a, il y a pas de il y a pas d'analyses faites dessus mais la grande majorité des gens qui refusent un CDI ont des bonnes raisons, donc on s'attaque à un aléa et non pas à la logique et on complexifie le code du travail à travers ça, mais combien même on le fait qu'une personne qui se retrouvent sans allocation parce qu'il aurait refusé 3 CDI vers qui se retourne-t-il s'il vous le contestez vers Pôle Emploi vers un des 3 employeur donc comment l'employeur doit justifier le fait que ça a été refusé, on est en train de mettre en place une usine à gaz pour les employeurs et une usine à gaz aussi pour les allocataires qui aurait un refus à cause de ça, donc je trouve que nous voulons aller vers le plein emploi, on doit fluidifier cet ensemble et là on le complexifier à loisir parce qu'on s'imagine que par principe, les gens qui refusent et CDD sont des gens qui veulent profiter de vacances, je, je ne suis pas dans cette, dans cette

Monsieur le président, madame la présidente, mesdames, messieurs les rapporteurs donc si vous voulez, cet amendement donc indique que la commission a introduit par ce nouvel Arctic la notification alors pour l'emploi dont refus de CDI au terme de CDD parmi les critères indiqués pour qu'un tel refus soit ainsi comptabilisés, celui de la rémunération et au au moins équivalente à essentiel pour sécuriser le dispositif à la fois pour les entreprises et les salariés cependant la rédaction actuelle ne précise pas que cette notion doit s'entendent pour une durée de travail équivalente, c'est tout l'objet de cet amendement, merci. merci président alors l'article 1er bis a adopté en commission sur proposition de nos rapporteurs ouvrent le principe de l'annulation des allocations chômage du salarié qui aurait refusé plusieurs fois sur une période donnée, que leurs CDD se poursuivent en CDI, je considère que le principe posé par la commission est opportun et je l'ai d'ailleurs soutenu en commission, cependant, nous ne disposons nous ne disposons pas des statistiques relatives tant à la durée moyenne des CDD qu'au nombre moyen de CDD par salarié sur 12 mois pourquoi on en met trois pour qu'on met sur 12 mois pour qu'on en met un comment on va le voir dans un prochain propose, enfin, que je vous suggère propose de conserver le principe mais confie à la prochaine convention d'assurance chômage, le soin de déterminer les critères, le temps restant entre l'adoption de ce projet de loi et la signature de la prochaine convention d'assurance chômage ou la publication du décret en Conseil d'État visé à la ligne à l'alinéa 1er de l'article 1er du présent texte permettra de collecter les données objectives afin de rendre ce principe opérant je voulais aussi préciser que j'avais en fait presque vingt cosignataires sur mon amendement, mais qu'une petite erreur technique clique oublié me fait apparaître seul donc je voulais m'en excuser auprès de mes collègues qui avaient cosigné cet amendement, merci bien. Merci de cette précision ensuite dans la série des amendements en discussion commune, nous avons l'amendement numéro 100 disque présente Monsieur le Gold. Merci monsieur le président, donc, l'article 1er bis à a introduit en commission vise à priver les salariés d'indemnisation du chômage en cas de refus répétés d'offres d'emplois en contrat à durée indéterminée au terme de contrats à durée déterminée, cet article ne semble toutefois pas distinguer les cas de recours au CDD aussi pour ne pas pénaliser les travailleurs saisonniers cet amendement propose de les exclure du dispositif proposé. Ensuite, nous avons l'amendement numéro 65 présenté par Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président, le présent amendement vise à remplacer le dispositif que nous jugeons comme particulièrement régressif de la majorité sénatoriale par le renforcement des pouvoirs du comité social et économique, en matière de recours aux formes précaires de contrat de travail, les contrats à durée déterminée, intérim par l'entreprise dans ce domaine, l'avis conforme du comité social et économique doit être requis pour pouvoir prévenir de manière effective, le développement de contrat atypique au sein du collectif de travail, voilà quel est le sens de notre amendement, je vous remercie.

pourquoi quand on regarde aujourd'hui l'actualité et quand on est sur nos chacune de nos circonscriptions, on a beaucoup de chefs d'entreprises qui nous disent : on a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvus. Donc à un moment donné, si on est d'accord pour se dire qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi non pourvues, si on est d'accord aussi pour se dire qu'après un CDD, la meilleure des solutions pour offrir du travail dans la pérennité, c'est d'offrir un CDI,

s'il refuse, il ne touche pas le chômage, il travaille ailleurs, s'il veut, mais il ne touche pas le chômage de façon à ce qu'on revienne à quelque chose qui soit : les vraies valeurs du travail à un moment donné le sens de l'histoire, c'est quand on fait un un contrat à durée déterminée, hé bien derrière quand il nous est proposé un contrat à durée indéterminée, c'est plutôt un Avantage qu'un inconvénient donc on revient à cette vraie réalité. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, en votre nom, j'ai le plaisir de saluer la présence dans notre tribune d'honneur. Une délégation du Sénat des Philippines, conduite par son président Monsieur Juan Miguel Fernandez Soubry cette délégation a été reçue par le groupe d'amitié France-Asie du Sud-Est, présidée par notre collègue Mathieu Darnaud, qui est dans la tribune, notre délégation, la délégation de nos visiteurs est en France jusqu'au 28 octobre pour un déplacement axé sur les thématiques de la sécurité alimentaire, de l'énergie nucléaire et de la Défense, il a visité hier le le chantier de la centrale de Flamanville et les chantiers de Naval Group, elle sera reçue ce soir par le président Larché et par le vice-président Roger Karoutchi investie sur les questions internationales, nous espérons que les rapports entre nos 2 Sénat s'intensifieront et seront au coeur de l'épanouissement des relations entre nos 2 pays dans une région indopacifique travailler, traversé par de vives tensions, monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est, permettez-moi de de souhaiter, en votre nom à tous, à nos homologues du Sénat, Philippe hein la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour.

reprenons. Sur un autre mode et donc je donne la parole à Madame, la rapporteure pour donner l'avis de la commission sur ces amendements en discussion commune qui sont cette. Alors merci monsieur le Président, je je vais. Je vais effectivement reprendre un peu amendement par amendement et non pas faire une un retour commun et je vais d'abord traiter les 2 premières amendement de la même façon le 95, ils sont 11, hein, qui sont les mêmes, hein, celle du gouvernement et celle de notre collègue Martin lévrier. Et je je vais du coup me permettent, monsieur le président, de, de, de répondre à notre collègue Madame Lubin : qui sommes-nous pour effectivement à un moment donné, considéré que l'on doit effectivement au terme d'un CDD

on peut bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi quand on est privé de façon involontaire d'emploi, je le répète, est ce quand on refuse un un CDI au terme d'un CDD, on est privé de façon involontaire d'emploi, la réponse est non, voilà ce que nous sommes, nous sommes des gens qui savent on lire tout simplement la 2ème chose. Monsieur le Ministre. Et ça me permet de faire aussi un petit clin d'oeil à mon à mon collègue est-ce qu'effectivement c'est difficile à mettre en pratique, peut-être que c'est difficile à mettre en pratique, mais si à un moment donné, quand c'est difficile à mettre en pratique, on s'y a-t-elle pas alors qu'on est d'accord sur le principe, ça veut dire que, excusez-moi de vous le dire : nous ne Servent pas à grand chose, je considère qu'à un moment donné, quand on a des ambitions, quand on a la volonté, le côté un peu opérationnel c'est du détail et cet anneau effectivement de le résoudre, donc à partir de là, c'est un avis effectivement négatif sur le 111 et sur le 95 du gouvernement en ce qui concerne l'amendement. Neuf de la commission, en ce qui concerne l'amendement neuf c'est un amendement qui vise, qui précise que la notion de rémunération au moins équivalence du CDI proposés à l'issue d'un CDD doit s'entendent pour une durée de travail équivalente c'est une précision qui nous sommes, qui nous semble utile, c'est donc un avis favorable de la commission, l'amendement quarante-cinq qui effectivement a 2 objectifs : le 1er c'est une non application contrat saisonnier de la suppression de l'allocation d'assurance en cas de refus du CDI répéter et le deuxième si un renvoi aux partenaires sociaux, du nombre de ces 10 refusé

l'amendement 110 de Madame Maryse Carrère c'est un amendement qui vise à une non application contrat saisonnier de la suppression de l'allocation d'assurance en cas de refus de ces 10 répéter, on est sur la même logique, hein, que que l'amendement que je viens d'énoncer c'est donc un avis défavorable de la commission, l'amendement 65 de Madame hein, pour se c'est un amendement qui vise à obtenir un avis conforme du CSE sur les modalités de recours au CDD et au travail temporaire, alors nous nous considérons que le CSE et consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, à ce titre, il est informé par l'employeur sur le recours aux CDD et au travail temporaire et puis émettre un avis sur le sujet, en revanche, il n'est pas un organe compétent pour déterminer la politique de recrutement de l'entreprise, c'est donc un avis défavorable quant à l'amendement 83 de monsieur du point messieurs Retailleau, vous comprendrez bien à travers mes propos que c'est un avis favorable de la Commission et du rapporteur. Bien, alors maintenant, le gouvernement se prononce donc sur cette série de cette enfin M6 le plus le sien. Merci monsieur le président, le gouvernement maintient évidemment le l'amendement numéro 95 de suppression de ces 10. Position nous considérons, je l'ai dit que c'est une question de principe et que lorsque un salarie engageant CDD est allé au bout de l'engagement contractuel en respectant le fait qu'il puisse être privés du bénéfice de la prime de précarité, telle que prévue par le code du travail nous paraît quelque chose de suffisant et il n'y a pas lieu de le sanctionner plus le code du travail prévoit déjà que lorsque l'employeur propose un CDI, avec les mêmes conditions, le même emploi les mêmes rémunérations et que celui-ci est refusé il y a possibilité de de ne pas verser la prime de précarité, cela m'amène évidemment à être défavorable à l'amendement 83 de de monsieur du plomb qui réduit de 3 à un refus,

l'avis du gouvernement, et est défavorable à 2 exceptions, c'est un avis de sagesse pour l'amendement numéro 9 de monsieur pu et le numéro 110 de Madame Carrère je répète l'opposition du gouvernement aux dispositions telle que prévue par le vote de la commission des affaires sociales, mais si, dans le cas de la navette ces dispositions devaient être maintenus les précisions apportées par Monsieur Capet Madame Carrère peuvent être utiles. Merci monsieur le ministre, alors j'ai une demande d'explication de vote de Madame Lubin et ensuite une de Madame là de Madame Le fait de savoir lire, ne nous donne pourtant pas la possibilité d'avoir toujours les éléments qui font que des personnes peuvent être amenés et j'ai cité un exemple tout à l'heure et c'est un exemple qui est fort répandue, donc le fait de savoir lire ne suffit pas pour que nous nous inscrivions cela dans la loi, je le maintiens, et puis, puisque nous sommes visiblement lancés dans une course à l'échalote, je voulais le dire après l'amendement numéro 83 mais je le dis maintenant moi j'ai une proposition à vous faire, nous n'avons qu'à supprimer les indemnisations chômage et l'Unédic comme ça, il y a fort à parier pour que tout le monde retrouve un emploi demain et pour que les 32000 et 320000 offres d'emploi, je ne sais plus combien non pourvus soit pourvu du jour au lendemain. nous allons nous prononcer d'abord sur les deux amendements du gouvernement et de Monsieur lévriers est ce qu'il y a des des explications de vote sur ces amendements là.

en attendant la date de sa formation et celui-ci peut enchaîner les CDD dits alimentaires et celui et ceux qui lui permet d'avoir des droits pendant sa formation en imaginant que malheureusement pour lui, on lui propose 3 CDI, il devra donc les refuser pour rentrer en formation, il n'aura plus le droit, que se passera-t-il le risque c'est qu'il n'entre pas en formation et donc ne sera pas former à un métier en tension, c'est un exemple parmi tant d'autres, cela revient donc à traiter les personnes qui ont rempli leur contrat, donc tenu leurs engagements, comme si elles avaient

comment on applique en fait le fait que ne de ne plus avoir de droits, s'il refuse un CDI, donc évidemment, je voterai pour les amendements présentés sur la suppression.

Ce qui est intéressant, c'est que quand on pousse justement le raisonnement et à la limite on dit au 1er CDD dès le 1er CDD s'il refuse le CDI qui est derrière, il doit rien touché.

et j'ai osé dire et ça a fait beaucoup de brouhaha que si vous faites un seul CDD et que toujours vous prévoyez derrière des CDI, c'est que vous prolonger, en fait, la période d'essai, c'est un contournement de la période d'essai, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mois de période d'essai, vous avez 3 mois, puis après vous proposez le CDI, il faut proposer le CDI tout de suite et effectivement, moi je suis d'accord que à la fin d'un CDD, si il y a un CDI, enfin, je suis d'accord, c'est dans le droit du travail qu'on paye pas la prime de précarité parce que effectivement on ne subit pas la précarité précarité qu'on a subi quand même pendant les 6 mois de CD de CDD, si vous avez voulu faire un prêt bancaire ou si vous avez voulu avoir un logement, donc il est vous proposer un CDI quand on propose un CDI, hé bien effectivement, il y a pas après la prime de précarité, mais l'emploi quand même qui a été proposé, c'est bien un emploi en CDD et je ne peux que que effectivement reprendre les termes les droits et les devoirs ont bien été de du côté des des 2 parties respectés, donc effectivement il n'y a pour un CDD, un CDI, et c'est que là où on voit toute l'absurdité de cette proposition.

Merci monsieur le président, oui je vais intervenir sur ces amendements en expliquant pourquoi je suis défavorable et puis en même temps, sera le gazon de dire pourquoi je suis favorable cet article 1er avec le renforcement un, un seul s'est dit d'abord, moi je suis dans une région de l'ouest de la France, ou à peu près partout dans toutes les zones industrielles, on trouve des

il a obtenu rapidement un CDD de 6 mois, avec 6 autres jeunes avec lui, donc c'était sept a commencé à à est de 6 mois et au bout de six mois il vient me voir en me disant j'ai un problème, je me suis fait avoir j'ai signé un CDI au bout de 6 mois, je dis : mais pourquoi tu t'es fait avoir parce qu'aucun des autres n'a signé le CDI et pourquoi ben tout simplement parce qu'ils avaient tous un projet, ils avaient tous à partir de là, un choix de pouvoir toucher les que sur le chômage, avant de revenir, reprendre un CDD puisque dans ce territoire, il est très facile de trouver des CDD et c'est ce que vivent au quotidien et donc c'est vraiment cette expérience qui me fait pousser à soutenir ces initiatives ces amendements parce que c'est le quotidien, le problème c'est pas le problème de l'emploi, on a une capacité à la fois la simplement le du temps de travail accompagner socialement les personnes le vrai sujet c'est l'adéquation de la vraie volonté pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que les entreprises s'y retrouvent et que les salariés, c'est trop, et je pense que c'est une bonne équation à la fois pour l'économie et programment la réinsertion. Merci monsieur le président, assez rapidement, je rebondis sur ce qu'a dit mon collègue mouillé et je et je, et j'ai déjà je connais aussi des exemples de ce type-là, mais on a aussi, dans ces cas-là, si on commence à rentrer dans les exemples d'autres exemples inversé, vous avez des employeurs, et j'en ai connu qui propose un CDI à un commercial par exemple, c'est le cas d'un commercial qui avait un CDD pour lui diminuer son salaire et ce qu'il est, ça existe et ce qui les non pas complètement, autre exemple, vous avez, vous avez, vous savez très bien qu'un CDD c'est très compliqué de l'arrêter et pour le salarié et pour l'employeur excessivement compliqué pour les deux c'est une bonne raison, aussi, pour certains d'employeurs que j'ai connu de transformer des CDD en CDI, pour se débarrasser des personnes et ce qu'il est légitime et est ce qu'on doit traiter ce problème là aussi moi je crois que là, on essaye de traiter des petits aléas sur une loi globale qui fonctionne plutôt bien ça me paraît, je le redis très dangereux de de complexifier ce système CDD, CDI ou alors quelque part, effectivement : posons-nous la question du rôle du CDD dans cette affaire, mais, mais, là, dans cette affaire, je, je, vraiment je, je suis certain que pour les employeurs, c'est pas une bonne idée, ce qu'on est en train de faire mais pas du tout une bonne idée.

Entendu donc je mets aux voix l'amendement 95 du gouvernement et l'amendement 100 on ça ne monsieur lévrier qui sont analogues, quels sont ceux qui sont pour.

pas adopté. Ensuite, nous avons donc l'amendement de Monsieur kaput qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement et ce qu'il y a des demandes d'explications de vote. Il y en a pas, je le mets aux voix, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Il est adopté, l'amendement de Madame Jacques a fait l'objet d'un avis défavorable de Madame la rapporteure et du gouvernement, et ce qu'il y a des explications de vote sur cet amendement. On ne voit pas, donc je le mets aux voix, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre n'est pas adopté l'amendement de Madame Carrère : avis défavorable de la commission et avis de sagesse du gouvernement. Et ce qu'il y a des demandes d'explications de vote non, donc je le soumet au vote, quels sont ceux qui sont pour cet amendement de Madame Carrère. Quels sont ceux qui sont contre. Il ne il n'est pas adopté l'amendement 65 de Manama pour se avec un double avis défavorable. Quels sont ceux qui sont pour.

Monsieur Ray Charles d'abord. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai dit tout à l'heure que j'étais sceptique en ce qui concerne la mise en oeuvre sans difficulté de la proposition introduite en commission, monsieur le ministre, a bien voulu abondait dans mon sens en reprenant le terme d'usine à gaz, hein, que j'avais un peu hésité à prononcer et pour le coup, ça va vraiment être une usine, une usine à gaz et je donne rendez-vous à celles et ceux qui vont voter cette proposition,

j'ai réfléchi à à la possibilité effectivement de donner une certaine efficacité à cette proposition de la Commission et la seule proposition possible c'est c'est c'est cet amendement du plan à partir du moment où on veut aller dans le sens indiqué par monsieur du plomb à savoir essayer de régler un tant soit peu les tensions sur le marché de l'emploi, à l'heure actuelle, je crois que c'est l'objectif de ce projet de loi, il faut avoir le courage politique d'emploi la privation d'emploi résulte du refus d'une proposition de contrat à durée déterminée, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut pas être ouverts aux demandeurs d'emploi dès le 1er CDI refusé je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, moi j'ai juste des questions la disposition telle que proposée aboutit à de nombreux effets de bord quid d'un couple dont l'un des 2 est au chômage et l'autre, c'est qu'il va être muté dans une autre région dans six mois avec cette mesure s'est assuré que le chômeur ne prendra aucun CDD au risque de perdre ses allocations puisqu'il devra assurément ne pas l'accepter ensuite qui dit que, par qui dit pas d'allocations chômage RSA potentiel sous 3 mois, alors ce sont des départements qui vont payer, d'ailleurs, on peut s'interroger sur la recevabilité, article 40 de cet amendement, qui va créer une charge de trésorerie pour les départements, enfin, constitutionnellement, je m'interroge : comment on justifie qu'on empêche la perception des allocations d'une personne qui a également participé à s'ouvrir des droits voilà donc je dirais que nous, notre groupe en tous les cas, ne votera pas pour

Que le président, Monsieur le Ministre, j'arrive pas bien à comprendre quel est le débat, on est à 7 % de chômeurs en France. On a des entreprises qui cherchent des salariés, on n'est pas en train de dire que celui qui refuse de CDD va se retrouver sans rien, non, on est en train de me dire que celui qui refuse ces dit derrière un CDD ne puisse pas toucher le chômage mais rien lui empêche d'aller travailler dans une autre entreprise. Purée mais quand est-ce qu'on va comprendre enfin dans notre pays que si on veut que les choses marchent, il faut créer de la valeur, si on veut pouvoir redistribuer, il faut créer de la valeur, si on veut créer de la valeur et qu'on ait plus personne dans nos entreprises, comment voulez-vous la créer et comment voulez-vous redistribuer en puisant dans la dette, on est à 3000 milliards donc à un moment, il faudrait qu'on sache un peu ce qu'on veut faire si on ne se dit qu'on a 7 % de chômeurs qu'on a 2 millions de personnes au RSA si on ne veut pas, à un moment donné, les inciter, on les oblige pas, mais si on ne veut pas les inciter à faire à l'État à faire aller au travail, mais comment on fera il y a qu'à continuer comme ça, tout le monde jouera le sport national qui consiste à prendre un CDD se dire à la fin et que j'ai un cellier ou j'en ai pas le but, c'est de toucher le chômage, hé ben continuons comme ça et on se posera des questions dans quelques années supplémentaires. Je crois que le Sénat est suffisamment éclairée peut se prononcer sur cet amendement 83 présenté par Monsieur. Du plomb et ses amis qui est l'objet d'un avis favorable de la commission est d'un avis défavorable du Gouvernement quels sont ceux qui sont pour.

je préfère un assis pour être sûr parce qu'on est à une voix près quels sont ceux qui sont pour.

Ce n'est pas adopté. Il y a égalité j'ai égalité. Hé bien, en cas d'ça n'est pas adopté. Et pour terminer, nous avons l'amendement dix de monsieur pu qui est présenté par Madame Mellow. Michel. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la commission a choisi d'inscrire dans la loi la possibilité de moduler les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture, ou le rechargement des droits et la durée des droits à la location d'assurance chômage, cependant, cet article ne précise pas comment ces modulations peuvent être opéré, ni par qui le présent amendement vise donc à compléter par l'article relatif au suivi financier du régime d'assurance chômage afin de préciser que le document transmis chaque année par le gouvernement au Parlement et aux partenaires sociaux, précisant les mesures à mettre en place pour atteindre l'équilibre financier à moyen terme peut faire apparaître des mesures de modulation, une telle indication permet Anne outre de préciser que les modulations son temps envisagé sur un rythme annuel afin d'épouser au mieux les évolutions du marché du travail tout en sécurisant les assurés merci. pour être efficace, la modulation de l'indemnisation du chômage en fonction d'indicateurs conjoncturels doit avoir un caractère automatique, elle ne serait donc pas conçu comme une mesure visant à corriger la trajectoire financière de l'assurance chômage, mais comme un mécanisme permet visant à lui donner un caractère plus incitatif en période d'expansion ou de tension du marché du travail et plus protecteur en période de ralentissement ou de récession, c'est le principe de la Contra cyclicité hein, mais même si nous partageons le souci d'améliorer la situation financière de l'Unédic, nous considérons que le mécanisme contracyclique n'est pas l'instrument approprié pour y parvenir, donc un avis défavorable de la commission. madame la présidente, souhaitez-vous une suspension. Monsieur le Ministre. Même avis que la commission donc défavorable, donc je soumets au Sénat l'amendement numéro 10 avec un double avis défavorable qui est pour.

De nos collègues du groupe CRCE et donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions de l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Donc, nous, le scrutin est clos. Alors voilà le résultat du scrutin. Si je peux recueillir un peu l'attention du Sénat. Nous. Votants : 343 exprimés 320. Pour l'adoption 215 contre 105 donc, cet article est adopté, nous allons poursuivre chers collègues jusque juste avant 20 heures si vous le voulez bien. Et donc, nous prenons les séries d'amendements après l'article 1er bis à et donc le 1er et un autre amendement de monsieur du plomb qui est le numéro 11 rectifié, qui a la parole. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, voilà un amendement qui ressemblent à peu près à celui qu'on vient d'étudier juste avant, si ce n'est qu'il a une petite différence et qui concerne les intérimaires aujourd'hui à quoi on assiste quand on est sur le terrain, moi j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent : on a des intérimaires qui font six mois d'intérim dans une entreprise à qui parce que content de les avoir, on leur propose un CDI et qui refusent, pour tout simplement avoir recharger leur droit au chômage et bénéficier du chômage, alors moi je dis pas que l'intérimaire est obligé de prendre le CDI, moi je lui donne deux choix : soit il refuse le CDI et donc dans ce cas-là, ben il continue de rester intérimaires mais dans tous les cas de figure, il ne touche pas le chômage, c'est-à-dire ce que lorsque un intérimaire qui a fait six mois dans une entreprise, aux mêmes conditions, à qui on propose un CDI, hé bien ne puisse pas toucher le chômage lorsqu'il le refuse ce même CDI. Alors l'amendement. 11 à l'avis de la commission madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président, alors écoutez je, je pense que la position ma position à celle de la commission va pas vous surprendre, nous sommes exactement dans la même logique, c'est ce que nous avons eu préalablement un intérimaire qui refuse un CDI est-ce qu'on peut considérer qu'il est privé de façon involontaire d'emploi, la réponse est non, donc c'est un un avis favorable pour cet amendement. Merci monsieur le président de la même manière le l'avis du Gouvernement est défavorable à l'amendement pour les mêmes raisons que sur le 83 relatifs aux CDD, j'appelle l'attention du Sénat sur le fait que si cet amendement était désormais adopter le traitement des salariés intérimaires sera finalement plus difficile ou plus sévères que ceux des salariés en CDD. Monsieur Chassaing, à la parole seul si vous voulez bien. Oui, monsieur le président, mes chers collègues, alors si vous voulez pour moi cet amendement, c'est pas le même que que les autres, hein, puisque les autres, on avait le droit de proposer refusé jusqu'à trois CDI là c'est différent, c'est quelqu'un qui a un choix de vie, c'est-à-dire que il, il prend un intérim, puis il s'arrête et ils préfèrent rester au chômage, mais le problème, si vous voulez, à partir du moment où on propose un CDI alors il a le droit de rester intérimaires d'accord, mais s'il s'arrête, alors qu'on a proposé un CDI pour aller au chômage, donc là je pense que franchement c'est quand même on, on doit pouvoir l'refuser sans problème, je rappelle que ces gens qui, tout à l'heure, j'ai entendu parler que les gens ne s'était précaires fragile mais là c'est pas du tout ça, si vous voulez, c'est des gens qui sont diplômés qui ne sont pas marginalisées mais qui souhaitent avoir un choix de vie, mais ça, ça les regarde, mais à ce moment-là, qui ne demandent pas de chômage, merci. Messieurs Savary. Oui, merci, moi, je voudrais remercier mon collègue d'avoir proposé cet amendement parce que je pense que on est dans une période où Monsieur le Ministre, vous voulez qu'on arrive à au plein emploi, bah il faut bien que les gens ils sont un petit peu quelque part inciter à travailler et ce qui me préoccupe notamment c'est toujours. La retraite. Voyez-vous, ces personnes-là qui font un choix que je comprends bien, moi je me souviens

après, je fais autre chose, et cetera, très bien, mais on est dans une société qui ne peut plus se permettent maintenant ce genre de liberté, me semble-t-il, donc il faut trouver un système incitatif parce que derrière on va payer la note, quoi, tout le monde va travailler plus pour équilibrer les systèmes de retraite parce que certains veulent travailler, moi, à un certain moment dans le dispositif sociétal en conséquence je me pense que je pense que cet amendement est un amendement qui rend service en incitant à un certain nombre de personnes a changé un modèle qu'on envierait presque si on était dans un état d'esprit à vivre de la société, à certains moments de son existence, donc je soutiens cet amendement. Je ne vois pas d'autres demandes d'explications de vote si Madame Guinness et ensuite monsieur le plan lui-même. Bah, ça va peut-être vous étonner, mais moi je vais voter cet amendement parce que en effet il y a un réel problème au niveau des des intérims au niveau surtout je dirais dans tout ce qui est sociaux, médicaux, où les gens sont complètement perdu parce qu'il y a pas le personnel, ils sont en CDI, arrête le CDI pour se mettre en en effet en intérim, donc là c'est vraiment pour moi de l'incompréhension, donc moi je voterai cet amendement. madame l'humain, sauf si vous voulez parler maintenant Monsieur du plomb. Oui, je, je veux bien Monsieur le Président, Monsieur le Ministre dire quelque chose au ministres. Ne pas régler ce problème des intérimaires s'est laissé la possibilité à toutes les infirmières qui sont dans les hôpitaux publics de démissionner, de rentrer dans une boîte d'intérim, de revenir dans le même hôpital en bénéficiant de de mesures supplémentaires en termes de salaire que celles qui sont leurs collègues quelques jours avant et de bénéficier au bout de 6 mois des droits recharger au chômage, c'est ça l'exemple qu'on donne quand on ne vote pas cet amendement ou quand, comme vous, vous êtes contre cet amendement, l'image du gouvernement, vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez dans les hôpitaux, vous ne réglerait pas le problème, si vous ne réglez pas ça cette possibilité là, parce que ça sera la gangrène de tous les systèmes. Non mais là vous êtes en train de parler d'une situation extrêmement particulière et sur cette situation extrêmement particulière, il faudrait pénaliser toutes, toutes les personnes qui travaillent en CDI, chers collègues, René-Paul Savary ce que vous avez cités sont des gens qui, effectivement, à un moment, faisait un choix de travailler tout le temps en intérim, mais étaient tout le temps en intérim, je vous ai laissé parler il il peu Pôle emploi finalement à cette époque-là, donc bon les, les, les, les infirmières dont vous parlez en ce moment où les aides-soignantes, il y a aussi un autre problème et j'aimerais bien que vous vous y attaquer à ce problème-là, c'est celui de l'auto-entreprenariat.

et qui ainsi vont faire gonfler le les Budgets des hôpitaux ou autre, moi j'ai même rencontré, je vais vous dire j'ai j'ai rencontré un artisan coiffeur qui me dit : bah, écoutez, j'ai j'ai, j'avais une salariée en CDD, elle s'est, elle, s'est elle s'est inscrite comme auto-entrepreneuse et elle va proposer ses services chez des employeurs, voilà où elle se fait rémunérer beaucoup plus que le SMIC et les employeurs en question n'ont pas d'autre choix que de, de, d'avoir recours à ses services, parce qu'effectivement, il ne trouve plus, et ça c'est le c'est le dévoiement du système de l'auto-entreprenariat et en plus c'est le miroir aux Alouettes pour tous ces gens qui vont là-dedans, donc moi je veux bien, si aujourd'hui les entreprises un certain nombre d'entreprises ne trouvent pas de demande de, de salariés, c'est aussi parce qu'il y a toutes ces choses là qui se mettent en place et contre lesquels on ne lutte pas, et pourtant c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, plutôt que de vouloir pénaliser absolument si c'est inscrit dans le marbre dans la loi, tous les demandeurs d'emploi qui à un moment seront concernés, moi je, je ne sais pas quelle mouche vous a piqué, mais je vous trouve vraiment extrêmement dur. on on est pas obligé de se prendre à partie mais Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président je j'entends un certain nombre d'arguments sur l'intérim dans le milieu médical, que ce soit pour des praticiens pour des infirmiers et effectivement avec une situation très particulière, liée à la démographie médicale mais mais l'intérim ne s'arrête pas aux seules professions médicales, il y a aussi des salariés intérimaires qui travaillent dans des entreprises où les dans lesquels les conditions de travail peuvent être extrêmement difficile, les mêmes entreprises qui, pour des questions d'attractivité, de conditions de travail ne trouvent pas d'autres personnels qu'en passant par des agences intérimaires, soit parce qu'ils ont ainsi accès à des personnels qui ne souhaite pas s'inscrire très longuement dans un emploi, soit parce que des primes de précarité liée à l'intérim, explique la possibilité d'aller vers ces emplois et et on les enfermerait par le refus du CDI, donc je je ne crois pas qu'il faille s'appuyer sur un exemple très criant qui est celui du domaine médical pour justifier cet amendement que je trouve particulièrement sévères pour les les salariés en intérim. Monsieur Seguin, vous avez demandé la parole. Oui, Monsieur le Ministre juste vous vont moi je comprends pas les arguments, je ne comprends pas vos arguments, parce que les infirmières, c'est un argument qui est criant la la personne si elle est dans un intérim et puis que ça lui convient pas son emploi, ça lui empêche pas de continuer à trouver un autre emploi intérimaire c'est c'est pas ça qu'on dit alors moi j'ai beau regarder le titre de votre projet de loi c'est en vue du plein emploi, mais chaque fois qu'on apporte des, des moyens pour pour aller vers le plein emploi vous botter en touche, donc je ne vois pas à quoi ça sert, ce texte, franchement je ne vois pas à quoi il sert en plus vous venez du budget, vous n'êtes pas sans savoir que grand nombre, moi je vois un exemple chez moi des entreprises de travaux agricoles, vous avez des intérimaire qui viennent pendant la période d'été qui sont conducteurs qui font des heures sup au maximum, on veut les embaucher derrière, ils refusent parce qu'ils veulent toucher le chômage par rapport aux aux revenus qu'ils ont eue pendant la période saisonnière, ça coûte une somme folle à l'État, vous êtes, vous étiez au budget, vous êtes pas sans savoir ce que ça coûte, et dès qu'on apporte des solutions, il y a plus personne, moi je ne comprends pas la position du gouvernement sur. Je vais Je vais mettre cet amendement numéro 11 de monsieur du plomb et de ses collègues, qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission et dans l'avis défavorable du Gouvernement quels sont ceux qui sont pour.

Il est adopté, nous passons à l'article 1er et nous avons d'abord un amendement de suppression du gouvernement. Qui va le défendre. Merci monsieur le président, la l'article 1er bis ah introduit par la commission des affaires sociales a pour objet de de prévoir au profit des agents et les employeurs territoriaux la la faculté de saisir le Centre de gestion de la fonction publique territoriale, pour qu'il se prononce après avis de la CMP sur des décisions individuelles. En matière d'indemnisation d'agents publics, démissionnaire de la fonction publique et en particulier de la fonction publique territoriale le problème est est manifeste et en réalité le sujet existe et je crois que cet amendement est adopté par la commission des affaires sociales, à l'initiative du questeur, Philippe Bas, qui pointe là une véritable difficulté une véritable différence de droit entre des demandeurs d'emploi en raison de leur statut antérieur différences qui sont assez peu justifiables, malgré tout, nous avons une difficulté de fonctionnement ou de mise en oeuvre de l'article puisque le Centre de gestion qui seraient ainsi consultés après la démission n'aurait ni légitimité ni véritables compétences pour apprécier l'effort de reclassements de la personne et la légitimité de cette même personne à bénéficier de l'allocation chômage, ce qui est une des conditions par l'instance paritaire régionale pour les démissionnaires du secteur privé et donc nous considérons que l'objectif de l'amendement et tout à fait louable puisqu'il s'agit d'harmoniser les droits de salariés ou d'agents publics, notamment dans la territoriale démissionnaire dans le cas de l'accès à l'assurance chômage, mais que le fait de passer par une consultation du Centre de gestion n'est pas opérant, donc c'est un un véritable chantier que nous devons mener, je remercie à nouveau Philippe Bas, le sénateur Philippe Bas, pardon d'avoir soulevé ce ce point parce qu'ils méritent d'être traités, il ne nous paraît pas opportun de traiter ainsi par contre évidemment cet engagement à pouvoir travailler sur ce sujet-là, à la fois avec les ministres en charge des collectivités, mais plus encore avec les le ministre en charge de la fonction publique, puisqu'il s'agit d'une harmonisation des droits concernant les agents publics, donc c'est la raison pour laquelle nous proposons cette suppression, non pas par désaccord mais plus par souci d'opérationnalité. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, j'ai j'ai aucune raison de remettre en doute votre parole, ceci étant, la liste des chantiers à traiter et longue on va rajouter un point supplémentaire, or on a une vraie difficulté aujourd'hui dans nos collectivités qui est peut être pas d'un an de très important, mais la réalité elle est laquelle nous avons aujourd'hui la majorité des agents qui sont dans les collectivités, ils sont des des agents de la fonction publique, prenant un ratio disons 90 % d'agents de la fonction publique et 10 % de CDD 2 CDI que font les collectivités, elle s'assure pour l'assurance chômage pour les 10 % le s'assure pas pour les fonctionnaires, elles s'en auto-assurance pour les fonctionnaires, or que se passe-t-il aujourd'hui, on a un certain nombre de fonctionnaires qui font le choix de démissionner, ils font le choix démissionné, ils partent dans le privé et puis au bout d'un moment, ça se passe mal dans le privé, ils vont effectivement taper à la porte de Pôle emploi en demandant effectivement l'allocation de retour à l'emploi que fait Pôle emploi il va regarder effectivement l'employeur qui a été sur lequel ses salariés a a été le plus longtemps en activité. Et il va apprécier si c'est qui va être effectivement celui qui va payer la location de retour à l'emploi et, en règle générale qu'est-ce qui va se passer à l'autre bout de la chaîne, vous allez avoir un maire qui va recevoir un petit papier et qui va lui dire : Monsieur Dupont, qui a démissionné de chez vous, il y a 4 ans en arrière, hé bien effectivement Dupont et pas du plomb, pardon, qui a démissionné de chez vous, il y a 4 ans en arrière, hé bien ce monsieur même s'il a démissionné, nous avons considéré qu'il avait le droit à l'allocation de retour à l'emploi, et en l'occurrence, il va falloir payer, croyez-moi, les maires qu'on rende compte, ils sont dans ces situations sont fous furieux en disant : mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et et qu'est-ce qui se passe effectivement dans les faits, Monsieur le Ministre, c'est qu'on a effectivement quelqu'un qui à un moment donné, se trouve dans une situation qui est une situation très atypique qui va apprécier cette situation, c'est en règle générale, le directeur régional de Pôle Emploi

que cette appréciation soit faite par le centre de gestion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça soit les maires et donc en l'occurrence les pères P I R E S des maires qui, à un moment donné puisse apprécier la situation et non pas le directeur régional de Pôle Emploi, voilà ce que propose cet amendement très honnêtement Monsieur le Ministre, je peux comprendre qu'il a peut-être d'autres perspectives aujourd'hui, c'est la seule solution que nous ayons trouvé. Pour effectivement résoudre ce problème, parce que croyez-moi les maires qui reçoivent ce papiers sont en règle général très mécontents, je ne voudrais pas ajuster cette liste à la liste important des chantiers à conduire, donc je propose donc que cet amendement soit en tout cas en ce qui concerne notamment amendement de retrait, c'est un avis défavorable de la commission parce que je propose qu'on traite le sujet quitte après à ce qu'on puisse l'apprécier de façon différente, donc c'est un avis défavorable à votre amendement de suppression. Monsieur Ministre. un mot monsieur le président, si je ne veux pas qu'il méprise le le sujet, il existe, il est fort et tout le monde en convient : nous avons eu l'occasion de d'échanger, nous considérons que c'est pas ainsi qu'il doit être traité nous pensons plutôt que les modalités d'auto-assurance qui sont propres au secteur de la fonction publique territoriale, y compris dans le cadre de quelque chose de plus collectif pour justement éviter le phénomène que vous avez ainsi décrit doivent être mises en oeuvre crayon et nous pensons que le dispositif proposé si il a un objectif que nous partageons ne ne sera pas opérationnel, c'est la raison pour laquelle je je maintiens cet amendement, c'est un sujet à traiter et vous avez raison de le rappeler Madame la la rapporteure pour finalement heureusement assez, assez peu de des personnes concernées, donc ça n'est pas forcément le le point nodal du texte, mais je crains vraiment que ce ne soit pas opérationnels, d'où le maintien de cet amendement. Madame Di Falco, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, monsieur président je suis assez embêté sur ce sujet-là, parce que je comprends complètement le le sujet posé par Philippe Bas c'est un vrai sujet et qui est très problématique pour les communes que vous dites, madame la rapporteure, qui reçoit ce papier et en même temps je comprends aussi la position de Monsieur le Ministre parce que réellement les cendres de gestion ne peuvent traiter des sujets que des des agents qui appartiennent encore à la fonction publique, or la personne a déjà démissionné, elle n'est plus dans la fonction publique, donc je comprend également le le le point de vue de Monsieur le Ministre, non moi ce sujet existe et vous avez raison d'insister sur le fait qu'il faut le traiter alors peut-être il y a des solutions à trouver et donc pour pouvoir effectivement se forcer à trouver des solutions, il faut peut être maintenir quand même ce ce, ce dispositif, même si je pense qu'il a des difficultés en tant qu'opérationnel peut-être Monsieur le Ministre, faut-il envisager que dans ces commissions qui statue sur le droit des salariés, il y a des représentants des collectivités, peut-être aurait-elle des arguments à donner, je ne sais pas, c'est une piste de réflexion également en tout cas je pense qu'effectivement, il faut vraiment traiter le sujet. Monsieur le Ministre. Pardon, je ne veux pas allonger le le débat mais je crains que la proposition de madame la sénatrice se au fait que l'instant paritaire dans les instances paritaires, il y a rarement pour ne pas dire jamais de représentants des des collectivités, ça peut être un sujet de débat et le nombre de cas concernés tellement marginal mathématiquement par rapport aux autres que la présence ne serait pas forcément opportune, ça ça ça se regarde, mais je ne pouvais pas ne pas réagir puisque le l'intervention de madame Di Folco me me rappelle quelques débats que nous avons, il a quelques années, à propos des cendres de gestion et la fonction publique territoriale. Je mets aux voix donc l'amendement de suppression du gouvernement qui fait l'objet d'un avis défavorable de la commission, quels sont ceux qui sont pour. pour. Quels sont ceux qui y sont opposés. Il est repoussé, nous avons un autre amendement de monsieur Lévy qui l'amendement 109 vous avez la parole cher collègue. Oui, monsieur le président, monsieur le Ministre, mes chers collègues par cet alinéa la loi prévu d'enfermer les 10 Létizi des agents territoriaux dans le cadre de l'Arctique elle 557 1 du code général de la fonction publique, dans un délai de 3 mois et d'en faire de même pour le délai de réponse des centres de gestion or afin d'aligner cette disposition sur le régime classique du contentieux administratif et des délais de droit commun de la procédure administrative, il semblerait plus opportun de faire passer ce délai de 3 mois, un délai de 2 mois en effet, sur l'ajustement permettrait d'aligner les nouveaux délais prévus par le dit alinéa avec le délit traditionnel de la procédure administrative qui est de de mois une telle réajustements serait gage de lisibilité pour les justiciables, dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice. Madame la rapporteure votre avis. Oui, merci Monsieur le Président, hein, c'est un amendement qui vise à réduire à deux mois les délais de saisine et de réponse du Centre de gestion, c'est vrai que nous étions préalablement nous sur trois mois, enfin en tout cas le le le questeur pardon Philippe a été sur sur 3 mois, mais c'est vrai que la la durée de moi en règle générale, le délit de principe de recours contre une décision administrative donc l'alignement ne paraître plutôt opérant et c'est donc à l'avis favorable de la commission. Je mets aux voix cet amendement cent neuf de Monsieur Lévy avec avis favorable de la commission est défavorable du Gouvernement quels sont ceux qui sont pour. pour. Il est adopté, et l'article 1er bis donc être soumis au vote de demandes d'explications de vote, donc je me soumets au Sénat, quels sont ceux qui sont favorables. Quels sont ceux qui sont opposés. Il est donc adopté. Nous poursuivons encore un peu à l'article 1er bis à grand nous avons trois amendements identiques de suppression, le 1er est celui de Madame Lubin, le numéro 16. Nous sommes totalement opposés au durcissement de la réforme de l'assurance chômage, voté à l'Assemblée nationale qui vise à considérer démissionnaire tout salarié présumé fautif d'un abandon de poste, et aussi le privé de toute indemnisation du chômage, parce que les données manquent pour légiférer, aucune donnée objective, encore moins chiffré n'est avancé, y compris par les rapporteurs pour justifier de la nécessité de légiférer sur les abandons de poste, le risque est de générer des impacts dramatiques pour les salariés et de compliquer la mise au jour des raisons pour lesquelles l'abandon, d'abandon de poste, il y a potentiellement liées aux caractéristiques inhérentes du management ou des conditions de travail expérimentée par le travailleur un abandon de poste quid par exemple du salarié qui ne serait plus payé par son employeur, mais toujours sous contrat de travail, la charge de la preuve incomberait aux salariés devant les prud'hommes, ce qui rend la procédure de facto difficilement opérante au vu des délais et des coûts d'une telle procédure nous considérons donc elle emporte en réalité plus de risque juridique pour l'employeur, qu'elle ne le sécurise à l'opposé de l'objectif recherché. Par les partisans de cette mesure, je voudrais préciser que lorsque cette mesure a été votée, elle m'a interpellé parce que, effectivement, nous savons que salarié qui abandonne son poste et ça pose des problèmes à l'entreprise, et ça ça ça peut poser des problèmes importants et donc avant de me faire un avis j'ai consulté notamment des des avocats en droit du travail et ce qui m'a été dit, c'est que, en fait, une fois de plus, aucune statistique devient nous viennent dire que les abandons de poste sont en constante augmentation, comme j'ai pu l'entendre de la part de notre rapporteur en commission des affaires sociales, voilà et donc je ne vois pas pourquoi il y a des abandons de poste, alors je sais que vous avez prévu des protections, mais quand même un employeur qui cesse de payer un salarié, ça s'est vu, ça s'est vu qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là, le salarié, quelle solution, a-t-il et ça c'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres attention donc de ne pas gravé dans le marbre des choses qui pénaliseront tout un ensemble de salariés pour finalement quelques-uns qui tire sur la corde. CRC Madame Cohen, vous avez la parole 68. Merci monsieur le président, à l'Assemblée nationale, les députés LR L et et d'ailleurs le RN ont voté cet article qui prévoit la créance, la création d'une présomption de démission en cas d'abandon de poste dans le but d'écarter de l'assurance chômage, toutes ces personnes qui n'ont d'autre choix que d'abandonner leur poste, ma collègue vient de d'exposer un certain nombre d'arguments donc contre 7 pour la suppression de cet article, pourtant, l'abandon de poste, c'est souvent contraints il constitue le dernier recours pour le salarié ou la salariée qui lui permet de se protéger, par exemple, face à un employeur brutale des collègues ou une organisation de travail dangereuses, c'est aussi un dernier recours, dois-je le rappeler ici pour échapper au harcèlement très souvent l'amende l'abandon et même négocié entre l'employeur, qui refusent de signer une rupture conventionnelle et le salarié qui ne veut pas démissionner comme je l'ai souligné dans la discussion générale, la procédure déséquilibré pour les salariés est inadapté à la réalité de la justice prud'homale, il est illusoire de penser que les salariés qui souhaitent contester leur démission pourront obtenir même en référé une réponse dans le délai d'un mois en supprimant l'indemnisation au chômage, vous allez conduire les salariés dans des situations de conflit à devoir rester en poste avec cet article, vous allez aussi conduire donc ses salariés, a déposé des arrêts maladie et en quelque sorte des porter le problème vers l'assurance maladie pour l'ensemble de ces raisons, donc nous demandons la suppression de cet article. écoutez cet article, ajouté à l'Assemblée nationale, il faut savoir pourquoi elle trouve sa raison d'être dans le contexte de la mise en place du dispositif bonus malus en en assimilant les abandons de poste à une présomption de démission l'objectif ici est de les exclure du décompte du taux de séparation, cependant, il convient de pointer l'insécurité juridique de cet article, ajouté à la va vite pour des raisons opportuniste, la jurisprudence est constante, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté non équivoque du salarié et d'ailleurs cet article rentrerait en contradiction avec la convention 158 de l'OIT, les raisons on déporte le débat, hein, maintenant qu'on a vu que c'était pour le bonus malus et pas pour autre chose, mais les raisons des abandons de poste ils sont multiples, ça a été évoqué avant elles peuvent effectivement résulter de situation professionnel dégradé

mais il a pas la main, hein. Donc c'est pas tout à fait la même chose et c'est vrai que souvent, c'est une réponse au refus d'une rupture conventionnelle et surtout bien sûr parce que, aussi, de toutes ces raisons-là la démission n'ouvre pas de droits et que l'annonce par Emmanuel Macron, qu'il allait ouvrir les quatre démission ouvrant les droits au chômage a été une vie une une vaste illusion et a produit beaucoup de désillusions, donc une solution durable et non des les Terres parce que je trouve cette situation assez des les délétère résiderait dans l'élargissement vraiment des motifs légitimes de de démission ouvrant droit au au chômage, et y compris jusqu'à une véritable sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie dont on a déjà parlé, et du côté des employeurs : ben c'est vrai qu'il faut et j'y reviens toujours il faut résoudre le problème des secteurs sous tension et quelquefois fois très faible attractivité plutôt que de contraindre les salariés soient les rejoindre

évoqué le fait qu'il en est de plus en plus j'ai franchement j'ai pas les chiffres, alors si, si, je me suis exprimé ainsi non pas moi, d'accord, OK, parce que, effectivement, on a, on a très peu de chiffres sur le sujet. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, de de quoi parle-t-on, on parle de présumé démissionnaire, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et qu'qui ne reprend pas le travail, après, je dis bien après avoir été mis en demeure de le faire et en prévoyant une voie de recours devant le conseil des prud'hommes c'est de ça dont on parle, de quoi est-ce qu'on ne parle pas, il existe et il existera toujours même après ce texte, des modifie des des motifs ou légitime, qui ne peuvent pas être qualifiées d'abandon de poste, le droit de retrait, le droit de grève, des problèmes d'état de santé des problèmes d'instructions contraires à la réglementation, ce n'est pas de l'abandon de poste, ce n'est pas de l'abandon de poste, donc on ne parle pas de ça dans cette dans ce dans cet article, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, l'abandon de poste n'existe pas dans le code du travail, donc la jurisprudence la jurisprudence considère effectivement que l'abandon de poste n'est pas une démission donc ça veut dire quoi, ça veut dire que quand on abandonne son poste, ce qui, permettez-moi de le dire, n'est quand même pas très élégant, on plante, pardon de le dire, ses collègues sur une situation et parfois c'est un peu compliqué, mais ça veut dire que l'abandon de poste est mieux traité que la démission est-ce que c'est juste la réponse est non, c'est est-ce que cet amendement qui précise effectivement. Qu'il faut considérer l'abandon de poste comme une présomption de 10 Mystery de démission et juste, la réponse est oui, c'est donc un avis défavorable à vos trois amendements. Monsieur le Ministre votre avis. Défavorable pour les raisons que j'ai évoquées en réponse à la discussion générale et par ailleurs j'ai indiqué que la les ajouts de la commission des affaires sociales, sécuriser le dispositif qui était bienvenue. Donc, après 2 avis défavorables je soumet au vote du Sénat ces trois amendements de suppression, quels sont ceux qui sont pour. Avis opposé. Sont pas adopté ensuite vous avez un amendement 27 de Madame Luba qui va le présenter. Oui, toujours avec les, les, les mêmes raisons, donc un amendement de repli, nous proposons que l'employeur est à démontrer qu'il n'ait commis aucune faute à envers le salarié et ce après une procédure contradictoire, cet amendement, nous semble l'encadrement minimal à apporter à une telle régression pour les travailleurs, d'autant que la procédure ainsi créé avec cette présomption de démission initialement dans le but de sécuriser les entreprises risquent d'introduire plus d'insécurité juridique pour l'employeur, en réalité, du fait même de son applicabilité pour soit disant clarifier l'abandon de poste est en effet introduite de équivaut qui, cité dans le régime de la démission elles-mêmes. La commission madame la rapporteure. Merci monsieur le Président, donc cet amendement effectivement vise à ce que l'employeur, il a démontré qu'il n'ait commis aucune faute envers le salarié et ce après une procédure contradictoire préalable à la présomption de démission pour abandon de poste, alors je je rappelle simplement, hein, que la présomption de de démission, l'article 1er Lisa est une présomption simple : il suffira aux salariés de démontrer que son absence est justifié ou légitime pour empêcher la qualification de démission lorsque l'absence, je le répète, injustifié du salarié résulte d'une faute de l'employeur, je les ai cité tout à l'heure, la jurisprudence considère déjà qu'elle ne peut être qualifiée d'abandon de poste, il ne paraît pas donc pas souhaitable que l'employeur soient contraints de démontrer son absence de foot, c'est donc un avis défavorable à cet amendement. amendement. Le ministre. Je je vous ai mal entendu si défavorable, l'accent tonique en langue française ne tombe pas toujours bien donc sur cet amendement vingt-sept je n'ai pas de demande d'explications de vote, quels sont ceux qui sont favorables à cet amendement de Madame Lubin. Quatre cinq six voilà. Quels sont ceux qui sont opposés. Pas adopté ensuite, nous avons un amendement de nos rapporteurs numéro 114. Rédactionnel, monsieur le président.

Il est défendu madame madame la rapporteure faisait pouvoir de dire de quoi il s'agit. Alors effectivement c'est un amendement qui énonce le fait que la rupture du contrat qui résultera de la présomption de démission pour abandon de poste sera systématiquement considéré comme une rupture à Buddy abusive du contrat imputables, salariés et sur ce fondement, le salarié devra donc payer des dommages et intérêts à l'employeur, bon là on va quand même un peu loin dans un autre sens, donc c'est un avis défavorable de la commission. Même avis. Quels sont ceux qui sont pour. pour. Quels sont ceux qui sont contre, voilà, il y en a plus, donc il n'est pas adopté, nous pouvons nous prononcer sur l'article 1er bis à dans son ensemble, pas d'explication de vote. Quels sont ceux qui sont pour. contre. Il est adopté.

Il est défendu, donc, même topo, on va le savoir de quoi il s'agit. dans le cas des enjeux liés à l'abandon de poste, alors le code général des impôts autorise déjà les entreprises à déduire de leurs résultats fiscal des provisions destinées à faire face à un certain nombre de pertes ou charge donc c'est un avis défavorable de la commission. Madame. Je le mets aux voix qui sont ce qu'elles sont Ah, par contre, voilà, il y en a plus d'un, donc c'est réglé, nous arrivons à l'article de donc, on a fait quand même un peu de chemin, je vous suggère qu'on se prononce simplement sur les trois amendements de suppression et que, on passe à la suite après dîner. Donc nous avons un amendement de suppression de Madame Lubin, qui est numéro 17. c'est un amendement donc qui vise à supprimer l'article de cette disposition, consistant en l'autorisation de communiquer aux employeurs les données personnelles à l'origine du malus sur les contrats courts pose question au regard du RGPD et du respect de la vie privée des effets pervers tête ont ainsi été observés aux États-Unis lors de la mise en place d'un bonus-malus similaire en effet si les employeurs peuvent avoir accès aux données personnelles des fins de contrats générant le paiement d'un malus, ils peuvent alors demander à ses salariés de ne pas s'inscrire à Pôle Emploi et leur promettre une réembauche ce afin de minimiser le montant de ce malus, il y aurait alors un contournement de l'objectif initial de l'assurance chômage, nous proposons de répondre à cet effet pervers par la suppression de cette autorisation de communication, nous entendons également revenir sur la minoration du bonus-malus visant à lutter contre les abus de contrats courts introduit par les rapporteurs, les modalités d'application et les taux de contribution fixée n'ont aucun effet des incitatifs à l'usage des contrats courts, il convient donc de renforcer ce dispositif plutôt que de l'alléger. Merci madame ah pour se même amendement numéro 72. Monsieur le président, le gouvernement a fait beaucoup de tapage publicitaire autour du bonus-malus, des entreprises qui ont recours aux contrats à durée déterminée, la première chose à dire ici, c'est que les contrats courts ont été encouragés par la majorité en 2017 au moment des lois de travail qui ont singulièrement accru les possibilités de recours aux formes précaires pour notre part, nous sommes toujours montré favorable au malus des entreprises pour inciter à favoriser le recrutement CDI mais nous ne comprenons pas qu'il existe un bonus dès lors qu'il ne s'agit que d'un comportement vertueux, mais pas d'un comportement vertueux, mais simplement le respect des règles, c'est comme si l'ont félicité les entreprises de ne pas avoir recours au travail dissimulé, d'autant que les contrats courts continue de bénéficier d'exonérations massives de cotisations sociales, selon la Cour des comptes en 40 ans, la perte de cotisations sociales dans le financement de la protection sociale est passé de 90 % à 38 %, ce qui pose un réel problème de financement pour la seconde chose, c'est que le dispositif de bonus-malus est particulièrement restrictive puisque, sur le 1000000 d'entreprises en France, seulement 18000 ont été concernés par le bonus-malus et seulement 6000 par un moule mais c'est déjà trop pour la majorité sénatoriale qui a limité le bonus-malus aux fins de CDD de moins d'un mois et limiter la majoration des entreprises à plus ou moins 0,5 points en clair peanuts, la droite sénatoriale a supprimé toute efficacité au système et restreint le périmètre de bonus-malus, de sorte qu'il ne concerne quasiment plus aucune entreprise pour toutes ces raisons, nous demande la suppression de cet article, je vous remercie.

par des dispositions modifiant sensiblement le système de bonus malus pour en limiter la portée l'article limite la majoration de cotisations sociales pour les employeurs abusant des contrats courts à 0 5 point de pourcentage, il nous apparaît que la faiblesse du montant des majorations privera aura très certainement le dispositif de son effet dissuasif, a fortiori sur les grandes entreprises car c'est minorer le coût pour l'Unédic du comportement des entreprises visées par le malus, dont le taux de séparation, rappelons-le, du fait de leur comportement d'employeurs est supérieur à la médiane de, de, de 7 secteurs déjà caractérisée par un taux élevé, hein, donc c'est une double couche. il faut pénaliser de plus l'article limite le calcul du malus à la prise en compte uniquement des CDD de moins d'un mois, cette restriction visant à sortir tous les CDD aider un mois et un jour, fait peu de cas de la définition de l'emploi dit durable, c'est-à-dire un CDI ou au moins un CDD d'au moins 6 mois, les périodes d'inactivité des salariés entre les contrats de si courte durée pour atteindre les 6 mois de filiation seront eux bien pris en compte, en faisant chuter le calcul de leur allocation, mais il est vrai qu'il serait par la réforme, plus à même d'exiger des CDD d'une durée plus longue donc cet article, le dispositif alors que la réforme durcit l'accès à l'assurance chômage pour les demandeurs d'emploi et encore plus après le passage au Sénat, dont de très amendement se propose de supprimer l'article de avant de rendre au malus un semblant un semblant de pertinence. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président, ces trois amendements visent à supprimer l'article de hein, je rappelle que l'article de visa éclairer les employeurs qui sont frappés par le dispositif du malus, c'est du bonus, on peut imaginer que c'est plus ceux qui sont concernées par le malus qui vont être intéressés, intéressés par les données qui sont encore. Tu es en leur apportant les données nécessaires, y compris la liste des personnes concernées par la fin de contrat, j'allais presque dire Monsieur le Ministre, on aurait presque pu prévoir en 2018 parce que, franchement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, chers collègues, le peanuts, chers collègues, c'est parfois 150000 euros, le pilote, on a eu quand même en audition, une entreprise qui avait effectivement un malus de 150000 euros, bon, c'est quand même pas rien du tout quand même à payer, et elle ne sait même pas pourquoi elle paye, elle, à l'aveugle très franchement, il est logique qu'elle puisse avoir un moment donné les éléments à la limite si c'est vertueux tant mieux mais à Nîmes a minima pour justifier cette somme, c'est donc un avis défavorable de deux sur ces amendements qui visent à supprimer l'article de. monsieur le président de sommes un peu dans le même cas que sur un des articles précédents les amendements sur nos amendements de suppression de la totalité de l'article, nous sommes favorables au maintien de l'article de dans sa rédaction initiale, je l'ai dit, nous ne sommes pas favorables aux restrictions apportées par la commission des affaires sociales au dispositif de bonus-malus tant sur la nature des contrats prise en compte que sur l'ampleur de la variation de cotisation mais au delà de ce de ce désaccord que j'exprimerai par la défense d'un amendement tout à l'heure je ne peux pas nous être favorable à la suppression de l'article tout entier donc défavorable. On parle d'un amendement de bonus malus et en employant l'expression de peanuts, on va se demander si l'article de la Constitution, qui rappelle que la langue de la République française et le Français est un peu perdu de vue, non, c'est une plaisanterie, je mets aux voix ces trois amendements, des collègues de suppression de l'article de quels sont ceux qui sont pour. Et quels sont ceux qui sont contre, ils ne sont pas adoptés donc comme vous partez ensuite. Pour un tunnel de 8 amendements en discussion commune, je pense que la raison m'amène à suspendre la séance, elle sera reprise à 21 reprend 21 heures 30 pour la suite de l'examen du texte, la séance est suspendue.